La séance est reprise. Nous reprenons la suite de la discussion du projet de loi finance pour 2020 nous sommes parvenus dans l'examen des crédits de la mission Écologie développement et mobilité durables à l'amendement numéro 202 rectifié bis au sein de l'article 38 états B je vais demande je vais donner la parole à me ce président et blé. avez madame la présidente. Pour examiner une vingtaine d'amendements de la mission Écologie nous avons consommé une heure 20 de temps avant la pause du dîner, or il nous en reste le double, une quarantaine sur cette même mission, donc si on n'accélère pas le rythme, nous en avons pour si je compte bien 2 autant dire que c'est beaucoup, il faudrait arriver à accélérer un peu le rythme car derrière, nous avons la mission enseignement scolaire dont la DG va prendre une heure et demie et qu'il y a, elle-même, une quinzaine d'amendements à examiner,

Pour y parvenir, il faut que chacun se responsabilise essaye d'être concis et rapide dans les explications, mais je pense. Que chacun aura entendu votre message, Monsieur le Président. Bien, donc à l'article 38 états B un amendement 202 rectifié.

en 2020, d'une enveloppe budgétaire de 300 grammes millions d'euros, en baisse de plus de 6 pourcent par rapport à 2019, or cette action finance principalement l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, elle assure principalement le financement et le versement des prestations diverses, aux retraités ou aux retraités des mines fermées et de certaines mines et ardoisières en activité, il s'agit par exemple des prestations de chauffage et de logement des pensions de retraites anticipées, des indemnités conventionnelles de cessation de l'activité les crédits diminuent chaque année, mais cette baisse des crédits, donc résulter en toute logique de l'évolution démographique à la baisse du nombre d'anciens mineurs et de leurs ayants droit, que les crédits de cette agence ont été rabotés au fil des exercices budgétaires bien au-delà de l'évolution démographique et ce à des fins de recherche et d'économie budgétaire substantiel, aujourd'hui, la trésorerie de l'agence atteint désormais un niveau trop faible, les crédits alloués aux actions sociales nous paraissent suffisants pour honorer les prestations indispensables à un public de plus en plus âgés, nous estimons donc il est nécessaire que le gouvernement préserve les actions ou les moyens d'action de de cette agence, dans les années à venir, pour toutes ces raisons, nous proposons de doter les crédits de l'action quatre gestion économique et sociale de l'après mine de 20 millions d'euros, bien sûr, nous avons engagé cet amendement, madame la présidente. Merci, monsieur le sénateur, quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur défavorable Madame la Ministre, quel est l'avis du gouvernement. Merci Madame le président, mais comme monsieur le sénateur Courteau l'a très bien décrit ce sont, c'est donc un programme qui doit financer des prestations sociales et on constate tout simplement l'évolution de la démographie dans ce secteur, et donc les crédits sont ajustés en conséquence non non pas au-delà, ils sont ajustés en conséquence. Donc, avis défavorable, madame la ministre. S'il n'y a pas de demande d'explication de vote, je vais mettre aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables qui est pour son adoption. Il n'est il n'est pas adopté. Nous examinons l'amendement 153 c'est

Comme l'a expliqué très brillamment tout à l'heure de la discussion générale, mon collègue Jean-Pierre Grin, il est plus qu'urgent d'accélérer le processus de la construction de la nouvelle ligne Montpellier-Perpignan, c'est une ligne stratégique qui répond à des âges considérable d'aménagement du territoire au niveau national et européenne, la création d'une société de projets vertu de l'article 1er du projet de loi d'orientation des mobilités permet d'espérer un déblocage de la situation, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, madame la ministre est telle est l'objet du présent amendement. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la madame Exactement comme pour l'amendement précédemment défendu la programme 203 novices uniquement des crédits de fonctionnement pour P. et des coûts et donc là, vous parlez d'une extension du réseau, donc ce n'est pas le bon programme, c'est pas la bonne, maquettes, donc avis défavorable. Merci madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement. je confirme que par ailleurs, compte tenu des articles qui ont été votés dans la loi mobilité, il sera possible d'accélérer la réalisation de cette ligne, en créant une société de projet, mais ça ne nécessite pas de maître de l'argent sur le programme de S'il n'y a pas de demande d'explication de vote, je vais mettre aux voix l'amendement 211 rectifié avec 2 avis défavorables qui est pour son adoption. Il n'est Il n'est pas adopté à présent 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune le 222 rectifié c'est Monsieur crémier qui va nous présenter. Merci madame la présidente, madame le ministre, mes chers collègues, cet amendement a pour but, tout simplement en droite ligne de ce qui a été fait au Sénat, déjà dans le budget 2019 en 2018 d'inscrire une ligne complémentaire fin d'abonder la ligne qui avait été créé au Sénat pour l'accompagnement de la fermeture des 4 dernières centrales à charbon, je vous rappelle que ce choix a été confirmé dans la loi énergie-climat que ce sont 4 territoires, ce sont 4 entreprises réparties dans nos régions qui ne demandait rien d'un décidé de les fermer d'ici 2 1000 22 et qu'il est absolument nécessaire que la solidarité nationale s'exerce pour la revitalisation de ces territoires, tant au niveau des salariés qui sont concernés, tant au niveau des entreprises sous-traitance qui sont concernées, mais aussi sur ces territoires, comme on l'a fait et comme on continue de le faire madame la Ministre, sur l'accompagnement sur la fermeture de la centrale de Fessenheim ce cette proposition, a pour but, tout simplement, d'accompagner d'une manière digne ces territoires au type de la solidarité nationale, puisqu'on a fait ce choix à des fins climatique un choix je dirais qu'il n'était pas portée par ces territoires. Merci, un amendement 207 rectifié, c'est monsieur Courteau qui va nous le présenter. Oui, madame la présidente, oui, le fonds de revitalisation des territoires, destiné à financer la reconversion des territoires impactés par la transition énergétique est abondé dans cette mission de 42 millions d'euros en 2020 les territoires seront impactés par la fermeture des centrales à charbon et celle de la centrale nucléaire de Fessenheim le montant des sommes consacrées à la reconversion des 4 centrales à charbon et à celle de la centrale de Fessenheim nous paraît vous ne paraît pas suffisant notre amendement propose donc d'augmenter de 10 millions d'euros, les crédits du fonds de revitalisation des territoires, il est essentiel, nous semble-t-il, d'accompagner au mieux nos territoires dans la transition énergétique, cela passe notamment par un renforcement des aides à la reconversion des territoires concernés par la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim ou la fermeture de ces centrales à charbon, mais notre amendement a aussi une autre portée à plus long terme, l'émission de se fondre le revitalisation des territoires, devront être élargi aux territoires qui sont impactés par la transition écologique qui ne se limite pas au secteur de l'énergie, on peut notamment penser aux industries chimiques aluminium qui devront elles aussi se verdir comment accompagner et dès lors toutes les transformations à venir dans le cadre de la mise en oeuvre de la transition écologique, je cite, que nous n'avions pas d'autre choix que de réussir la transition écologique et cette fédération chiffre les besoins de financement à 50 milliards chaque année, soit 1500 milliards sur 30 ans ce prépare pardon aux bouleversements à venir qu'il faut que nous aussi nous anticipions en prévoyant sur le long terme, Anne, il y a une vision à long terme, quelques dizaines de millions d'euros ne suffiront pas, la transition écologique penser dès aujourd'hui pour le long terme, peut aussi être une chance pour l'emploi et pour les territoires, telle est le sens de notre amendement que nous avons engagée évidemment, madame la présidente. Merci, quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. c'est une vraie préoccupation, moi, je vais demander à Madame la ministre de bien vouloir nous dire quelle est la maquette, prévue pour 2020 sur la montée en charge des dispositifs d'accompagnement on peut comprendre en matière de budget que les fonds qui sont fléchés soit dépensé le mieux possible, vu les l'état des finances de la France, donc, madame la ministre, je donnerai l'avis définitif après vous avoir entendu, je vous remercie. Madame la Ministre, quel est l'avis du gouvernement. Merci madame la présidente, moi je suis comme vous évidemment attachés à ce qu'on accompagne de façon exemplaire les territoires qui sont concernés par les fermetures de centrales à charbon et c'est bien le sens des 40 millions d'euros d'autorisations d'engagements qui ont été prévues et qui correspondent au programme qui sont en cours de discussion dans chacun de ces territoires, donc les crédits nécessaires sont bien prévus à hauteur de 40 millions d'euros, plus généralement, j'entends la préoccupation qui a été exprimé d'accompagner les entreprises dans le cadre de la transition écologique le fonds chaleur peu précisément permettre d'accompagner les entreprises pour décarboner leur processus de production, par ailleurs, on a des programmes de certificats d'économie d'énergie, qui sont aussi ouverts aux entreprises et aujourd'hui il y a que 20 pourcent des certificats d'économie d'énergie qui sont utilisées au profit de l'industrie, on réfléchit également dans le cadre de la démarche pourra pacte productif à des avantages fiscaux qui pourra être donnés pour accompagner les uns vers les investissements permettant de décarboner notre production, mais en tout cas pour 2020 les crédits tels qu'ils sont prévues correspondent aux besoins qui ont été recensés pour les territoires concernés par la fermeture des centrales à charbon, donc avis défavorable sur ces deux amendements. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission, regard de ces éléments. Au regard de ces éléments et on aura l'occasion, je pense, enfin c'est pas je pense, de regarder dès le prochain budget qu'elle aura été le l'état des dépenses par rapport à ce qui est prévu, puisque pour les 4 sites, donc moi je vais m'en remettre, enfin j'ai j'ai, je propose de faire confiance, évidemment, à ce que vient de nous dire la ministre et pour cette raison, je rendrai un avis défavorable. S'il n'y a pas de demande d'explication de Monsieur et je vous en prie pour explication de vote. Oui, madame la présidente, voilà le ministre monsieur le rapporteur, chers collègues, moi je vais maintenir cet amendement pour une raison simple, c'est qu'effectivement on n'a peut-être pas eu les mêmes sources, j'ai passé beaucoup de temps, auditionné sur ce sujet, déjà l'an passé et à nouveau cette année, je peux vous assurer que les besoins, ils sont là, qu'on ne peut pas abandonner ces territoires comme nous sommes en train de le faire l'ampleur de ce qui est en train de se passer sur ces territoires en terme de conséquences économiques nécessite qu'on mobilise des moyens supplémentaires, c'est pour ça qu'à titre je, il a été cosigné d'ailleurs par un certain nombre de collègues sénatrices et sénateurs, la solidarité nationale doit s'exercer sur ces territoires, puisque ce sont des sujets qui ne sont pas délibéré par rapport à une situation problématique d'un territoire et je veux dire autre chose, je m'en excuse, je vais peut-être un peu être un peu plus long dans le temps qui me reste. Madame la ministre, si on dit la vérité aux Français aujourd'hui avec les événements qui s'est passé, qui se sont passés il y a peu de temps au niveau du séisme, avec les difficultés à juste titre de précaution de fermeture de production au niveau des centrales. Si on disait aux Français, qu'aujourd'hui, on a fait tourner à fond les les centrales charbon les centrales à fioul centrales à gaz et qu'on a dû importer du courant venant d'Allemagne, c'est un véritable sujet, je crois qu'il faut faire très attention, je crois qu'aujourd'hui on est face à quatre centrales qu'on a décidé de fermer pour des raisons purement écologique purement d'affichage au niveau national, je reviens pas dessus, madame la Ministre, je l'ai défendu avec vous, nous l'avons voté au niveau du sénat sur cette décision de fermeture de ses 4 centrales charbon et quatre dernières qui reste en France, mais notre responsabilité c'est d'accompagner d'Irène dignement ses territoires et celles et ceux qui ont vivaient. En quelques secondes, mais c'est un sujet important, moi je vais voter, c'est un moment même si après on va on on ne confirmera pas tous les amendements qu'on est en train de voter sur un point très précis qui, effectivement, on a une transition à mener cette transition oblige à fermer un certain nombre d'outils de production ou dans d'autres domaines des industries si les territoires ont le sentiment qu'ils vont être laissés seuls face à cette transition et c'est une sorte d'ailleurs du c'était au début qui a été, après qu'un peu partout dans tous les sens et qui a perdu une partie de sa signification si on donne le sentiment que la solidarité nationale n'accompagne pas ses territoires, alors à chaque fois qu'on devra prendre une décision de transition, on aura des blocages sur les territoires, donc c'est absolument essentiel, effectivement, qu'on montre qu'on accompagne fortement tous ces territoires, parce qu'on est sur une transition nécessaire. Monsieur Courteau vous souhaitiez prendre la oui. J'aurais voulu vous poser une question : est ce que je peux rectifier mon amendement. C'est à dire le le porter à 20 millions puisqu'il est aujourd'hui telle que présentée, vous voulez. Tout simplement le rendre identique à l'amendement de monsieur comme cela Si c'est possible et, ce faisant, finalement, je me rallie à l'amendement de monsieur parce que bon, les besoins qu'il a ils sont exprimées par ces territoires sont sont d'une autre ampleur que que les financements qui sont aujourd'hui prévues.

Pour qu'il y ait pas de méprise, moi je, je maintiens la position que j'ai évoquées simplement Madame la Ministre, ce que je vous demande, c'est dans un an, de nous donner un état précis

c'est pas ça le plus important, je pense que le plus important c'est de de travailler à la fois dans la sérénité et dans la transparence des chiffres voilà et je pense même que si les 40 millions prévus fin de mon point de vue venait à ne pas suffire, je pense que le gouvernement à ce moment-là, quel qu'il soit

Bien, s'il n'y a plus d'autres demandes d'explications de vote, je vais mettre aux voix, ces 2 amendements identiques, le 222 rectifié l'207 rectifié, qui est pour leur adoption.

Merci madame la présidente, Madame le Ministre, mes chers collègues, l'amendement que que je vous propose VISA à renforcer les les moyens financiers nécessaires à la surveillance de la qualité de l'air à l'information et à l'évaluation des des actions pour lutter contre la pollution de de l'air et en protéger, comme vous le savez, une bonne surveillance de la qualité de l'air est un est un préalable indispensable à l'action, tout comme la la sensibilisation et l'information de la population, ses missions de surveillance et d'information a été confié en France à des associations agréées de surveillance et et de qualité de l'air, les AASQA, qui existe en France depuis, depuis 40 ans et qui reçoivent un agrément ministériel, il vous est proposé, donc de transférer 5 millions d'euros de dotation supplémentaire en autorisation de d'engagement aérien en crédits de paiement en faveur de l'action 5 du programme 100 60 14 aujourd'hui en France, le, le, l'État ne finance ces associations régionales qu'à hauteur de 22 centimes par habitant et par an en moyenne c'est un amendement qui vise à porter ce financement à 29 centimes par an et par habitant. Merci, quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur.

qui exerce une mission de service public sous forme associative, pour le compte de l'État, on a vu d'ailleurs l'importance du travail réalisé sur l'incendie Lubrizol puisque une partie non négligeable des temps de d'expertise, à la fois techniques et scientifiques sont faites par les donc madame la ministre, je pense que vous allez rassurer notre collègue Stéphane Piednoir sur les montants suffisants, programmée pour l'année 2020 pour les associations agréées sur Jacques et d'de l'air parce que ça revient souvent, et il faut toujours jongler, ce qui à mon avis, est un peu dommage, d'autant qu'on reste sous le coup de d'contentieux européens dont la France n'est pas sorti et ça remonte maintenant une décennie. Quel est l'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Merci madame président alors vous proposez de baisser les crédits du programme de prévention des risques après l'accident Lubrizol je peux naturellement pas être d'accord avec l'idée de baisser les crédits consacrés à la prévention des risques et s'agissant des crédits des Afcae évidemment, le gouvernement est très attaché à la qualité de l'air et améliorer cette qualité de l'air, c'est bien pour ça que, depuis 2016, les crédits alloués aux qui sont par ailleurs co-financé par les collectivités n'ont pas baissé et je voudrais aussi souligner que par ailleurs nous menons des nombreuses actions pour améliorer la qualité de l'air, il y a notamment un programme de 140 millions d'euros sur géré par l'ADEME, le fonds air-mobilité qui permet, notamment, pour 35 millions d'euros d'accompagner des territoires concernés par des dépassements de normes pour les particules fines et les oxydes d'azote et puis j'ajoute enfin que dans la loi mobilité, vous avez voté la création de zones à faibles émissions qui vont donc pouvoir se mettre en palace, y compris avec des dispositifs de contrôle adaptés, donc je pense que non seulement on agit pour soutenir les ASCA pour mesurer la qualité de l'air, mais par ailleurs on agit aussi pour améliorer la qualité de l'air au travers des différents dispositifs que j'ai évoquée donc avis défavorable. S'il n'y a pas de demande d'explication de vote, je vais mettre aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables qui est pour son adoption. Moi qui est contre.

il est adopté. à présent, nous examinons 3 amendements qui font l'objet d'une discussion commune le 125 rectifié monsieur Dantec va nous présenter. Merci, c'est un amendement qui vient en soutien dans des des joyaux français de la protection de la biodiversité qui est notre grand réseau de réserve naturelle nationale à ne pas confondre avec nos parcs nationaux, les parcs nationaux sont sous la responsabilité de l'État avec du du, du personnel de l'État, les réserves naturelles sont en gestion souvent par des associations avec des contrats avec l'État, ce qui est l'occasion de redire Madame limite j'ai bien entendu ce que vous avez dit tout à l'heure à la fin de la de la discussion générale concernant le maintien des effectifs des parcs nationaux, je reconnais que ce n'est pas du tout ce qui nous remonte d'un certain nombre de parcs nationaux, mais j'ai bien entendu à votre explication que nous essaierons de recroiser des informations, de toute évidence divergentes sur le le maintien des effectifs des parcs nationaux concernant donc le le réseau de réserve naturelle nationale qui joue un rôle important sur la biodiversité, avec de vrais résultats alors que la biodiversité, par exemple, des oiseaux, les populations s'effondrent en France, elles ont augmenté dans les réserves naturelles, hein, où il y a souvent des des espèces rares et il faut savoir que donc depuis 2012, il y a bientôt 10 ans, elles n'ont vu aucune réévaluation de leur dotation alors que pourtant on leur a demandé d'aller sur d'autres sujets, en plus de la gestion directe des réserves notamment toutes les questions de sensibilisation et d'éducation à la nature, ce qui veut dire que les salariés eux-mêmes depuis 2012 n'ont pas été revaloriser, donc il est temps de donner un signal vers les gestionnaires de ces réserves un vers ce réseau extrêmement important qui complète notre réseau de de parcs nationaux d'où cet amendement qui propose donc de doter ce réseau des réserves naturelles nationales de 2 millions d'euros supplémentaires.

je tiens à dire que c'est un amendement que j'avais déjà présenté l'année dernière, qui n'avait pas passé le stade de la de la commission, mais cette année, j'ai des j'ai décidé de le le présenter en séance parce que il y a quand même un enjeu on on a un souhait et et une volonté du président de la République qui a été affiché encore en en mai dernier, annonçant qu'il fallait augmenter globalement de 5 réserves naturelles par an le le cheptel des réserves naturelles, sauf que les crédits baissent chaque année, donc il y a une petite contradiction entre le fait qu'on veuille porter qu'on va y porter des, des, des éléments ambitieux et peut-être une stagnation voire une baisse des crédits, donc il faut être attentif, donc je, je tiens à le présenter et puis, il y a aussi un élément complémentaire c'est que Madame le la présidente, je vais parler pour vous, je me permettrais puisque vous défendez vous-même une réserve en Alsace qui est la réserve de la petite couronne alsacienne qui est située dans le dans qui est situé dans la bon et et donc la petite couronne alsacienne qui est qui est défendu par la présidente Catherine Tremblay dans le même esprit de ce que je défends Hauts-de-France nos réserves naturelles nationales, donc je sais que que le rapporteur a émis un un avis en commission parce que c'est pas un sujet qui est facile, mais je pense qu'il est, il est vraiment à prendre en compte, en tout cas, même s'il n'est pas adopté cette année, je le redéposera l'année prochaine. Pour rectifier un tout petit peu, c'est la petite Camargue en Alsace. Je vais vous avouer que je n'ai pas mais mes lunettes de vue de près. Un amendement 179 qui n'est pas soutenu monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission sur ces amendements. l'avis de la commission, il y a, il y a d'abord 2 sujets : le 1er c'est que les montants, les amendements ne se correspondent pas complètement puisque les montants sollicités pour le budget 2020 ne sont pas les mêmes, moi je vais rendre un avis de sagesse madame la la ministre pour une raison simple, c'est que la biodiversité est aujourd'hui dans les est, vous prenez la dernière enquête sur les attentes des Français en matière de préoccupations environnementales, la première attente c'est pas une surprise et ça continue de monter à plus de 50 pourcent c'est la lutte contre le changement climatique et pour la première fois depuis longtemps la 2ème attente et la lutte contre la biodiversité, alors en général on pour pardon oui. ça démontre que quand je fais une erreur, vous savez moi rectifier. Et vous êtes attentif mais je, je vais continuer, c'est un, c'est un vrai sujet d'autant que dans la biodiversité, on oublie souvent que plus de 50 pourcent de la biodiversité, c'est dans les sols et comme on en a parlé tout à l'heure, je pense qu'il y a des moyens à à mobiliser et honnêtement les moyens mobilisés à hauteur de 10 millions d'euros pour l'année 2020 paraissent je l'ai effectivement dit dans le leur, que j'ai rendu paraissent notoirement insuffisant, d'autant qu'une part non négligeable de ces crédits Servent pour enfin serviront pour le congrès mondial qui va avoir lieu à Marseille donc mobiliser davantage de fonds au profit de la biodiversité, me semble aujourd'hui nécessaire, indispensable, et contrairement aux autres avis je propose la sagesse. Madame la Ministre, quel est l'avis du gouvernement. Merci madame la présidente, l'avis du Gouvernement est défavorable parce que les crédits consacrés aux réserves nationales ne baisse pas, il y a 163 réserves et 23 millions d'euros sur le programme 113 pour financer ces réserves, il est prévu de créer 20 réserves supplémentaires et les crédits correspondants seront inscrits au fur et à mesure, donc notamment 500000 euros pour la création de ces vins réserve complémentaire, un abondement automatique au fur et à mesure de la création des réserves, donc je pense que les crédits sont suffisants : avis défavorable. S'il n'y a pas de demande d'explication de vote oui monsieur Dantec, je vous en prie. Mais si les crédits ne bouge pas, il ne bouge jamais il baisse, donc ça n'est pas ça n'est pas des crédits totalement maintenu, c'est des crédits qui baissent peu à peu chaque année, j'ai bien entendu mal la mise pour les nouvelles réserves il y a une dotation supplémentaire, pour le réseau de réserve depuis 2002, alors qu'on demande alors gestionnaire de plus en plus d'actions et d'actions légitimes, notamment de sensibilisation d'accueil du public d'accueil des jeunes, ça veut dire qu'en fait par rapport à la charge de travail qu'on leur demande on est en baisse légère, année après année, donc moi pour pour qu'on ait un vote assez unanime parce que ce sont bien un potentiel compte Sansus dans notre assemblée, j'ai retiré mon amendement et pour montrer qu'on est raisonnable

le réseau national demandé bien de passer de 23 millions 25 millions donc des 2 que je proposais, c'est la demande du réseau national mais je propose qu'on vote au moins 800000 qui est un signal et puis effectivement, je pense que du coup vous entendrez ce ce signal est notre préoccupation. l'amendement 125 rectifié retiré à la demande de Monsieur Dantec et je vais mettre aux voix l'amendement 109 rectifié avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du gouvernement qui est pourcent adoption. pourcent adoption. Il est adopté. Nous examinons à présent l'amendement 124 rectifié, c'est monsieur Dantec qui nous le présente. Oui, c'est un amendement qui fait évidemment tout à fait écho à la à l'actualité actuel et à ce qui s'est passé avec la l'accident majeur de de Lubrizol en 2018, 18200 visites ont été un effectué par les les inspecteurs des installations classées en 2009, il y en avait 22000 alors qu'on sait très bien que la préoccupation sur les enjeux environnementaux ont depuis plutôt augmenté, donc on a un véritable problème aujourd'hui de suivi des installations classées, nous le savons et donc cet amendement propose que le budget un permettent de créer une trentaine de postes supplémentaires d'inspecteurs des installations classées, très honnêtement, madame la Ministre, ça n'est pas du luxe par rapport à l'enjeu en France et c'est toujours c'est c'est de l'argent qui est investi en amont et, derrière, c'est beaucoup de conséquences et de drames ou de conséquences environnementales éviter donc c'est généralement de l'argent très bien investi. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. puisque j'ai relayé comme Ronan Dantec les préoccupations à la fois en réaction évidemment à l'incendie de Lubrizol mais également parce qu'il faut pouvoir commencer à se projeter sur l'avenir, on va voir ce que vous nous dites, Madame la Ministre, moi je pense, si on veut être raisonnables, il y a une mission d'information à l'Assemblée nationale, il y a une commission d'enquête au Sénat, on va voir donc le les conclusions et les propositions à la fin du 1er trimestre 2020, ce qui veut dire qu'en fonction de ses conclusions et notamment si il est les 2 assemblées, font des propositions pour renforcer parce que on observera des carences ou à d'autres endroits, des simplifications, je pense qu'on peut honnêtement se dire qu'à défaut de le budgétés pour 2020 et sous réserve qu'Emmanuel Rist vous nous confirmiez, bien qu'il n'y a pas de réduction, on pourrait imaginer qu'en 2021, enfin en 2020 soit prévue une nouvelle maquette pour qu'en 2021 sur le budget, il y a des recrutements progressivement supplémentaire parce qu'il faut aussi avoir les profils correspondants, mais je ne doute pas madame la vie ce que vous allez nous donner de nombreuses garanties. Madame la Ministre, quel est l'avis du gouvernement. Qui est l'année de l'accident d'AZF, il y avait 848 équivalents temps plein sur les missions des installations classées en 2018, il y en avait 1300 donc, les effectifs ont été très significativement renforcés après l'accident d'AZF et je me suis engagé à ce que les effectifs ne diminuent pas en 2020, ça fait partie des missions prioritaires qui ne nous voilà n'auront pas de diminution d'effectifs, il est exact que le nombre de contrôles a baissé ces dernières années mais c'était lié notamment à l'élaboration des PPRT qui ont également été décidées suite à l'accident d'AZF, heureusement on arrive au bout, hein, d'élaboration de ces PPRT et l'objectif, c'est qu'on augmente de 50 pourcent les contrôles des installations classées, d'ici 2000 22 ans, voilà en redonnant de la disponibilité à nos inspecteurs qui seront moins accaparé par la réalisation de ces PPRT, donc je pense que ces effectifs permettent de répondre aux enjeux et je vous propose le retrait sinon avis défavorable. Monsieur Dantec, je vous en prie. Oui pour dire que le le le raisonnement, la proposition Jean-François Husson est effectivement tout à fait logique donc je vais je vais retirer c'est cet amendement et nous aurons l'occasion avec la la commission d'enquête avec Madame la Ministre de de refaire le point juste pour dire que c'est vrai que les effectifs n'ont pas baissé que le sentiment qu'on peut déjà en avoir sans sans aller tout de suite sur les conclusions de la commission d'enquête, c'est qu'on avait quand même un certain nombre d'années après AZF, commencer à rebaisser la garde sur cette question du risque d'accident industriel, y compris dans la culture des territoires et les responsabilités sont aussi partagées et que donc je crois que cette année, doit nous servir à à reconstruire une doctrine pour éviter d'autres accidents de type Lubrizol mais je retire l'amendement. Bien, par conséquent, le 124 rectifié et retiré à présent nous examinons 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune le 206 et j'invite monsieur Courtois nous présenter. Merci madame la présidente, oui, alors au vu des des enjeux actuels le rôle d'et et les missions de l'Autorité de sûreté nucléaire ne cesse d'évoluer à titre d'exemple, l'ASN n'aura dans les prochaines années à se positionner sur le contrôle lui seulement et la durée de fonctionnement des réacteurs électronique. Le contrôle de la mise en un service de l'EPR, l'encadrement et le contrôle du démantèlement des réacteurs électronucléaires l'encadrement et l'analyse des réexamens de sûreté des installations exploitées par Areva et le CEA, l'instruction des dossiers réglementaires des nouvelles installations réacteur Jules Horowitz et Cigéo et autant de dossiers qui demanderont un investissement dès lors il semble pertinent d'augmenter le nombre d'équivalents temps plein, au sein de l'ASN cette proposition s'inscrit dans la continuité de l'avis de l'ASN, en date du 1er juin 2017 qui demande 15 équivalents temps plein supplémentaires pour le triennal 2018, 2020 et d'une recommandation émise dans le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires publié 1 juin 2018, qui préconise une augmentation de 13 équivalents temps plein d'ici 2020 réparties entre les budget 2000 19 et 2020. Afin de faire. Accroître l'effectif de l'ASN, de 9 équivalents temps plein, lui permettant d'atteindre l'objectif de 15 équivalents temps plein supplémentaires sur le triennal 2018, 2020, cet amendement augmente de 800 10000 euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement alloués aux dépenses de personnel titre de de l'action 9, contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection du programme 181 et bien entendu, nous avons engagé cet amendement.

de disposer des crédits nécessaires la couverture complète de ses dépenses en personnel, en effet, l'AS et l'ASN est confronté depuis 2018 à un problème de sous-budgétisation des crédits des titres de par rapport aux créations d'emplois obtenus par l'autorité en 2017 en exécution ce décalage conduit donc depuis 2018 à un report des charges au détriment d'autres dépenses de fonctionnement sur le titre III pour continuer à rembourser l'intégralité des conventions de mise à disposition pour remédier à cette sous-budgétisation chronique et signalé de 2018 le présent amendement et bien entendu gagé d'une diminution de crédits imputé à l'action 5 et augmentent du même montant, les crédits à l'action 9, contrôle de la sûreté nucléaire, de la radioprotection programme 181, prévention des risques, je vous remercie. Merci monsieur rapporteur, quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements. Alors 2 amendements sur un même sujet pour l'un et l'autre, c'est pas les mêmes montants qui sont demandés, moi je vais vous faire retour des de l'audition, qu'on a eue avec l'Autorité de sûreté nucléaire qui sollicitait qui avait obtenu du gouvernement une revalorisation triennal de 2 postes par an à l'Assemblée par amendement, c'est passé à 5 postes, la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire. C'est de d'avoir 5 postes chaque année, moi ce que je peux vous dire c'est que, en l'état actuel, les 5 postes étant obtenu cette à prendre en compte et je vais également porter à votre connaissance que nous exerçons actuellement, enfin nous avons missionné dans une mission de contrôle le type du 58 2 la Cour des comptes sur les opérations de démantèlement des centrales nucléaires, le nous aurons le les conclusions seront rendues le rapport sera rendu au début du printemps ou à la fin de l'hiver et nous aurons à mon avis, à ce moment-là, d'autres éléments qui nous permettront d'apprécier en dehors du point de vue de la seule autorité de sûreté nucléaire parce que je ne veux pas me limiter à cette demande une appréciation plus complètes sur les besoins éventuels et supplémentaire qui pourrait se faire jour, donc avec ces explications, je crois que je proposerai un avis défavorable. Madame la ministre qu'est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements. Merci madame la présidente, même avis : moi, je voudrais rappeler que l'ASN a bénéficié de 10 créations de postes en 2016 de 30 en 2017, le projet de loi de finances, telle qu'il est entré à l'Assemblée nationale prévoyait, comme vient de le dire, monsieur le rapporteur, de création de postes supplémentaires, les députés ont rajouté 5 postes. Avec les crédits correspondants, donc je pense qu'on est sur une trajectoire voilà de renforcement de l'ASN qui me paraissent satisfaisantes et aller au-delà se ferait nécessairement au détriment d'autres missions du ministère, donc avis défavorable. Je vais mettre aux voix l'amendement 206 avec 2 avis défavorables qui est pour son adoption.

Très bien monsieur Courteau vous maintenez votre amendement donc je remets aux voix l'amendement 206 avec 2 avis défavorables qui est pour son adoption. Qui est contre,

Oui, cet amendement vise à élargir le le Champ de compétence du médiateur de l'énergie afin qu'ils puissent prendre en charge un dispositif de médiation des litiges liés à la rénovation énergétique des bâtiments à la loi relative à l'énergie et au climat, récemment votée permet d'instaurer des dispositifs pour lutter contre les fraudes sur le marché des certificats d'économie d'énergie, mais également pour éradiquer les passoires thermiques en 10 ans, de façon progressive, l'agitation à la rénovation, obligation de performance énergétique des logements, interdiction de la mise en location ces avancées s'inscrivent dans la continuité de la fiabilisation du diagnostic de performance énergétique et du développement du carnet numérique des bâtiments instauré par la loi mais mais afin de parvenir réellement massifier les travaux de rénovation énergétique et atteindre ainsi le niveau bâtiments basse consommation pour l'ensemble du bâti à l'horizon 2050, il est essentiel de lutter contre les pratiques abusives, en effet, la DGCCRF a récemment dénoncé des pratiques peu sérieuse et les arnaques dans ce domaine, faute de disposer d'une aide à et d'une alternative à la voie judiciaire souvent l'homme et coûteuse, les consommateurs perdent souvent le bénéfice des aides à la rénovation Cide prime transition énergétique, c'est eux qu'ils escomptaient et se retrouvent victimes de travaux de mauvaise qualité ou dans une situation financière difficile afin d'assurer le bénéfice des aides à la rénovation énergétique plus simple, plus juste et plus efficace par le projet de loi de finances pour 2020, il semble essentiel de pouvoir proposer un de pouvoir proposer un service neutre et le vient de médiation de ces litiges, c'est dans l'objet du présent amendement qui vise à élargir le Champ de compétence du médiateur de l'énergie aux litiges relevant de la rénovation énergétique des bâtiments, et cela se traduit donc par la création de 2 équivalents temps plein supplémentaires pour analyser la recevabilité des litiges, informer et orienter les consommateurs dans les 10 je ne serais pas recevable et instruire à médiation ce qui serait effectivement recevable la masse salariale de ces 2 équivalents temps plein, ainsi que le budget de fonctionnement associés suis la base des hypothèses précédemment mentionnés nécessiterait d'augmenter de 200000 euros, le budget du médiateur de l'énergie, raison pour laquelle notre amendement propose d'augmenter le budget du médiateur national de l'énergie de 200000 euros. Merci, quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. C'est un avis défavorable je pense mon cher collègue, qu'il est préférable de travailler notamment avec les plateformes de rénovation énergétique c'est-à-dire, c'est-à-dire non pas dans la réparation mais en amont et d'améliorer le conseil et je pense que, avec un travail étroit Ademe Agence cas de l'énergie, c'est là où on doit renforcer la, je dirais, le niveau de compétence, notamment pour faire diminuer ce que vous évoquez les cas de de contentieux. Madame la Ministre, quel est l'avis du gouvernement. soutenir la mise en place de ces plateformes de conseils et d'accompagnement par ailleurs nous avons fortement renforcé le contrôle des ses 2 E le contrôle des certification RGE et par ailleurs, la DGCCRF a également renforcé ses contrôles sur le démarchage abusif que l'on peut observer sur un certain nombre de travaux de rénovation énergétique, j'ajoute que je pense que ça serait une fausse bonne idée de confier au médiateur de l'énergie qui est habitué à gérer les relations entre beaucoup de clients de peu d'énergéticiens, un rôle de médiation dans le domaine de la rénovation énergétique qui s'apparente beaucoup plus à la mission de de médiation dans le domaine du bâtiment, étant entendu qu'en plus on a un nombre très important d'acteurs, donc ça n'est absolument pas le même métier, donc pour toutes ces tous ces raisons avis défavorable. Je vais mettre aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables qui est pour son adoption. Qui est contre. Il n'est pas adopté l'amendement 192 c'est monsieur Gillet et qui va nous présenter. les 16 au centre de sécurité des navires CSN répartis sur le littoral français ont pour mission de contrôler les navires sous pavillon français, de même que les navires étrangers en s'assurant qu'ils respectent bien les normes sociales, environnementales et de sécurité, il joue notamment un rôle fondamental dans la lutte contre la pollution atmosphérique due au transport maritime en contrôlant le respect par les navires des normes internationales et européennes relatives à la teneur en soufre des carburants marin, le projet de loi de finances pour 2020 prévoit une baisse de leurs crédits de fonctionnement, lesquelles sont fixées à 1,1 1000000 d'euros en 2020 contre 1,21 millions d'euros en 2019 cette diminution des crédits est particulièrement mal venue en effet au 1er janvier 2020 entrera en vigueur une nouvelle norme internationale limitant à 0,5 pourcent la teneur en soufre des carburants marin contre 3,5 pourcent un telle durcissement de la réglementation vertueux pour la réduction de la pollution due aux navires-doit s'accompagner d'un renforcement transitoire c'est non permanent des contrôles effectués par les services de l'État, il est donc impératif que ces analyses en laboratoire devienne effective partout sur le territoire, à compter du 1er janvier 2020 pour donner au durcissement des normes toute sa portée, en effet, ces analyses permettent aux services de l'État de confirmer l'infraction et de la signaler au procureur, or précisément, il y aura 110000 euros de crédits en moins cette année pour financer le fonctionnement du CSN, en particulier les analyses en laboratoire, comment les CSN pourront-ils amplifier leur contrôle avec un budget en diminution, cet amendement prévoit donc d'abonder l'action sécurité et sûreté maritimes du programme 205 affaires maritimes sous-actions de contrôle des navires à hauteur de 150000 euros, ceci afin de permettre au CSN de poursuivre et d'amplifier leur contrôle bien évidemment cette demande. madame le rapporteur, quel est l'avis de la commission. Oui, merci, alors il me semble que ce cela résulte d'une erreur, peut-être un peu rapide des documents budgétaires, puisque donc effectivement dans le pape pour 2020 nous avons une ligne qui est de 1 1000000 100 de crédits pour les crédits de fonctionnement descend de sécurité des navires mais juste en dessous, nous avons une autre ligne pour 350000 euros, qui s'appelle action internationale et qui porte plusieurs dépenses, à savoir les adhésion annuelle aux 3 réseaux régionaux et le maintien en condition opérationnelle de la base Gina donc pourquoi est ce que je vous dis ça, parce que si j'aime, on va regarder le pape le rap, pardon de l'année 2018, donc ils sont les derniers crédits qu'on connaît, dépenser, 1000000 0 20 de crédits de paiement consommer qui portait à la fois 777000 euros de dépenses de fonctionnement, donc pour les 100 de sécurité, plus de 250000 euros de crédits pour les marchés publics d'analyses et de prélèvements des combustibles, la cotisation au mot de l'océan Indien et l'exploitation et la poursuite du développement du système d'information Gina donc si en fait, on regarde un 1000000 0 consommer 2018 et qu'on additionne les 2 lignes de 1000000 100 plus 0 plus de 350000 on a des crédits qui sont plutôt en fonction en croissance, donc là rien ne me laisse à penser que les crédits sont en diminution, donc c'est un avis défavorable. Quel est l'avis de du gouvernement, Madame la Ministre. Tout est dit, mais Je vais mettre aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables qui est pour son adoption. Qui est contre, il n'est pas adopté. Nous allons procéder au vote des crédits de la mission Écologie développement et mobilité durables figurant à l'état B je n'ai été saisi d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite, par conséquent je mais on voit les crédits de la mission qui est, pour leur adoption.

et 76 qu'acquiesce et les amendements portant articles additionnels qui seront rattachés pour leur examen aux crédits de la mission Écologie développement et mobilité durables à l'article 76 je. La parole est à Madame Éliane Assassi. Je vous en prie, chers collègues. Nous sommes convaincus de l'utilité de la reprise de la dette à ce que nous regrettons simplement ce sont les conditions de cette décision, je rappelle que cette reprise de la dette et le Coran au corollaire du changement de statut de la SNCF et la SNCF en société anonyme, puisque chacun sait qu'une société anonyme ne peut porter une telle dette, il s'agit donc d'une décision en réalité purement comptable, alors si nous voulions faire les oiseaux de mauvais augure, nous parlerions même d'un cadeau pour les futurs acquéreurs de la société anonyme à 100 pourcent public puisque tout le monde sait qu'elle ne restera pas 100 pourcent public sinon, bien évidemment, ce changement de statut était inutile pour cette raison, nous avions demandé la possibilité de rompre ses actions incessibles ce qui a été refusé, depuis l'adoption du projet de loi qui a marqué un pas supplémentaire dans la libéralisation du rail, le démantèlement de l'entreprise publique et le désengagement de l'État, nous avons étudié la qui fait de la route, la meilleure alternative au train, tout cela est décidément bien cohérent depuis également un énième rapport de la Cour des comptes pointe les cheminots, il estime ainsi que la SNCF je suis devra, dans les années à venir poursuive sa politique de réduction des emplois au même rythme qu'en 2017 soit 2000 emplois à temps plein, il appelle particulièrement à des coupes chez SNCF réseau donc, quand on voit le travail immense de rénovation ferroviaire à produire ce rapport est juste excusez-moi d'expression délirant, comment ne pas voir également que cette politique de réduction de postes à porter les germes de la dégradation du service public et porte des risques lourds pour la sécurité, nous souhaitons pour notre part au contraire plus de personnel dans les trains pour éviter des accidents, comme par exemple celui du 16 octobre dernier, mes chers collègues, ce projet de loi de finances en témoigne. C'est encore loin des enjeux de de développement des transports collectifs et du service public ferroviaire et croyez bien que nous le regretterons et nous continuerons à être aux côtés des cheminots pour que vive le service public ferroviaire. La parole est à madame Angèle Préville. Merci madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je prends la parole à à ce moment pour exprimer un sentiment général par rapport à ces crédits effondrement des espèces massif dramatique marqueur de notre présence sur terre, on n'a jamais autant parlé de biodiversité et elle n'a jamais été aussi menacée que maintenant la baisse s'accentue, s'emballe, les chiffres sont consternants crimes contre la vie qui Crime contre l'avenir, comme le dit l'astrophysicien Nicolas Barrot, où allons-nous tristesse infinie de cette multitude d'espèces qui s'éteignent ce chatoiement de la nature dont notre génération aura effacer à jamais la présence sur terre. Il est clair qu'il nous faut faire différemment, ne pas attendre les préjudices aux écosystèmes pour réagir, ne pas courir après les catastrophes pour juste panser les plaies, nous devons être capables de exister avec notre puissance, comme le dit Hubert Reeves nous sommes face à une situation inédite dans l'histoire de l'humanité, l'enjeu ultime étant notre existence même. Espèces menacées comme les autres, l'important n'est pas d'être optimiste ou pessimiste, c'est d'être déterminé, c'est d'enclencher des politiques à la hauteur et de mettre des moyens pour une politique environnementale ambitieuse, c'est-à-dire que notre responsabilité : responsabilité devrait être régulé davantage changer les lois réinterroger les objets de recherche, les investissements pour une transition économique en miroir à la transition écologique bref osé mettre en cause nos priorités nos habitudes et peut-être certaines de nos valeurs, je ne sais pas si il nous faudra faire des sacrifices, mais une chose que je sais, c'est que cela passera par l'acceptation de nos concitoyennes et concitoyens des changements nécessaires et certainement par une politique plus transparente et plus simple, il nous faudra aussi lutter contre l'amnésie environnementale, largement répandue, cette forme de délitement dans notre rapport à la nature cette extinction de l'expérience de la nature et s'ajoute à cela un paradoxe : le mal de terre où l'éco-anxiété et notre impossibilité à cristalliser un changement véritable or nous continuons Business S. Usual l'accord de Paris n'est pas contraignant, il montre le chemin, prenons-le, il est temps, les gaz à effet de serre continuent d'augmenter la biodiversité 10 mais il faut conclure chers collègue il faut conclure, nous n'avons pas encore vraiment commencé la dimension écologique. Madame privilège quand même vous rappeler que nous étions sur une prise de parole sur l'article 76 qui porte sur la SNCF. Donc à présent la parole, la parole est à monsieur Olivier Jacquin, une prise de parole sur l'article 76. Prise de parole brève car lors de la discussion générale, Madame le Ministre, je vous ai posé une question très précise relatives au budget de SNCF, réseau, nous parlons là du désendettement de la SNCF j'ai salué dans cette même discussion générale la reprise de la dette de la SNCF, comme c'était prévu dans le nouveau pacte ferroviaire je salue aussi la trajectoire croissante du budget de la AFITF, j'ai déploré que le budget de la FIT ne soit pas bien connu en ce moment, idem pour SNCF, réseau, vous nous dites qu'il y a 3 milliards en 2019, le rapporteur spécial, vous a rappelé qu'au budget de la fille, il a déjà manqué plus de 200 millions d'euros, or cette année, la rapporteur spécial, vous a dit aussi que nous avions des informations relatives au budget de SNCF, réseau qui nous inquiéter puisque selon certaines sources, et moi je ne parle pas de la presse, des sources sérieuses au conseil d'administration, il manquerait 254 millions d'euros en investissement pour permettre la régénération du réseau, une autre source indique près de 400 millions d'euros, plus précisément, 345 millions d'euros, j'ai besoin, nous avons besoin de votre réponse hier l'endettement réseau aujourd'hui, c'est la régénération impossible du réseau qui risque de l'étouffer, car vous nous l'avez avoué tout à l'heure, il n'y aura pas de débat sur les petites lignes ferroviaires, nous n'aurons pas le rapport Philizot qui est porté aux régions et donc en permanence SNCF réseau risquent d'être mises la tête dans l'eau et ne pas avoir l'espace nécessaire pour réussir à régénérer le réseau et offrir des sillons plus économique. Merci madame la présidente, alors moi je ne sais pas, quelles sont vos sources, monsieur le sénateur, mais je peux vous confirmer que le budget de la SNCF, réseau sera adopté demain et nous n'avons pas fait cette réforme pour ne pas tenir nos engagements ce budget il prévoira plus de 6 milliards d'euros investis par SNCF réseau en 2020, je pense que nous n'avons pas à rougir des comparaisons internationales, nous avions annoncé un investissement de 3,6 milliards d'euros par an pour régénérer le réseau cet engagement sera strictement tenu le budget 2020 prévoit effectivement une augmentation de 91 millions d'euros par rapport à 2019, dont plus de 23 millions sur la régénération des voies, donc je pense que ceux qui soutiennent qu'il manquerait 400 ou 500 millions d'euros au mal lu les comptes de SNCF, réseau.

Qui est contre, il est adopté, après l'article 76 un amendement 197 c'est monsieur Courteau qui va nous représenter. En 2018, madame la présidente, la quasi-totalité des chèques l'énergie ont été utilisées pour payer des factures sur 3,6 millions de chèques l'énergie consommée, seuls 843 soit 0,0 2 pourcent ont été utilisés pour participer au financement des travaux forcés de souligner que le montant du chèque énergie en moyenne est de 200 euros par an, et déjà insuffisant pour faire face à la hausse régulière des prix de l'énergie, nombreuses sont dans les ménages un situation de précarité qui sont contraints de réduire leur consommation d'énergie de chauffage pour réduire leurs factures, selon le rapport annuel de 2018 du médiateur de l'énergie, les ménages en précarité qu'on le sacre en moyenne 1925 euros par an en énergie contre 1584 par an en moyenne nationale, on comprend donc aisément les raisons pour lesquelles le chèque énergie est en grande majorité, utilisé pour payer des factures, or le PLF pour 2020 dans son article 4 pour les foyers modestes, le crédit d'impôt pour la transition énergétique en prime immédiatement perceptible dès le début des travaux, et cette prime devrait permettre de financer pour partie des travaux de rénovation énergétique, elle sera distribuée d'ailleurs par l'Anaes, ne serait-il donc pas pertinent au vu de cette réforme proposée par le PLF pour 2020 de recentrer le chèque énergie sur le paiement des factures d'énergie, puisque je le rappelle, seulement 0,0 2 pourcent des bénéficiaires ont utilisé ces financements pour la rénovation thermique et je rappelle encore une fois que la dépense des ménages modestes et de plus de 1000 900 euros en moyenne par an et que le chèque en moyenne et de l'ordre de de ça et un petit peu plus par un aussi. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. J'ai bien entendu ce que ce qu'a dit notamment à la fin, le sénateur Courteau pour 0,0 2 pourcent vu le faible nombre de dossiers, je ne vois pas l'utilité de restreindre la liberté laissée les Français faire ce qu'il souhaite et puis s'ils sont à peine mis là-bas, c'est mieux que rien, voilà donc moi je suis plutôt pour une liberté plus large, je suis étonné de voir que vous restreignez liberté d'utilisation des chèques énergie donc avis défavorable pardon. Quel est l'avis du gouvernement, Madame la ministre. Même avis madame la présidente, moi je pense qu'il faut faire confiance aux Français qui utiliseront voilà selon leurs souhaits, le chèque énergie qui leur est proposé. vous maintenez votre amendement monsieur Courteau vous le retirez je vous remercie. L'amendement 172 rectifié monsieur Lafond va nous le présenter. Oui, madame la présidente, il porte aussi sur le chèque énergie et en fait consiste tout simplement à ce qu'une évaluation de ce chèque énergie soit faite et rendue publique chaque année en effet, on sait que le gouvernement a utilisé assez massivement le chèque énergie l'année dernière pour sortir de la crise sociale ce chèque énergie présente bien des avantages, notamment dans la distribution de pouvoir d'achat de simplification, néanmoins il interroge aussi sur son efficacité et c'est pour ça que nous demandons, cette évaluation efficacité au au, au regard de de l'aide apportée, on sait qu'elle est inférieure à ce que pouvaient bénéficier certaines familles ont précarité avant on on sait aussi, et, et c'est un chiffre qui devrait nous alerter qu'en 2018 le le nombre d'impayés s'est augmenter malgré la mise en place du du chèque énergie et que du coup les les coupures à la demande des fournisseurs ont été des coupures d'électricité ont été elles-mêmes en augmentation, c'est le médiateur national de l'énergie qui ont fait le constat, donc tout ça pour dire qu'il serait bon d'avoir une évaluation de ce chèque énergie. Un porteur qu'il est l'avis de la commission. c'est un avis défavorable, bon, d'abord c'est un dispositif qui débute, on a les chiffres chaque année, moi je pense que ce qu'on peut faire, c'est d'ailleurs tenir un tableau

je suis plutôt pour la continuité dans les missions d'évaluation de contrôle donc l'engagement, en tous les cas que je prends en ce qui nous concerne aujourd'hui au titre de la commission des finances, c'est d'avoir un tableau exhaustif demander des renseignements, on peut travailler ensemble, on se met d'accord sur l'ensemble des et des données que vous souhaitez sur l'utilisation du chèque énergie c'est la proposition, je vous fais ce qui permettrait en plus pour vous d'avoir les éléments éventuellement de retirer votre demande d'amendement. Madame la Ministre, quel est l'avis du gouvernement. Merci madame la présidente, moi je vous confirme que le gouvernement se tient à la disposition du Parlement pour fournir toutes les informations sur le chèque énergie ou tout autre sujet, sans qu'il soit nécessaire de l'inscrire dans la loi, donc je vous propose le retrait. Monsieur Lafont pour explication de vote. Sous cette double proposition concordantes, évidemment je vais retirer mon amendement et donc je me joindrai à l'élaboration de, de, de ses tableaux, sur la base des données fournies par le ministère. Toujours après l'article 76, 2 amendements identiques qui font l'objet d'une discussion commune qui ne sont pas soutenus, les suivants non plus, et enfin les 2 suivants non plus et nous arrivons à l'amendement 167 rectifié, c'est monsieur Lafond qui va nous présenter. Le 167 rectifié. Merci, quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, qu'elle est l'avis du gouvernement. Je vais mettre aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables qui est pour son adoption qui est contre, il n'est pas adopté après l'article 76 un amendement 128 c'est monsieur Gontard, qui va nous présenter. madame la présidente, cet amendement qui a été présenté à l'Assemblée nationale par de nombreux groupes politiques, notamment la malheureusement sans, sans succès, celui-ci est pourtant simple, il demande au gouvernement la mise en Oeuvres d'un nouveau et massif plan d'investissement pour le climat, afin que notre pays respecte ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, la stratégie nationale bas carbone et les Budgets carbone nationaux, en effet, alors que l'urgence climatique est à son paroxysme, nous pensons qu'il convient que le gouvernement pose des actes enfin en faveur de la transition écologique en arrêtant par exemple de subventionner les énergies fossiles, mais c'est aussi de mesures positives dont nous avons besoin, l'objectif est, dans ce cas d'vient de connaître toutes les mesures d'investissements publics et privés à mettre en place pour combler les entre l'investissement actuel et l'investissement jugé nécessaire de faire converger les Front national dans un but de transition écologique, disons, il manque 15 milliards d'euros par an pour que la France agisse concrètement compte le réchauffement du climat, ce chiffre, c'est celui de l'annexe du budget, un document qui s'appelle stratégie bas carbone et lutter con quartier filialisation des sols, développer des transports propres, promouvoir l'agriculture durable, il faut que l'avance que la France investissent 15 milliards d'euros par an dans les secteurs public et privé et même 30 milliards à partir de 2024,

Merci madame la présidente, madame le ministre, monsieur le rapporteur, pour faire face à la crise écologique, la France s'est notamment fixé comme objectif, celui de réduire de 40 pourcent nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et ceci dans le cas de la loi de transition énergétique pour une croissance verte et solide, atteint de la neutralité carbone à l'horizon 2050 dans la loi énergie-climat or force est de souligner que sans un effort considérable, la France ne parviendra pas respecter ses engagements pourtant décliné dans une feuille de route qui s'appuie sur la stratégie nationale bas carbone et la programmation pluriannuelle de l'énergie pour répondre à l'urgence climatique il avant tout nécessaire de réorienter les investissements vers le développement durable, ça suppose donc de contrôler les flux financiers de réorienter la finance vers le financement de l'économie réelle et au service de la transition écologique, il s'agit là, donc d'un enjeu de taille aujourd'hui la finance est toujours principalement orientée vers le financement des énergies fossiles, selon l'Institut de l'économie pour le climat, les investissements fossiles défavorable au climat représentent plus de 70 milliards d'euros en France et se concentrent principalement dans le secteur des transports, il faut donc agir pour que les investissements marron diminue au profit des investissements verts tant privé que public, cet enjeu est d'autant plus de taille que les chantiers de la transition énergétique nécessite des investissements massifs tant public peut privé, force est donc de souligner que dans un contexte de faible croissance et de faiblesse des investissements privés un nouveau grand plan d'investissement public pourrait jouer un rôle moteur, il pourrait donc permette d'enclencher une dynamique vertueuse, en relançant les investissements privés : ceci est d'autant plus envisageable que les taux d'intérêt au long cours sont aujourd'hui extrêmement faible, voire négatif ainsi donc les taux souverains français à 10 ans sont dans ce contexte particulièrement favorable, ce contexte de faiblesse des taux d'intérêt public accroît donc les les marges de manoeuvre et des États, en améliorant les conditions de soutenabilité des dettes publiques et donc on pourrait donc aller vers, respect des limites fixées par rapport au PIB pour le déficit public, PIB pour le déficit public, il serait pour le moins illogique de ne pas saisir cette opportunité pour élaborer, au service de la transition écologique de grand plan d'investissement dans tous les secteurs de de l'économie, ceci afin de faire basculer notre mode de production et de consommation vers un mode plus sobres et moins émetteurs de gaz à effet de serre donc cet amendement propose en conséquence que le Gouvernement remette au Parlement un rapport portant sur l'élaboration d'une stratégie nationale d'investissement pour accélérer la transition écologique et solidaire, l'objectif est de recenser les investissements publics et privés à programmer, il faut conclure, l'écart entre l'investissement actuel et l'investissement jugé nécessaire pour atteinte des objectifs fixés par les Budgets carbone prévue dans la stratégie nationale je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements. Alors l'avis de la commission, il y a une demande de Pékin de plan d'investissement climat qui vient s'ajouter à à toutes les démarches notamment conduite par le gouvernement avait pas seulement depuis l'épisode il y a celui des gilets jaunes, donc il y a eu d'abord le Haut conseil pour le climat, le conseil de défense écologique, il y a aussi 150 de nos concitoyens, a tirées au sort réparties sur toute la France qui doivent rendre un avis des conclusions pour la fin de l'année et le Haut conseil pour le climat qui doit, après avoir obtenu la réponse du gouvernement avant la fin de l'année, venir présenter des conclusions un rapport devant les assemblées parlementaires notamment, donc, Madame la Ministre, moi ce que je pense c'est que vous sentez qu'il y a un appétit et une envie de faire, j'ai l'occasion de le dire, je pense que le gouvernement, à mon avis a eu tort de vouloir sortir le débat des enceintes où il doivent avoir lieu, c'est-à-dire dans les assemblées parlementaires dans les assemblées dans les territoires et puis, avec des démarches diverses et multiple ne contournait par les élus, associer les les élus, vous font une proposition : moi je prends ça comme un amendement d'appel alors je ne sais pas dans quelle salle vous allez réunir tout le monde parce que entre les assemblées, le Conseil économique et social, et puis toutes celles et tous ceux qui veulent participer mais je vous invite en tous les cas à intégrer ces démarches qui sont des démarches qui démontre que nous avons besoin, c'est le plus important de nous approprier les enjeux parce que les enjeux écologiques et environnementaux, il concerne tous les secteurs, série concerne évidemment les particuliers mais concerne aussi les entreprises, ils concernent le monde agricole, il concerne la question des déplacements et des mobilités, si on veut trouver une trajectoire à la fois accepter demain après qu'elle eut été voté ou après qu'elle aura été voté ce que j'attire votre attention sur les 2 épisodes, pour moi, qui ont vu la la France trébucher, d'abord l'écotaxe puisque les bonnets rouges et puis la ministre qui vous a précédé avait souhaité arrêter complètement le dispositif et puis là, l'accélération de la trajectoire carbone en plus vous la connaissez bien puisque, à l'époque, je crois que vous étiez très proche d'elle, mais il faut vraiment faire attention sur les enjeux qui sont ceux de l'approche. Je vous invite à conclure le sur le rapport. Oui, mais j'entends madame le maire présente, mais je crois qu'il faut être très attentif a perdu beaucoup de temps et on a, je pense qu'on aura pas le droit à une 3ème erreur. Je vous rappelle, mes chers collègues, veut nous avançons très lentement. Madame la Ministre, quel est l'avis du gouvernement. Merci madame la présidente, alors moi je partage tout à fait l'idée qu'il est indispensable de mobiliser à la fois des investissements publics et privés pour atteindre nos objectifs climatiques, je voudrais rappeler que la programmation pluriannuelle de l'énergie définies, les mesures concrètes nécessaires dans les différents secteurs pour atteindre nos objectifs à l'horizon 2028 notamment en terme de subvention publique et d'incitation aux investissements privés alors effectivement il y a d'autres démarches qui sont en cours, moi je voudrais citer par exemple la démarche pacte productif pour le plein emploi en 2025 dans lequel nous menons un travail très approfondi avec l'ensemble des filières économiques avec un objectif d'atteindre une une économie neutre en 2050, dans une France qui devra, au demeurant à être neutre et puis par ailleurs, comme vous l'avez rappelé monsieur le rapporteur, on a effectivement une Convention citoyenne dans lesquelles 150 Français travaillent pour faire des propositions sur les mesures qui les concerne, qui concerne tous les Français et qui peuvent nous permettre d'atteindre nos objectifs en termes de réduction de d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, je voudrais enfin souligner qu'on a également une démarche de budget Vert qui permettra de faire continuellement progressé la contribution du budget de l'État à nos objectifs environnementaux et, enfin, de nombreux travaux sont 2 sont menées pour donner suite au rapport qu'enfin Zaouati pour mobiliser davantage des financements privés, donc je crois qu'on ne manque pas de rapport et qu'effectivement maintenant il faut passer aux actes et je voilà, je ne pense pas qu'il soit utile de prévoir à nouveau un rapport telle que vous le proposez donc avis défavorable. S'il n'y a pas de demande d'explication de vote, je vais mettre aux voix l'amendement 128 avec 2 avis défavorables qui est pour son adoption. Qui est contre. N'est pas adopté le 190 avec 2 avis défavorables qui est pour. Qui est contre, il n'est pas adopté. Toujours après l'article 76 un amendement 194 c'est monsieur monsieur Gillet qui va nous présenter. Merci madame la présidente, madame la Ministre, monsieur le rapporteur, nos investissements sont-ils suffisants non, c'est pourquoi il faut assurer le financement de la programmation des investissements prévus par la loi d'orientation des mobilités, sur la période 2019, 2037 les auteurs de l'amendement propose que l'État lève un emprunt à moyen et long terme et demande au gouvernement de remettre un rapport au Parlement à ce sujet pour attester de cette opportunité en effet afin de répondre aux besoins d'entretiens, de renouvellements de modernisation et de nouvelles capacités en matière d'infrastructures de transports et de mobilité, la loi d'orientation des mobilités comporte une programmation financière des investissements réalisés sur le moyen et long terme, qui, selon l'exposé des motifs, s'appuie sur des ressources pérennes, le comité d'orientation des infrastructures avait présenté, dans son rapport de janvier 2018 3 scénarii en amont des débats sur le projet de loi d'orientation des mobilités, le gouvernement avait annoncé privilégier le scénario numéro 2, or il faut aller beaucoup plus loin pour déployer les transports de demain : favoriser le déploiement des nouvelles mobilités revivifier le rail et développer le fret ferroviaire, les donc de la responsabilité du politique de se donner les moyens d'entretenir comme de développer des infrastructures de transport pour permettent d'assurer à nos enfants et petits-enfants un Patrimoine à la hauteur des enjeux qui exige aujourd'hui la transition écologique à laquelle le secteur des transports et des mobilités peut fondamentalement contribué, il faut donc faire aujourd'hui, dans ce contexte de faiblesse des taux d'intérêt de révolution numérique et d'urgence écologique à Paris sur les structures nouvelles et programmer les investissements nécessaires pour éviter de transmettre aux générations futures une dette écologique insurmontable car celle-là, nous ne pourrons jamais la rembourser. Quel est l'avis de la commission madame le rapporteur. Alors, la Commission va vous dire, chat échaudé craint l'eau froide, donc étant donné ce qu'on a vu pour le rapport sur la Société du Grand Paris, qui devait permettre de justifier les taxes supplémentaires à voter pour assurer le financement, et notamment explicité les leviers financiers permis et qu'on n'a absolument rien eu dans un rapport qui nous a été délivrée, bien après la date limite, et je pense qu'on a eu le rapport parce qu'on n'a plus qu'insister pour l'obtenir, si on veut vraiment séjour du sujet ben le Parlement est tout à fait capable de rédiger un telle rapporte donc avis défavorable. Madame la Ministre, quel est l'avis du gouvernement. Merci madame la présidente, alors on peut refaire le débat de la loi mobilité mais je pense que pour la première fois, on a une trajectoire à 10 ans. Avec 13,4 milliards d'euros sur ce quinquennat 14 3 sur le prochain 13 4 c'est 40 pourcent de plus que dans le précédent quinquennat et par ailleurs, les mesures fiscales qui ont été proposées permettent d'assurer la correspondance entre les dépenses et les ressources, donc je pense que votre amendement est pleinement satisfait. Je vais mettre aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables qui est pour son adoption. Qui est contre, il n'est pas adopté. Toujours après l'article 76, l'amendement 171 rectifié monsieur Lafond va nous présenter. il s'agit de 2 des subventions sur les énergies fossiles, l'accord de Paris en signé en 2015 à engager les pays qui l'ont signé, à sortir des subventions ou à l'énergie aux énergies fossiles, l'abandon vise tout simplement à mettre en place un calendrier pour cette mesure et d'ici 2025, que la France s'engage à sortir de ce système de subventions publiques pour les énergies fossiles. vous aviez dit 3 donc défavorable. en général, du fait de la concurrence internationale, donc il y a déjà une réduction de ces niches qui est prévu dans le cadre du projet de loi de finances que vous examinez au-delà, je pense que ce sont des mesures qui ne peuvent pas se prendre de façon isolée c'est tout le sens de la démarche que nous avons porté au niveau de l'Union européenne d'avoir un prix du carbone un prix plancher du carbone et d'avoir une démarche harmoniser au niveau européen, comme vous pourrez d'imaginer si on devait supprimer les avantages fiscaux pour le transport routier alors qu'on a déjà un différentiel de de taxation du gasoil professionnel avec nos voisins, on voit que tout seul, ça ne donnerait pas les effets escomptés, donc moi je vous propose le retrait sinon avis défavorable. défavorable. Je veux mettre aux voix l'amendement 171 rectifié bis avec 2 avis défavorables qui est pour son adoption. Qui est contre. Il est adopté. Le 171 rectifié est adopté, toujours après l'article 76 ans, amendement 195 c'est Monsieur Jacques non mais Merci madame la présidente, d'une trajectoire qui vise à la suppression progressive de ces subventions à l'horizon 2025 et enfin des mesures d'accompagnement des secteurs concernés, alors vous allez me dire, encore un, un rapport de plus mais, néanmoins, faute d'action immédiate, il est bon de donner une orientation politique, en effet, le montant des remboursements et des exonérations sur la TICPE qui concerne la consommation des énergies fossiles, en 2019 va s'élever à 11 milliards d'euros à ces exonérations et taux réduit, il faut ajouter les subventions en faveur des énergies fossiles, sous forme de garanties à l'export qui sont donc délivré par Bpifrance assurance Export pour le compte de de l'État, la France en 2019 qui était pays hôte du du G7 s'était engagé en 2016 à supprimer les subventions aux énergies fossiles d'ici à à 2025, elle s'est dotée d'un objectif de réduction de la consommation d'énergies fossiles, également de 30 pourcent en 2030, qui a été porté à 40 pourcent donc il faut maintenant que cet engagement soit suivie d'actions en France pour éviter que ces objectifs ne restent des voeux pieux, ne restent des voeux pieux, tout comme il faut trouver des solutions avec les secteurs concernés, pour permettre que cette suppression progressive des des subventions n'ait pas eu un impact sur l'emploi et sur le développement des entreprises. Si monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission. Sur le 195. Oui, c'est ça défavorable. Quel est l'avis du gouvernement, Madame la Ministre, je vais mettre aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables qui est pour son adoption. Qui est contre. Il n'est pas adopté toujours après l'article 76 un amendement 196 monsieur Merci madame la présidente, un un un Ministre le présent amendement vise à évaluer les conséquences économiques et financières d'un élargissement de l'assiette de la TICPE à l'ensemble des carburants fossiles dans le contexte de transition écologique et énergétique absolument nécessaire, les autres, l'auteur de l'amendement estime qu'Intel rapport permettrait au gouvernement et au Parlement de disposer de l'ensemble des informations nécessaires pour prendre à bras-le-corps cette question à travers l'outil qu'il estime être le plus important en matière de fiscalité nationale. nationale. Ce rapporteur, quel est l'avis de la commission défavorable, quel est l'avis du gouvernement. Je veux mettre aux voix l'amendement 196 avec 2 avis défavorables qui est pour son adoption. Qui est contre, il n'est pas adopté. Toujours après l'article 76 le 188.

ce rapport étudie notamment l'opportunité d'une révision de la prime à la conversion de bonus écologique dans l'optique de mieux cibler les véhicules et logique régime instauré des règles d'éligibilité ouvrir ce dispositif à l'achat de véhicules d'occasion, moins polluant, ouvrir la prime à la conversion de véhicules verts électrique instaurer un prêt à taux 0, ouvrir la prime à la conversion à d'autres solutions de transport pour encourager le rapport moral les dispositifs d'aide doivent également pouvoir soutenir l'ensemble des ménages, et en particulier des plus modestes et les plus dépendants du transport individuel afin que l'ensemble de la flotte automobile évolue plus rapidement vers un modèle de mobilité compatible avec les exigences climatiques. il y a 2 aspects : il y a à la fois les les demandes que vous faites les propositions. Pour améliorer les critères d'éligibilité, l'ouverture le le sujet des véhicules propres et puis il y a une demande de rapport sur les aides à l'acquisition des véhicules propres, moi ce que je vais vous faire comme propositions c'est comme je l'ai fait tout à l'heure aux sénateurs, Laffont, au pire, on regarde, on travaille un petit peu ensemble, on se met d'accord,

je pense qu'il vaut mieux avoir un tableau qu'on remplit chaque année qui donne une trajectoire que de multiplier les rapports, honnêtement, on ne fait qu'alourdir le travail parlementaire, je n'en vois pas l'intérêt, je pense qu'on a plutôt intérêt à tenir une évaluation permanente, ce qui nous permet de mieux suivre les éléments donc avis défavorable. C'est l'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Merci madame la présidente, même vie je souligne qu'il y a une récente étude du Commissariat général au développement durable, qui a été publié il y a peu de temps, et par ailleurs il y a une mission spécifique qui a été confiée à l'inspection des finances sur l'accès pour les ménages à faibles revenus à des véhicules propres, donc un rapport supplémentaire supplémentaire ne me paraît pas nécessaire. Je vais mettre aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables qui est pour son adoption qui est contre. Il n'est pas adopté toujours après l'article 76 3 amendements qui font l'objet d'une discussion commune le 129 c'est monsieur Gontard, qui va nous présenter. Merci madame la présidente, cet amendement est à la fois la la reprise d'un amendement, présenté à l'Assemblée nationale par le rapporteur mais enrichie en fonction de ce que j'avais moi-même proposé de l'examen de la proposition de loi de notre groupe sur la renaissance renationalisation des autoroutes, il s'agit ainsi de remettent la main sur une manne non négligeable lui ni Pef a ainsi estimé les ressources possibles à 2 milliards d'euros en 2032 2004 2 4 milliards en 2000 33 6,4 milliards en 2035 et 11 5 milliards en 2037 cette proposition reprend ainsi l'idée émise dans le rapport de l'examen de la proposition de loi visant à la renégociation des sociétés concessionnaires d'autoroutes, en effet, à défaut de s'orienter vers la nationalisation, que nous appelons de nos voeux, il convient, a minima, de prévoir l'avenir et d'anticiper la fin des concessions et le retour dans le giron public des sociétés concessionnaires et cela par la création d'un état d'établissement industriel et commercial, nous considérons en effet que seule la confirmation de l'Epic permet un statut réellement public contrairement à une société anonyme dont les évolutions de capital sont beaucoup, beaucoup quoi qu'il en soit, une telle réflexion doit s'engager dès à présent, elle pourrait se traduire par la création d'un établissement public industriel et commercial dénommé routes de France, compétent pour gérer l'ensemble des 9200 kilomètres de réseau routier avec un contrat d'objectifs et de performance des critères fort en matière d'aménagement du territoire, d'efficacité environnementale et de différenciation des tarifs selon des motifs sociaux ou environnementaux, ce qui permettrait par exemple de taxer bien plus lourdement les camions et autres poids lourds, le Patrimoine routier pourrait ainsi être utilisé comme un vrai Champ d'action publique pour l'intérêt général plutôt que de le laisser le de laisser le privé agir à sa guise, L'amendement 174 rectifié monsieur Cabanel, qui va nous représenter. Oui merci madame la présidente, madame la ministre et chers collègues, c'était amendement de notre collègue Nathalie Delattre, il vise à anticiper la fin des différentes concessions autoroutières entre 2031 et 2036, il demande la remise d'un rapport sur l'opportunité de créer une société anonyme à capitaux publics, assure la gestion des autoroutes à la fin de ces concessions, et sur les mesures législatives adoptées pour permettre la poursuite de la perception des péages pour le compte de l'État, ainsi que la possibilité d'affecter ces nouvelles ressources ces Et pour un amendement identique le 212 Monsieur Jacquin. Il est défendu. Il est identique,

on n'a pas une boule de cristal, donc je pense qu'on irait vraiment beaucoup trop loin, sachant qu'en même temps quand je vous ai entendu vous connaissez déjà le nom du futur établissement qui serait créée, donc c'est fantastique parce que généralement le nom de l'établissement est souvent ce qui vient, ce qui vient en dernier, et ensuite il me semble que, aujourd'hui, le réseau autoroutier n'est pas le réseau le plus mal entretenus donc peut-être, concentrons-nous sur les vrais sujets, la régénération dans le ferroviaire, la régénération dans le fluvial et puis laissons le temps aux autoroutes de vivre. Madame la minuscule est l'avis du Gouvernement sur ces amendements. Merci madame la présidente, alors moi je note l'influence croissante de l'Uni pense que enfin je je ne pense pas qu'il soit urgent de produire un rapport sur la fin des concessions qui se situe entre 2031 et 2036 donc avis défavorable. Oui, déjà pour réponde sur le nom n'a pas dit qu'on connaissait déjà le nom, c'était une proposition qu'on avait fait dans la proposition de loi sur la renationalisation des des concessions de d'autoroute par compte sur Madame me souviens justement quand on avait débattu de ce texte, vous ne disiez pas tout à fait ça, vous disiez que il fallait clairement s'occuper de la fin de ces concessions, vous disiez même que la la privatisation des autoroutes avait été une une erreur, il me semble que que c'est ce que vous avez ce que vous aviez dit, donc là on on est plus dans cette logique-là, et du coup de de prévoir justement l'avenir, alors peut-être qu'on s'y prend tôt mais en tout cas je pense qu'il vaut mieux s'y prendre tôt prévoir les choses avec la fin d'arriver des des concessions. me Monsieur Jacquin. Très rapidement, une question comme celle-là doit s'anticiper un maximum, faut-il rappeler à nos chers collègues et très rapidement que cette idée a été proposée pendant la loi des mobilités, à l'Assemblée nationale par un député qui s'appelle Jean-Baptiste Djebbari et la question est revenue pendant la discussion budgétaire à l'Assemblée où, paraît-il, il s'est engagé à réfléchir à la suite, cette question doit s'anticiper véritablement à l'avance et donc s'y prendre à l'avance, ce n'est pas chercher à perdre du temps, j'en ai assez perdu. s'il n'y a pas d'autres demandes d'explication de vote j'mettre aux voix l'amendement 129 avec 2 avis défavorables qui est pour son adoption. Qui est contre. Il n'est pas adopté les 2 amendements identiques 174 112 avec 2 avis défavorables qui est, pour leur adoption. Qui est contre. Ils ne sont pas adoptés toujours après l'article 76 un amendement 143 madame Préville va au présent, merci. Si Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, cet amendement vise à donner de la visibilité aux opérateurs de la biodiversité en matière d'évolution de leurs effectifs dans les années à venir, comme nous l'avons déjà dit, la réduction des effectifs enregistrée cette année par le ministère de l'écologie n'est pas acceptable 5 pourcent des postes disparaîtront en 2020 et ce chiffre atteindra 10 pourcent en 2022, des milliers de postes sont impactés, or dans le même temps l'urgence climatique se précise et la nécessité de décliner nos politiques publiques de préservation de l'environnement et de presse, prévention des risques sur les territoires aide urgente de plus le gouvernement mène des réformes et je pense notamment à celles de l'économie circulaire qui nécessiteront un suivi et une mise en oeuvre et sur le terrain, nous estimons donc indispensable d'enrayer cette diminution croissant des effectifs et de sanctuariser les moyens financiers et humains, les opérateurs de la biodiversité qui oeuvrent dans la lutte contre le changement climatique et la transition écologique nous proposons donc ainsi qu'un rapport du gouvernement dresse un bilan précis des évolutions d'effectifs des principaux opérateurs agissant dans le Champ de la biodiversité, puis recommande une trajectoire d'effectifs à 5 ans leur permettant d'une part, de mener à bien leur mission, et d'autre part, de leur donner de la visibilité, je vous remercie. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Il est défavorable. Quel est l'avis du gouvernement, Madame la ministre. Je vais mettre aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables qui est pour son adoption. Qui est contre, il n'est pas adopté toujours après l'article 76 un amendement 189. Madame Préville. Merci madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, réaliser des travaux de rénovation énergétique peut se révéler extrêmement compliqué pour les particuliers qui ne disposent souvent pas d'expertise technique solide sur le sujet, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage et déterminant dans la réalisation des travaux pour établir un programme de travaux mobiliser les différents financements poste disponible et c'est un garde-fou précieux vis-à-vis de toute forme d'escroquerie, la nouvelle prime résultant de la transformation du grain, du crédit d'impôt, transition énergétique CTE devrait permettre de renforcer l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, le présent amendement demande un rapport au gouvernement sur le sujet afin de renforcer dans le PLF 2021 les aides finançant l'assistance à la maîtrise d'ouvrage,

Je vais mettre aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables qui est pour son adoption. Qui est contre, il n'est pas adopté toujours

en élaborant une feuille de route de présenter en juillet 2019, le gouvernement a réaffirmé son engagement à mettre en oeuvre les objectifs de développement durable, tant sur le plan national qu'international, en s'emparant de en s'emparant de l'agenda 2030 la France a souhaité ainsi assurer la cohérence de ses engagements internationaux et des politiques en faveur du développement durable notamment renforçant la synergie dans la mise en oeuvre de l'agenda 2030 et l'accord de Paris mais sans un volet budgétaire budgétaire claire les politiques de développement durable sont difficilement évaluables en ce sens, cet amendement propose que le rapport annexe présente l'impact des mesures proposées dans le cadre du projet de loi de finances et du projet de bois de financement de la Sécurité sociale de l'année par rapport aux objectifs de développement durable fixés par l'agenda 2030, ce rapport pourrait être élaboré en concertation avec des organismes indépendants et s'appuyer sur le travail déjà réalisé par l'INSEE, il permettra ainsi de mesurer les efforts du gouvernement dans l'attente des 17 au aider ainsi que les avancées spécifiques réalisées chaque année, merci. Merci, quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. ce sur quoi il travaille, c'est-à-dire le livret de la transition énergétique j'alors je reconnais que le livret aujourd'hui hé bien maigre, qu'il s'approprie une partie de ce qui a été fait avant même qu'il souhaite au pouvoir mais c'est pas, c'est je fais confiance à un travail collectif, en tous les cas à cet instant, je pense qu'on aura notre mot à dire et notre part prendre lorsque les choses ont avancé dans les propositions du gouvernement, donc je pense que c'est un amendement d'appel. Madame la mise, quel est l'avis du gouvernement. Merci madame la présidente, alors je voudrais rappeler que les mesures budgétaires en lien avec l'environnement font déjà l'objet d'un rapport spécifique intitulée Financement de la transition écologique les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l'environnement et du climat annexé au projet de loi de finances 2020 l'Inspection générale des finances et le CGEDD ont rendu un rapport en septembre 2019 visant à mettre en place un budget Vert rapporte qui comporte déjà une première évaluation du budget 2000 19 et ce rapport servira de socle à la présentation du budget vers de 2021 par rapport, par ailleurs, pardon, le rapport économique, social et financier annexé chaque année au projet de loi de finances détails quant à lui les aspects sociaux du PLF, donc je pense que c'est c'est votre amendement est globalement satisfait. monsieur Montaugé pour explication de vote. dans nos processus parlementaire, nous ne le ferons nous nous faisons référence à ses objectifs de développement durable, qui, pour autant, constituent des engagements qu'a pris la France dans le concert international elle est en pointe sur sur ces sujets qui touchent à tout développement durable, donc moi je pense, pour aller dans le sens de l'amendement qu'il faudrait que dans l'esprit de la LOLF on on mettre

de faire le lien entre l'évolution de 2 de ses objectifs et les actions que nous votons dans le cadre des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la Sécurité sociale, il y a un lien Direct qui doit pouvoir être être fait et qui qui irait dans le sens je pense du purin de transparence, de, de, de notre action au service de nos concitoyens et et de notre pays. Je vais mettre aux voix l'amendement 193 avec 2 avis défavorables qui est pour son adoption. Qui est contre, il n'est pas adopté. à l'article 76 bis, un amendement 127 et c'est Madame Assassi qui va nous représenter. Oui merci madame la présidente, je vais aller très vite, puisque c'est un sujet dont on a souvent parlé ici dans cet hémicycle, c'est à propos du Charles-de-Gaulle Express donc avec cet amendement, nous souhaitons au delà d'un report de la taxe de financement du Charles-de-Gaulle Express qui est donc prévu dans cet article, son abandon pur et simple, afin notamment de tenir compte de la priorité donnée aux transports du quotidien dans les objectifs définis par la loi d'orientation sur les mobilités madame la Mini j'aimerais attirer votre attention sur l'état catastrophique de la circulation du RER B notamment sur sa partie nord est et Sud aussi monsieur Giulia mais plus souvent sur le nord-est de la multiplication des jours où Les Hall de gare et les guichets sont fermés, laissant à l'abandon des centaines d'usagers notamment la veille ou ces derniers doivent renouveler leur passe Navigo, je dois vous dire sincèrement que cette situation devant devient vraiment insupportable. Merci madame la présidente, voilà le ministre, chers collègues, d'abord je voudrais dire la présente à ceci que temps même usager des mêmes ligne à une gare près par rapport à à la vôtre, je partage votre appel à ce que l'état des gares et des services fournis aux voyageurs en gare s'améliore, bien évidemment, cela dit, je ne suis pas certain que l'amendement puisse y contribuent, puisque l'abandon du projet Charles-de-Gaulle Express peut paraître démesurée par rapport à la question des services en gare et au-delà, je vous donne tout à fait crédit de votre constance sur ce sujet, bien évidemment, parce que vous l'avez rappelé vous-même, il y a eu beaucoup d'occasions illicite débattre du CDG Express, je pense que le gouvernement a pris une position les assemblées ont pris une position ce projet maintenant avance alors la ministre avait souhaité s'assurer, à la demande de nombreux élus locaux et de nombreux parlementaires d'ailleurs que l'évolution des travaux du CDG Express ne viennent pas trop contraindre ou ne pas plus contraindre encore le fonctionnement du RER B et notamment l'avancée il y a des des programmes de rénovation du ARB qui prennent c'est vrai du temps et c'est à ce titre-là que le gouvernement a décidé de décaler le CDG Express pour que justement la priorité soit faite aux travaux du Uber et moindre contrainte si je puis dire sur sur le B, donc moi j'ai tendance à vous répondre d'abord avec un avis défavorable, on vous dit, indiquant que l'article 76 Vista qu'il est rédigé prend acte tout ce que la ministre a annoncé c'est-à-dire décalage CDG Express et permet de faire que la taxe qui permettra notamment de le financer soit décalé et je pense qu'il faut laisser cet article en l'état et donc l'avis est défavorable sur votre amendement. Madame la Ministre, quel est l'avis du gouvernement. qui porte à la fois sur la nouvelle signalisation les travaux à réaliser sur l'infrastructure pour accueillir les nouvelles rames du du RER B, la mise en accessibilité des gares et compte tenu de cet important programme de travaux, vous savez que nous avons fait le choix, comme vient de le rappeler, Monsieur le Sénateur, Capo Canellas de décaler la mise en service de CDG Express, dont je rappelle qu'il n'est financé par aucune subvention publique et qu'ils contribuent à un programme de 500 millions d'euros qui améliorera lui aussi le fonctionnement du RER B, donc avis défavorable. Merci, je vais mettre aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables qui est pour son adoption. Qui est contre et n'est pas adopté Je vais mettre aux voix l'article 76 bis qui est pour son adoption. Qui est contre. Il est adopté à l'article 76 terre un amendement numéro 11 au nom de la commission des finances monsieur Capo Canellas. Merci madame la présidente, alors nous avons eu, là aussi, est très long moment de débat à l'occasion de de la loi pacte et Jean-François Husson en tant que rapporteur à l'époque, s'en souvient et il y a puissamment contribué et le ministre de l'Économie et des Finances lors de ces débats, s'est engagé à ce qu'il ait une avance qui soit faite au bénéfice des riverains de l'aéroport de Paris Charles-de-Gaulle afin d'accélérer les travaux d'insonorisation de leur logement, c'est un sujet majeur bien évidemment et l'article 76, terre de ce projet de loi de finances vient matérialiser cet engagement et donc le process, c'est que Aeroports de Paris fait une avance et que se rembourser a posteriori par le produit et la taxe sur les nuisances sonores aériennes simplement Aéroport de Paris étant une société anonyme avec un actionnaire majoritaire qui est l'État, il est plus sûr de prévoir que l'avance se rembourser avec des intérêts, les intérêts qui sont faibles, parce que c'est l'intérêt faibles aujourd'hui mais simplement sinon un actionnaire minoritaire pourrait reprocher pourrait reprocher à l'État, actionnaire majoritaire d'avoir ainsi bénéficier d'un d'un Avantage et je précise que sur d'autres, le procès s'il y a d'autres sujets sur lesquels, aéroports de Paris fait une avance à l'état et qu'il y a toujours un petit mécanisme d'intérêt dont les discussions de le sinon actionnaire minoritaire pourrait chercher noise sur ce plan, merci. Madame la miss qu'est l'avis du gouvernement. Merci madame la présidente, alors je voudrais souligner que, effectivement, cet article 76 terrain constitue une avancée très importante, hein, pour les riverains d'aéroports puisqu'il va permettre d'accélérer les travaux d'insonorisation, avec une avance de 77 millions d'euros par aéroports de Paris, on sait qu'on a un stock conséquent de dossiers qui est en attente, et donc ils vont pouvoir être dans ce cadre, l'article L qu'il a été voté, exclut la prise en compte des intérêts qui ne paraît pas un enjeu très important au moins à court terme compte tenu des taux très bas, toutefois, compte tenu de la durée, sur plusieurs années de l'avance que pourrait consentir à ADP, je pense qu'effectivement, l'amendement pourrait contribuer à la mise en oeuvre. Enfin, à motiver, aéroports de Paris, on va dire pour réaliser cette avance, donc je m'en remets à la sagesse de votre haute assemblée. Je vais mettre aux voix cet amendement de Miro 11 de la commission des finances, avec un avis de sagesse du gouvernement qui est pour son adoption. Qui est contre, il est adopté. Et je vais mettre aux voix l'amende l'article 76 terre qui est pour son adoption qui est contre, il est adopté, je mais aux voix, l'article 76 quater, qui est pour son adoption. Qui est contre, il est adopté. Je mais également on voit l'art, l'article 76 qu'inquiet, ce qui est pour son adoption. Qui est contre. Il est adopté. Un article additionnel après après l'article 76 qu'inquiet, ça l'amendement numéro 66 monsieur Jean Sol qui va nous représenter. Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les rapporteurs madame le rapporteur, mes chers collègues. ça concerne un article additionnel après l'article donc 76 qui inquiète les moyens prévus dans le PLF 2020 aux 176 réserves naturelles nationales existantes s'élève à 22 86 millions d'euros en autorisations d'engagement y a 22 91 millions d'euros en crédits de paiement ces réserves naturelles nationales le représente un acteur incontournable de la mise en oeuvre de la stratégie nationale pour la biodiversité, les fédérations des réserves naturelles de nos territoires, indique que les moyens attribués aux réserves pour assurer leur mission de connaissances, de gestion et de surveillance, l'ont pas été réévalué depuis 2012, ce qui les met en difficulté pour répondre aux objectifs assignés et préserver s'est dite réserves, véritable poumon pour notre pays aussi cette dernière avance que pour réaliser pleinement étant de bonnes conditions leur mission et les sécuriser les besoins sont estimés à 25 millions d'euros, l'article 55 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, reconnaît tôt réserve naturelle nationale le rôle d'animation de mise en réseau et de coordination technique des réserves naturelles en métropole et Outre-Mer et de représentation, même si j'ai cru comprendre que la commission n'était pas favorable au rapport cet amendement propose de réaliser un rapport faisant le bilan de la situation des réserves naturelles nationales bilan non réalisé, faut-il le rappeler, depuis 2012, soit depuis 7 ans. Merci, quel est l'avis de de la commission, monsieur le rapporteur. soutenus ou suggérés par la fédération des réserves naturelles, je pense que le sujet n'est pas négliger, on l'a évoqué à plusieurs reprises sur tous les sujets touchant à la biodiversité au moyen et vous l'avez dit, je crois que c'est important, la question de l'animation pour qu'on ait une bonne appropriation, je ne suis pas sûr qu'il faille établir un rapport notamment un rapport annuel, par contre, je souhaite que le gouvernement puisse proposer pour 2020, un état des lieux de la situation depuis 2012 pour faire droit à votre demande, pour bien évaluer et tracer les perspectives, là encore on pourrait convenir que dans les rapports dès l'année prochaine, on est des premiers éléments retenir là encore quelques éléments objectifs partagés avec la Fédération des réserves naturelles qui pourraient être joints chaque année par un tableau de bord dont on pourrait convenir des modalités et des critères retenus. Madame la mise, quel est l'avis du gouvernement. le périmètre de ces aires protégées et puis également sur les modalités de gestion de ces aires protégées, en particulier dans l'atteinte de l'objectif qui a été fixé par le président de la République de transport en aires protégées, dont 10 pourcent sous protection forte il y a des débats sur ce que signifie protection forte et donc nous avons lancé fin nuançant je préside un comité de pilotage demain pour lancer la révision de notre enfin la l'élaboration de notre nouvelle stratégie nationale sur les aires protégées, donc dans ce cadre-là, on aura notamment l'occasion de faire le bilan de la gestion nous réserve naturelle et et je pense que tous ces éléments doivent aboutir à une. Proposition de nouvelle stratégie nationale sur les aires protégées au début de l'année 2020 avec l'objectif de pouvoir adopter cette stratégie pour le congrès de Luyssen qui se tient au mois de juin, à Marseille donc tous les éléments seront sur la table au 1er trimestre de l'année 2020, donc je propose le retrait de votre amendement qui me semble pleinement satisfait.

à présent, nous allons procéder à l'examen de l'amendement portant sur les crédits du budget annexe Contrôle et exploitation aériens figurant à l'État, grand, à l'article 39 un amendement numéro un de la commission des finances présenté par monsieur le rapporteur Capo Canellas. du prolongement d'une discussion que nous avons eu longuement dans cet hémicycle, lundi, vous savez que nous avons adoptée à l'initiative du rapporteur général un amendement auquel j'avais le plaisir de de contribuer, qui visait à l'effet sur la compétitivité de l'éco-contribution sur le transport aérien du transport aérien qui est proposée par le gouvernement, nous avions plusieurs options supprimer l'éco-contribution, essayer de dons fléchés le produit mais vous savez que la loge ne nous le permet pas moduler et ce n'était pas aussi une chose facile, et nous avons pas pris ces options-là, nous avons préféré laisser les contres contribution telle quelle, mais choisir d'en atténuer fortement l'impact et donc de baisser la taxe d'aviation civile de 72 1000000 72 millions pourquoi parce qu'elle progresse d'ailleurs d'un peu plus de 29 millions d'euros cette année, vu l'augmentation du trafic et ensuite ben nous tirons les conclusions parce que il était prévu dans le projet de loi de finances, qui est présenté par le gouvernement est sorti de l'Assemblée, une baisse de l'endettement du budget annexe, vous savez que c'est ce budget annexe a connu une dette qui avait cru fortement après la crise de 2008, cette dette a été très fortement diminué d'à peu près 40 pourcent elle a été ramenée à peu près à 600 millions je cite ce chiffre de mémoire et donc voilà on propose cette année de ne pas franchir un cap supplémentaire de désendettement de reporter et donc de d'abaisser le désendettement de 172 millions et vous savez que lundi, ben nous avons utilisé ces 72 millions pour abaisser la taille avait ça veut dire que les compagnies seront en partie compensés penser 72 millions de baisse de la taxe d'aviation civile, alors qu'il y a 230 millions proposés par le gouvernement de taxe supplémentaire, ça vient compenser voilà. Quel est l'avis du gouvernement, Madame la Ministre. la diminution de 72 millions d'euros des crédits du bassin du BSCA signifierait une baisse des remboursements d'emprunt de 72 millions d'euros, or les remboursements d'emprunts qui sont prévus dans le PLF correspondent exactement aux échéanciers contracté avec l'Agence France Trésor donc ses rangs pour remboursement font partie d'équilibre global de la gestion de la dette et le non-remboursement de 72 millions d'euros, renchérit renchérirait immanquablement le coût de la dette en conséquence : avis défavorable. Je vais mettre aux voix cet amendement de la commission avec un avis défavorable du gouvernement qui est pour son adoption. Il est adopté. Il est adopté. Nous allons procéder au vote des crédits du budget annexe Contrôle et exploitation aériens figureront à l'État, c'est : je n'ai été saisi d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite je mais on voit les crédits du budget annexe qui qui est pour. Leur adoption qui est contre et sont adopté. Nous allons procéder au vote des crédits du compte spéciale Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale figurant à l'état D, je n'ai été saisi d'aucune demande d'explication de vote avait avant l'expiration du délai limite jamais on voit les crédits du compte spécial qui est, pour leur adoption. Qui est contre, ils sont adoptés, nous allons procéder au vote des crédits du compte spécial services nationaux de transport conventionnés de voyageurs figurant à l'état D, je n'ai été saisi d'aucune demande d'explication de vote avant avant l'expiration du délai limite je mais on voit les crédits du compte spécial qui est, pour leur adoption. Qui est contre, ils sont adoptés, nous allons procéder au vote des crédits du compte spécial Transition énergétique figurant à l'état D, je n'ai été saisi d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite je mais on voit les crédits du compte spécial qui est, pour leur adoption qui est contre, ils sont adopter. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille est parvenu à l'adoption d'un texte commun.

Mes chers collègues, l'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finance adoptée par l'Assemblée nationale pour 2020 nous poursuivons l'examen au sein de la seconde partie du projet de loi de finances différentes missions : le Sénat va examiner les crédits de la mission enseignement scolaire et articles 76 70 76 obtiennent la parole est à monsieur Gérard Longuet, rapporteur spécial de la commission des finances pour 7 minutes. Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, il m'a dit une malédiction s'abat sur le budget de l'enseignement scolaire qui, chaque année, passent un peu plus tard pour des interventions un peu plus courtes sur des sommes plus plus importantes et avec des difficultés croissantes, nous avons donc à relever un défi, celui de la sobriété dans le propos, ce qui n'est pas mon tempérament naturel donc je vais essayer d'être extrêmement bref et peut-être même parfois télégraphique. Monsieur le Ministre, la commission des finances à la demande de son rapporteur, c'est-à-dire votre serviteur propose au Sénat d'adopter votre budget en l'amendant, d'une façon extrêmement modeste et qui ne porte pas sur les sommes pourquoi le faisons-nous, motif de la commission des finances et et Germain mais nos collègues partagent ce soutien, nous le faisons parce qu'il pour des idées simples, la 1ère c'est que vous êtes dans la continuité de l'année précédente et surtout dans la continuité d'une demande constante du Sénat soutenir le primaire qui est constitutif de la réussite scolaire qui a parfois dans notre pays les chiffrent qu'on de comparaisons internationales établissent clairement été sacrifiés, c'est la première raison, la seconde raison, c'est que vous maîtrisez les effectifs.

puisque, en effet, le primaire voit ses effectifs augmenter d'une façon significative et évidemment au détriment des effectifs du secondaire qui était. Doté très convenablement, c'est la 2ème raison de notre soutien, la 3ème et que vous avez pris l'initiative d'un bac à lauréats réformée rénovée et manifestement ce défi audacieux semble porter ses fruits, ainsi qu'en témoigne la restructuration des options choisies par nos élèves de terminale, une quinzaine de tripler pourcent des élèves et correspond bien à une plasticité qui leur permettra d'aborder l'étape de Parcoursup et donc de l'intégration dans l'enseignement supérieur dans des conditions plus favorables. 4ème point et je crois que c'est un sentiment, une volonté partagée par l'ensemble des collègues vous soutenez l'effort engagé depuis Nicolas Sarkozy d'ailleurs d'une façon significative en faveur de l'inclusion des élèves handicapés, et vous avez en particulier consolider le statut matériel des A. et c'est un effort méritoire qui permet dans une active dans un secteur qui pose des questions de d'une autre nature, et en particulier le fait que si l'Éducation nationale, prend en charge ce n'est pas elle qui décide, situation inconfortable ou possible le 5ème point que que j'évoquerai parce que j'y tiens comme ancien président de région et d'ailleurs, président de l'Association des régions de France, vous avez décidé de transférer aux régions, l'orientation professionnelle et c'est un effort important, c'est en tous les cas un changement tant il est vrai que l'enseignement s'organise autour de ses débouchés, à condition, naturellement, de les connaître, s'organise pas seulement à raison des débouchés, mais il s'organise aussi à raison des débouchés tout va-t-il pour le mieux dans le meilleur des mondes, la réponse est naturellement non parce que nous, nous avons des interrogations très légitimes qui ne nous interdisent pas de soutenir votre action, mais qui nous font vous de poser des questions auxquelles vous aurez, j'en suis certain le coeur et le bonne volonté de répondre la première concerne l'effort en faveur de l'enseignement primaire, vous avez fait cet effort de dédoublement en cours préparatoire et on ancée premières années vous suivez vos élèves à travers des évaluations qui sont suivis. Et la question qui nous vient naturellement à l'esprit : avez-vous déjà des indications significatives sur l'effet du dédoublement des classes dans les secteurs d'éducation prioritaire pouvez-vous décelé devrait mouvement dans l'aptitude des élèves du primaire qui bénéficient de C. dédoublement, c'est une question extrêmement importante pour nous et pour la commission des finances, parce que le dédoublement n'est pas gratuit, ce qui est une évidence, et s'il est, s'il est productif de réussite, nous la campagne rendions plus volontiers encore, c'est une ouverture, il faut en avoir la confirmation. Le 2ème, sujet sur lequel vous interroge. C'est en fait le statut des enseignants-j'ai évoqué tout à l'heure, la maîtrise des effectifs mais dans le budget, on s'aperçoit que le mouvement le plus significatif, ce sont les mesures catégorielles, que vous n'avez pas décidé, dont vous avez hérité, je parle du célèbre PPCR, parcours professionnels carrières rémunération dont l'impact sur la progression budgétaire et de près de 400 millions cette année, c'est-à-dire le triple de ce qu'il était pour l'année 2019, payer mieux, pourquoi pas, à condition de pays et mieux ceux qui sont les plus exposés et ce dont on a le plus besoin et le PPCR est exactement le contraire, c'est une mesure sympathique, généreuse, chaleureuse, payés par le contribuable de Pro personne de proportionnalité absolue aboutit à soutenir les enseignants en fin de carrière, j'ai de la sympathie pour eux parce qu'ils ont la proximité de mon âge, mais nous avons surtout besoin de jeunes enseignants qui s'engage et nous avons besoin dans certaines filières de pouvoir attirer des enseignants qui sont tentés par d'autres et à juste titre d'autres débouchés professionnels, donc nous avons une maîtrise des effectifs des enseignants, c'est qu'une bonne chose, mais nous n'avons pas de d'une vision très claire de la politique salariale que vous souhaiteriez sur moyen terme, j'ajoute que dans cette politique, il y a aussi la politique des effectifs qui doit tenir compte de la démographie française nous avons hélas, et nous le savons, car rien n'est plus prévisible que la démocratie Des chiffres qui vont évoluer et qui vont évoluer d'une façon.

les décisions de la conférence des présidents, mais je trouve très honnêtement que ce n'est pas une bonne façon de traiter l'enseignement et l'éducation dans notre pays que de l'année au rapporteur, un temps dont il n'abuse pas et donc je confirme que le problème de des effectifs de la des enseignants est un problème majeur et je terminerai enfin parce ce que je vais quand même vous faire plaisir je trop de sympathie pour vous terminera enfin par les conséquences de transfert aux régions D de l'orientation, l'éducation nationale choisira suivra-t-elle les conséquences de décisions qu'elle ne maîtrisera plus

Non, je trouve très franchement. Tous, tous les rapporteurs sont dans la même situation, oui, mais tous les juges n'ont pas la même importance madame tous les buts. La parole est à monsieur Jacques Grosperrin, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication pour l'enseignement scolaire. Madame la présidente, monsieur le Ministre, madame la présidente de la commission monsieur les rapporteurs injuste quelque peu l'année dernière avec vous, monsieur le ministre, je serai plus équilibrée 6 jours 3 minutes qui me permettront uniquement de vous poser quelques questions. Le président de la République a lancé priorité fort de nos pliait au primaire avec le plafonnement de la taille des classes à 24 élèves en grande section, CP, CE1, sur l'ensemble du territoire d'ici la rentrée 2022 ainsi que le dédoublement des classes de grande section de maternelle en REP et REP plus votre engagement en tant que ministre Éducation nationale a été également déterminant, or l'effort à faire est important 26000 classes seront concernées par le plafonnement des effectifs à 24 élèves Cottreau dédoublement des classes de grande section 10000 postes ont été nécessaires pour ce dédoublement des classes de CP, CE1, certes la démographie des élèves à la baisse, mais nous ne sommes que plusieurs milliers de postes seront nécessaires pour mener à bien ces annonces, or c'est le 440 emplois dans l'enseignement primaire ont été créés dans le budget 2020, peut-être pourriez-vous, Monsieur le Ministre, revenir sur le schéma précis d'emplois pour la rentrée 2020, 2021 et 2000 22 et nous rassurer ainsi par ailleurs de nombreuses communes s'interrogent sur les conséquences financières des récentes annonces relatives à l'éducation, l'abaissement de l'instruction obligatoire et coût du vrai forfait les conséquences foncière du d'éboulements des classes en REP et REP plus dans des zones souvent densément peuplé et où il n'est pas facile au construire avec un plafonnement des effectifs à 24 élèves ou encore le plan pauvreté selon les informations qui nous ont été transmises la rentrée actuelle est-il dans certains endroits tendue pour les dédoublements de ces cas se révélerait plus en raison de problèmes de bâtiments, certaines communes ont utilisé des locaux destinés à d'autres usages comme l'accueil périscolaire, d'autres ont avancé des sommes importantes pour rénover ou construire de nouveaux locaux scolaires dans l'attente d'un remboursement par l'État, ce sont autant de sommes actuellement gelés au détriment d'autres investissements de la collectivité pour la ville de Grenoble par exemple le montant serait de 600000 euros, monsieur le Ministre, nous avons été contactés par plusieurs maires qui s'interroge sur les modalités pratiques de remboursement des dépenses qu'elle doit faire du fait de vous un de ces annonces et de vos annonces vous connaissiez les contraintes budgétaires qui pèsent sur les collectivités locales, je souhaite que des directives détaillées soient soient rapidement transmises aux préfectures pour pouvoir éclairer les élus locaux sur la marche à suivre, néanmoins, malgré ses inquiétudes, nous constatons que le budget dédié à l'enseignement scolaire est en hausse, plus 1,37 milliards d'euros enracinement agricole il traduit l'engagement du gouvernement en faveur de l'acquisition des savoirs fondamentaux primaire ainsi que la prime, il aurait été accordé à l'école exclusive je reconnais en cela votre engagement ainsi ce sont 220 millions d'euros supplémentaires, soit un bond de 14 pourcent qui sont consacrés à scolarisation des élèves en situation de handicap, nous ne pouvons que nous en féliciter, c'est la raison pour laquelle la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication, a donné un avis favorable sur l'adoption des crédits de la mission enseignement scolaire je vous remercie. la. Parole est à monsieur Antoine Karam, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication pour l'enseignement technique agricole. Madame la Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous avons eu l'occasion, il y a moins d'un mois de débats sur l'avenir de l'enseignement agricole débat riche et constructif à cette occasion, nous avons pu constater l'attachement de tous nos groupes politiques à cet enseignement, véritable pépite pour la formation de nos jeunes, pour reprendre les mots du Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture dans ce budget un milliard 4 d'euros sont consacrés à l'enseignement agricole, c'est une augmentation de 7,15 millions d'euros, celle-ci a dû au protocole PPCR et là, à la poursuite de la campagne de communication et de promotion de langue segments agricoles, l'aventure du vivant des métiers, grandeur nature, la rentrée 2019 a constitué, du moins je l'espère un tournant pour l'enseignement agricole après une érosion continue des effectifs, et encore une baisse de 4000 élèves l'an dernier, on constate pour la première fois depuis 10 ans, une augmentation des effectifs à la rentrée 2019 de plus de 750 élèves, cette hausse est la conséquence des efforts importants d'information et de valorisation de l'enseignement agricole, il a toutefois nécessaire de poursuive l'effort de communication au niveau local, en effet, l'enseignement agricole présente la spécificité d'être un enseignement national ancrage territorial, la déclinaison de cette campagne de communication sur les territoires et donc essentiel, en outre, il me semble nécessaire de prendre en compte cette inversion de la tendance sur les ETP dans les prochains arbitrages budgétaires et si elle venait à se pérenniser l'enseignement agricole perd en effet 60 ETP en 2020 et selon le schéma d'emploi pluriannuel il devrait peur 80 ATP en 2021, nous sommes donc dans une situation où le nombre d'élèves augmente et le nombre de personnels diminue, je souhaite pour terminer ce propos évoquer la crainte d'un décrochage entre l'enseignement scolaire et l'enseignement agricole pour les personnels d'assistance éducative, il semblerait que le budget de l'enseignement agricole n'est pas pris en compte la revalorisation de l'indice des assistants d'éducation, de septembre dernier, les personnels d'assistance éducative jouent un rôle essentiel, nous le savons, particulièrement dans les lycées agricoles en effet près de 60 pourcent des élèves sont internes de plus l'enseignement agricole accueille un homme important d'élèves à besoins particuliers sur le ministre, nous connaissons la priorité de votre gouvernement en faveur de l'école inclusive aussi j'espère qu'une solution sera rapidement trouvée sur ce sujet, j'en suis convaincu l'enseignement agricole est une filière d'avenir en prise avec les défis émergents ce budget en hausse et le rapprochement tant attendu entre les 2 ministères, témoigne de l'intérêt que porte le gouvernement à cet enseignement, c'est pourquoi la Commission de la culture, de l'éducation, de la communication, a donné un avis favorable à l'adoption des crédits du programme 143 consacré à l'enseignement agricole de la mission enseignement scolaire je vous remercie. Merci. Dans la suite de notre discussion, je vous rappelle que le temps de parole attribués à chaque groupe pour chaque discussion qu'on prend le temps d'intervention général et celui de l'explication de vote par ailleurs le gouvernement dispose au total de 20 minutes pour intervenir. La parole est à monsieur Jacques Bernard Magner pour 5 minutes.

Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, ce projet de budget est en hausse de 1,9 pourcent par rapport au précédent mais restent malheureusement bien inférieur aux objectifs fixés par la loi de programmation des finances publiques, adoptée en 2017, c'est donc une augmentation en trompe-l oeil car le milliard d'euros supplémentaires permettra seulement de financer des augmentations de charges mécanique sans même il suffirait d'ailleurs en ce qui concerne les emplois on déshabille Pierre pour habiller Paul, puisqu'on observe que si 440 emplois sont créés dans le 1er degré 440 postes sont supprimés dans le second degré, on sait que, suite à l'abaissement de l'âge de la scolarité obligatoire à 3 ans, la rentrée 2020 verra l'arrivée de 28000 élèves supplémentaires dans le 1er degré de plus, monsieur le Ministre, vous annoncez que toutes les classes de grande section de maternelle en repérer plus seront dédoublées, à la rentrée 2020, après celle de CP et de CE1 et que les effectifs de toutes les autres classes de ces 3 niveaux seront progressivement limité à 24 élèves, c'est très bien mais pour satisfaire tous ses objectifs au demeurant parfaitement louable, les 440 créations d'emplois que vous prévoyez dans le 1er degré seront très insuffisante, selon nos calculs, il faudrait procéder à la création de 10000 postes sur 3 ans, soit 3300 emplois par an dans le 1er degré pour un coût d'environ 200 millions d'euros, je rappelle qu'il y avait eu 1850 suppressions de postes en 2019 dont 1050 pour le 1er degré public au total il y aura eu plus de 6200 suppressions de postes dans le second degré pour les trois exercice 2018, 2000 19 et 2020, alors que les effectifs dans le même temps, enregistré une hausse de 99 mise de 99000 élèves on est donc très loin du compte et tous ces chiffres ne sont pas du tout satisfaisant mais Monsieur le Ministre, vous balayez souvent d'un revers de main la problématique des postes pour privilégier les heures supplémentaires et, là, justement, comme en 2019 aucun fléchage n'apparaît quant aux crédits destinés au financement des heures supplémentaires demandées aux enseignants pour compenser les suppressions de postes, sans compter que ces heures supplémentaires sont subi et n'ont pas choisi par les professeurs, le fameux travailler plus pour gagner plus que vous prenez s'accorde mal avec le métier d'enseignant et ses contraintes. S'ajoute à cela la non prise en compte de la revalorisation salariale des enseignants, la non-résolution des difficultés que connaissent les directeurs d'école et vous le savez bien, ce n'est pas la mobilisation des jeunes gens, service civique qui va y remédier, toutes ces questions non réglées, ainsi que l'insuffisance du nombre des ASH et des moyens de remplacement restent des points sensibles dans la bonne prise en charge de nos élèves, enfin votre volonté affichée de vouloir faire former les enseignants sur leur temps de vacances me paraît extrêmement grave, quel salarié accepterait cela. Je rappelle d'ailleurs à tous ceux qui considéreraient que les vacances des enseignants sont trop nombreuses, trop longue, si l'on compte leurs heures de correction de recherche de préparation des cours, les enseignants dépasse et ceux qui l'ont été, ou le savent, dépasse largement les 35 heures par semaine. Les fonds sociaux dédiés aux collégiens et lycéens en difficulté 10 minutes exceptionnellement de moitié alors qu'ils permettent d'aider tous ces jeunes issus de milieux défavorisés, ils sont d'une grande utilité et on sait que beaucoup n'y accède pas alors qu'ils le pourraient. C'est pourquoi le groupe socialiste, vous propose un amendement visant à rétablir les crédits destinés à ces fonds sociaux à hauteur de leur montant de 2019. Monsieur le ministre vous affichez des volonté légitime, mais vous ne prévoyez pas les moyens qui doivent y être cela cela engendre beaucoup de frustration et d'inégalités. Vous dites que vous essayez de rendre la profession d'enseignant attractive c'est bien. Mais les actes de pas même si nous soutenons certaines actions comme le pré-recrutement des enseignants qui ressemble étrangement d'ailleurs aux emplois d'avenir professeur lancée par un de vos produits prédécesseur, Vincent Peillon, qui les avait créé en 2013, monsieur le ministre, le projet de budget que vous nous présentez s'il apparaît volontariste dans les intentions affichées et tout à fait insuffisant si l'on se réfère à l'avenir et aux enjeux de notre système éducatif en 2020 dans ces conditions, malheureusement nous ne pourrons donc pas l'approuver, Merci, la parole est à Madame Françoise Laborde. Pour 6 minutes chers collègues. Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous évoquons les crédits alloués à la mission enseignement scolaire qui sont en progression de 1,37 milliard d'euros cette année si l'évolution de l'investissement de la France dans l'éducation augmente encore en 2020, elle est à remettre en perspective les comparaisons internationales nous enseigne que le budget public total de l'éducation représente en moyenne 10,8 pourcent des dépenses publiques totales des pays de l'OCDE, alors qu'en France, cette part n'est que de 8,4 pourcent cette hausse de crédit à vocation notamment rééquilibrer les financements vers l'élémentaire en accompagnant la très importante : poursuite du dédoublement des classes de CP et de CE1 dans le réseau d'éducation prioritaire, ainsi que son extension aux classes de grande section, alors que la France dépense l'équivalent de 7600 dollars pour un élève en élémentaire, contre 8500 pour la moyenne des pays comparables, l'effort qui est fait en faveur de ces classes depuis 2018 paraît fondée, toutefois nous aimerions disposer d'un bilan scientifique précis de cet effort en matière de résultats scolaires peut-être pourrions-nous saisir le Cnesco cette progression des dépenses vise également des mesures de revalorisation catégorielle d'une profession qui, nous le savons, manque d'attractivité sur le long terme en raison du salaire des enseignants qui reste en 2019 inférieur de 7 pourcent la moyenne de l'OCDE en début de carrière avec un écart qui se creuse à 22 pourcent en milieu de carrière 58 millions d'euros sont ainsi utilement consacré en 2020 au renforcement des rémunérations des enseignants, on respirait plus que nous avions appelé de nos voeux dans notre rapport conjoint avec Max Brisson, la progression couvre également l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap, ce qui comprend une amélioration des conditions de d'emploi des AESH dont nous avons beaucoup discuté cette année puisque, depuis la rentrée 2019 tous les accompagnants sont recrutés en contrats de droit public de 3 ans renouvelable une fois, avant une possible transformation en contrat à durée indéterminée, les mesures de la conférence nationale du handicap et l'CDI sation 10 AESH explique ainsi une variation de 28,6 millions d'euros du programme vide l'élève en augmentation de 5 pourcent là où les autres programmes de la mission plafonne à 1 ou 2 si nous approuvons globe globalement ces progression des crédits et les politiques qui le soutiennent, cela ne peut masquer certaines interrogations pour l'avenir de notre enseignement par exemple la suppression de 440 emplois d'enseignants dans le secondaire public n'est pas acceptable, il faut garder l'Avantage de l'investissement fait sur plusieurs décennies dans l'enseignement secondaire et ne pas le détricoter pour alimenter le 1er degré le groupe RDSE propose donc plusieurs amendements visant à annuler ces suppressions de postes par ailleurs des solutions urgentes doivent être apportées pour faire face au nombre croissant de postes d'enseignants non pourvus lors des concours 1400 je crois cette année, la question de la formation continue est aussi un enjeu majeur dont nous avions débattu lors de l'examen de la loi sur l'école de la confiance, or ces crédits sont en baisse de 3,45 pourcent, soit près de 30 millions d'euros pour les enseignants du 1er degré, ce qui est contradictoire avec l'objectif affiché sur le plan de l'accompagnement social des élèves, nous regrettons la baisse drastique de 29 millions d'euros, soit la moitié des financements affectés aux fonds sociaux versés aux établissements qui permettent d'apporter une aide exceptionnelle aux familles défavorisées afin, alors que la pauvreté ne cesse de progresser dans notre pays, si cette baisse par un habile le langage budgétaire n'aura pas d'impact sur les fonds versés par les établissements en raison de la sous-consommation de ces crédits d'année en année nous ne pensons pas que la solution est de les supprimer, mais plutôt d'encourager les établissements à mieux identifier et accompagner leurs élèves en difficulté, comment cette baisse, monsieur le ministre est-elle compatible avec la stratégie du gouvernement de lutte contre la pauvreté et notamment la division par 2 du taux de pauvreté des enfants d'ici 2022, je propose donc un amendement visant à annuler cette baisse des crédits affectés aux fonds sociaux des établissements, cela fait plusieurs années que le Sénat, alerte sur l'état inquiétant de la santé scolaire en France déjà, dans son rapport pour avis sur le PLF 2017, le rapporteur noté une baisse des effectifs de médecins de l'Ordre de 20 pourcent en 10 ans, qui ne permet pas de couvrir le territoire, les derniers chiffres nous montrent que le nombre de médecins et infirmiers a encore baissé en 2019 le rôle de la médecine scolaire est pourtant essentiel en matière de dépistage précoce et de médecine préventive afin d'affirmer notre priorité, nous proposons 2 amendements permettant de renforcer l'attractivité de la profession de médecin scolaire dont la rémunération est aujourd'hui la plus faible de la fonction publique je conclurai mon propos en évoquant l'enseignement technique agricole, nous nous interrogeons concernant la cohérence du coût du schéma d'emploi pluriannuel pour la période 2019, 2022, cette année encore, il prévoit une réduction de 60 ETP, alors que 2020 est une année charnière qui voit au contraire le nombre d'élèves de cette filière, progressé de 750 nouveaux entrants grâce à l'action positive de la communication du ministère de l'Agriculture, nous devrions donc redoubler d'efforts dans la valorisation de ces cursus qui font aussi la richesse de nos territoires, en conclusion, malgré une hausse des crédits pour les 3 principaux programmes de la mission, ce budget soulève encore trop de questions dans un contexte budgétaire que nous savons, contraint et qui applique le principe des vases communicants, en conséquence, le groupe RDSE s'abstiendra sur les crédits de la mission, je vous remercie. Pour 6 minutes chers collègues. Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, vous présentez ce budget sous l'angle d'une augmentation des moyens de l'Éducation nationale, malheureusement nous ne partageons pas votre enthousiasme, puisqu'on assiste en effet à une hausse de 1,9 pourcent de ce budget, mais c'est à dire une hausse inférieure à l'inflation et ça a été dit, qui sert essentiellement à la ligne budgétaire glissement glissement vieillesse technicité qui augmente mécaniquement et à la ligne, parcours professionnels carrières et rémunérations qui permet une augmentation de salaire des professeurs décidés par le précédent gouvernement, avant d'être gelé par le vôtre, puis finalement mise en oeuvre, surtout ce budget semble bien loin des engagements du gouvernement comme du président de la République, on voit mal en effet comment la création de 440 postes seulement dans le 1er degré permettra de soutenir les dédoublements en REP et REP plus ou le développement de de classes à 24 élèves en grande section, CP et CE1 d'ici la fin du quinquennat pas plus que la concrétisation des annonces faites dans le plan de rattrapage des services publics en Seine-Saint-Denis absentes de votre budget, on aurait d'ailleurs pu espérer que le soutien aux collectivités locales pour adapter les lieux d'enseignement au dédoublement concerne aussi les autres départements puisque bien des communes rencontrent des difficultés en ce sens, on est donc loin de la priorité affichée pour le 1er degré dans le secondaire, les coupes sont clairs, avec une diminution de bien plus de 440 postes redéployés vers le primaire, alors que l'on attend entre 30 et 40000 nouveaux élèves, vous n'avez à l'évidence pas pris la mesure du malaise qui traverse l'éducation nationale, dans le cas par exemple des directeurs d'école, des solutions concrètes pour les soulager d'une charge de travail trop lourdes, manque cruellement, je regrette d'ailleurs que notre amendement proposant un plan de recrutement d'assistants d'éducation à même de prendre en charge une partie du travail administratif qui incombe au directeur était déclarée irrecevable, mais je ne désespère pas de vous convaincre et de cette idée que nous continuerons bien évidemment à défendre, il y a donc les sujets pour lesquels les financements nécessaires manquent, il y a aussi ceux pour lesquels les bulles, les Budgets sont carrément réduits, il en va ainsi des fonds sociaux dont les Budgets sont quasiment divisé par 2 au prétexte que les familles ne les sollicite pas assez, c'est là un raisonnement qui n'est pas entendable pour les élus de terrain que nous sommes qui savons à quel point la précarité des familles combien le pouvoir d'achat est une préoccupation quotidienne et combien les efforts de notre système scolaire pour y répondent sont insuffisants, l'école française est l'une de celles qui perpétue le plus les inégalités et alors que la précarité des élèves et des étudiants s'impose comme un problème central, cette décision est pour le moins choquante, autre question centrale concernant la précarité, celle des accompagnants d'enfants en situation de handicap, sans contrat, sans salaire, ou avec des acomptes qu'on leur demande ensuite de rembourser, j'ai déjà j'ai déjà pu évoquer ce sujet avec vous, monsieur le ministre, en commission, mais ces problèmes, je vous le confirme, reste malheureusement d'actualité, avec des contrats non signés ou bâclée, sans parler de notification toujours non pourvus à plus de 3 mois de la rentrée, et si pour ces femmes, parce que ce souci, ce sont souvent de jeunes femmes, la situation reste catastrophique en Seine-Maritime, il me semble que les choses ne sont guère mieux dans un certain nombre d'autres départements, votre budget sur ce point nous renseigne bien sur votre vision, l'augmentation de 17 pourcent du budget de recrutement des AESH par le or titre 2, c'est-à-dire par les établissements pour des postes mutualiser et de droit privé et sans équivoque, vous vous éloignez de l'objectif de faire des AESH, un corps de fonctionnaires en déresponsabilisant l'état de leur recrutement et vous confirmez bien nos craintes d'une inversion des priorités entre les besoins des enfants en situation de handicap leur besoin d'accompagnement prescrit parler MDPH et les moyens que l'institution dans une approche purement comptable envisage de mobiliser la colère gronde chez ceux et celles qui sont méprisés et ainsi que dans les familles d'enfants en situation de handicap, la colère secoue aussi l'enseignement agricole frappée de plein fouet par votre réforme du lycée qui doit faire face à d'autres mesures comme les modifications des seuils de dédoublement pour la réalisation, par exemple, de travaux pratiques entre autres problèmes spécifiques à cette filière, je ne peux pas clore mon propos sans évoquer la situation des collectivités territoriales, situation d'abord marquée par une grande désertification scolaire qui continue malheureusement d'avancer au grand désarroi de nos concitoyens des territoires ruraux et de leurs élus, malgré les promesses présidentielles cette rentrée a été celle de 112 nouvelles fermetures d'écoles et de 240 Fusion sur cette question des fermetures, je me permets de vous rappeler, Monsieur le Ministre que lors de l'examen du projet de loi pour une école de la confiance, vous m'aviez assuré que les élèves relevant d'Ulysse serait désormais comptabilisés dans les effectifs et ce n'est malheureusement toujours pas le cas, c'est non seulement un manque d'humanité assez insupportable pour les familles concernées mais cela conduit aussi dans bien des cas, à des fermetures de classes qui pourrait, qui devrait même être maintenus, même chose pour les enfants qui ont 3 ans durant l'année scolaire et qui entrent à l'école, en cours d'année et qui ne sont pas toujours comptabilisées non plus pour toutes ces raisons, vous le comprendrez, nous ne voterons pas ce budget qui est pour nous une preuve supplémentaire de la déconnexion de ce gouvernement, des besoins de notre système scolaire et de la souffrance de ceux qui le font vivre au quotidien, je vous remercie. Merci, la parole est à Madame Colette Mélot. Pour 6 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, messieurs les rapporteurs avec 74 milliards d'euros en crédits de paiement, soit 1 milliard 200 supplémentaires par rapport à 2019 le budget de la mission enseignement scolaire pour l'année 2000 va représente le 1er poste de dépenses de la nation et témoigne de la volonté du gouvernement de poursuivre les efforts engagés en direction de l'égalité des chances et de l'acquisition de savoirs fondamentaux. Le gouvernement fait le choix de renforcer les moyens du 1er degré, cela se concrétise dans le programme 140 consacré à l'enseignement scolaire public du 1er degré avec le dédoublement des classes de CP, CE1 en REP iraient plus étendu aux grandes sections de maternelle de ces mêmes zones le plafond, le plafonnement progressif des effectifs à 24 élèves par classe en grande section, CP, CE1, ainsi que l'entrée en vigueur depuis la rentrée de l'abaissement de l'âge obligatoire de scolarité à 3 ans les réformes destinées à renforcer la scolarisation en milieu ordinaire des élèves présentant un handicap se poursuivent avec pour objectif de faire de l'école républicaine, une école véritablement inclusive dans les 3 années à venir, des avancées importantes sont à saluer comme le recrutement de plus de 4000 AESH cette année, rattaché au programme 230 la transformation des contrats des AESH en CDD de 3 ans, ainsi que le déploiement de 3000 pôles inclusifs d'accompagnement localisé, il faut poursuivre sur cette voie pour valoriser le métier d'accompagnant d'élèves en situation de handicap et améliorer le taux d'encadrement particulier des enfants qui n'ont besoin l'école et plus largement l'enseignement scolaire doit être le lieu qui gomme les différences et accompagne chaque enfant sur la voie de l'émancipation et de la réussite ce programme contient également les premières mesures destinées à simplifier le travail des directeurs d'école avec une journée supplémentaire de décharge leur permettant de ne pas être dans une classe, ainsi qu'un allégement de charges administratives, le programme 141 de la mission porte sur l'enseignement scolaire public du second degré il finance notamment la nouvelle obligation de formation pour les 16 18 ans, nous regrettons la suppression de 440 postes au sein de ce programme redirigés vers l'enseignement du 1er degré si la lutte contre les décrochages scolaires commence dès l'école maternelle, le collège et le lycée sont les moments les plus sensibles pour les jeunes les plus exposés et les plus fragiles. L'allongement des durées d'enseignement à travers la généralisation des heures supplémentaires pour les enseignants ne pourra remplacer pleinement les postes supprimés, d'autre part, la revalorisation du métier d'enseignant, tant en terme d'image que de salaire reste une priorité. Le programme 230 consacré à la vie de l'élève bénéficie de la plus importante hausse avec 5 11 pourcent de crédits supplémentaires, bénéficiant en grande partie au financement de l'école inclusive, il consacre également les crédits réservés à la lutte contre le harcèlement scolaire dont plus de 11. Ce sont des élèves sont victimes ces crédits serviront au financement de plateforme de signalement de situations de harcèlement, et en particulier de cyber harcèlement la vie de nombreux enfants peut basculer à cause d'insultes et de moqueries ou de photos postées sur les réseaux sociaux et leur scolarité peuvent devenir un calvaire. Au sein du programme 143 nous devons poursuivre nos efforts pour valoriser l'enseignement agricole, notamment auprès de jeunes élèves urbain, ils sont plus de 108000 élèves à s'engager dans cette voie, mais ses effectifs baissent d'année en année monsieur le Ministre, j'aimerais attirer votre attention sur une problématique souvent occulté dans le débat public 60 pourcent des jeunes vivent en dehors des grandes métropoles comme le dit la présidente de l'association Chemin d'avenir Salomé Berlioz une un jeune qui a grandi dans le Puy-de-Dôme où les Vosges pour ne citer que 2 exemples à moins accès à l'information, moins de figures modèle auquel s'identifier pour choisir un métier moins confiance en lui, moins de mobilité, cette accumulation d'obstacles fait qu'une grande partie de la jeunesse issue de la France périphérique reste prisonnière d'un plafond de verre et n'a pas la liberté je choisir son avenir. Pour paraphraser les mots de Nelson Mandela, je dirais que l'éducation est une est une arme d'Intelligence massive nous rêvons d'une école qui soit le lieu de tous les savoirs, un temple de la culture partagée de la tolérance, une école du courage, de la saine curiosité où l'on apprend aussi le respect de la République et de ses valeurs, voilà ce que nous souhaitons pour tous nos enfants et ce que nous souhaitons pour chaque citoyen, le groupe les indépendants républiques et territoires votera le budget de cette mission en vous demandant de poursuivre vos efforts pour faire monsieur le Ministre véritablement de l'école un levier de réussite pour tous les élèves. Je vous remercie, merci, la parole est à Madame Dominique V. rien.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis 2 ans, vous avez mis en place Monsieur le Ministre, hein, plusieurs mesures devant assurer une meilleure prise en charge, ainsi qu'une meilleure réussite des élèves, le dédoublement des classes ont repéré plus la réforme du Baccalauréat ou encore la scolarité, la scolarisation obligatoire dès l'âge de 3 ans et nous vous avons soutenu dans ses démarches, qui nous semble positive pour l'avenir de nos enfants, par ailleurs, la revalorisation des salaires dans le cadre de la mise en oeuvre du parcours professionnels carrières et rémunérations : le PPCR nous paraît utile utile et indispensable, en effet, le salaire des enseignants est en moyenne inférieur aux autres fonctionnaires de l'État, de plus, les salaires des enseignants sont 13 disparates entre le primaire et le secondaire, de même la revalorisation de l'enseignement aurait plus et l'augmentation du nombre d'heures supplémentaires défiscalisées sont les bienvenus pour autant ce fameux PPCR est encore axé sur nous une hausse de salaire en fin de carrière, ce qui peut poser question quant au futur, calcul des retraites s'il devait se faire par points, il en est de même d'ailleurs d'une augmentation au travers des heures supplémentaires, un travail de revalorisation tout au long de la carrière des enseignants est donc nécessaire pour rendre à ce métier, sa valeur et son attractivité il nous paraîtrait également intéressant de trouver un juste équilibre et de se rapprocher de la moyenne salariale européenne je voudrais également Monsieur le Ministre, vous faire part d'une inquiétude des territoires ruraux, qui s'est exprimé déjà lors des annonces de des bouts doublement des CP, CE1, avec quels moyens humains, notre collègue Jacques Grosperrin rapporteur estime entre 7 et 8000 le nombre d'enseignants supplémentaires nécessaires à ces dédoublements et au plafonnement à 24 élèves pour les classes des grande section, CP, CE1, sur l'ensemble du territoire, or et cela a déjà été dit plusieurs fois, seulement 440 nouveaux postes sont créés pour l'année à venir, sachant que les calculs du nombre de professeurs par élève sont faits sur la base de moyenne départementale, ce qui ne veut rien dire dans des secteurs aussi vaste et hétérogène que les départements ruraux, vous comprendrez que l'on craignent qu'il ne faille déshabiller Pierre pour habiller Paul, et si j'ai bien compris qu'aucune école ne serait fermé, je crains que ne nombre de nombreuses classes le soit encore malgré tout. Pourtant, comme vous le constatez vous-même, on enseigne mieux dans une classe qui n'est pas surchargé, un élève apprend mieux s'il n'a pas 2 heures de transport par jour et nos classes à plusieurs niveaux sont très souvent gage de réussite, merci donc de ne pas les sacrifiés et puisque je suis arrivé à la campagne, je poursuis en évoquant les petits-déjeuners que les écoles rurales sont également invitées à mettre en place, mais étant donné les transports scolaires étant donné qu'on ne va pas demander aux enfants de se lever 30 minutes plus tôt ce petit-déjeuner doit alors être servi sur le temps scolaire, or les enseignants n'ont pas de consignes claires sur ce sujet, ce petit déjeuner doit-il être pris sur leur temps, doit-il être servi par eux en maternelle, il y a les Atsem mais en primaire, cela mérite donc d'être éclaircies et pour en finir sur la ruralité, j'aurais aimé apporter mon soutien à l'amendement de mon collègue Laurent Lafon, qui demandait un observatoire de la scolarité en milieu rural car il semblerait qu'aucune donnée sur ce sujet n'ait été collectées depuis 1995 je comprends que la création d'un observatoire puisse être coûteuses, ce qui a justifié le rejet de cet amendement mais observé de la part de l'Éducation nationale présente sur tout le territoire et faire remonter des données devrait être considéré comme un devoir, et non comme un coût supplémentaire, voilà monsieur le ministre, quelques inquiétudes bien légitimes mais qui n'empêcheront pas le groupe Union centriste de voter le budget de la mission enseignement scolaire. Merci, la parole est à monsieur Max Brisson. Pour 5 minutes chers collègues.

Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le ministre, vous nous avez récemment encouragé à penser le professeur du XXIe siècle. La mission enseignement scolaire consacrant 92 pourcent de ses crédits aux dépenses de personnel pour près de 1 1000000 de personnes, voilà l'occasion en 5 minutes d'aborder concrètement ce sujet par c'est le professeur du XXIe siècle, c'est d'abord dessiné un métier qui demain serait redevenu attractif, attractif parce que mieux payés attractif car bénéficiaire du de GRH de proximité, promouvoir l'individu en lieu et place de Christian de masse attractif en fait grappiller sur un système de formation rénovée oui, monsieur le ministre, et vous le savez l'attractivité passe par la revalorisation des traitements, évidemment, ce ne fut jamais le seul considérant qu'il a fait choisir ce métier, mais comme l'a dit notre excellent rapporteur Jacques Grosperrin, on ne peut sous-estimer le sentiment de déclassement social des professeurs de France ainsi : est-il acceptable que leur salaire Net moyen, soit 1000 euros inférieur au traitement moyen donc fonctionnaire de catégorie A hors Éducation nationale certes on constate ces dernières années une réelle volonté de revalorisation, je pense au protocole PPCR pour lequel près de 400 millions d'euros sont inscrits au budget 2000 Vert je pense également à la proportion plus grande de promo sur leur classe à la casse au niveau assez exceptionnel ou encore aux heures supplémentaires défiscalisées je ne sous-estime donc pas l'effort fait je connais aussi les effets de masse sur le budget de l'État pour les coureurs les plus nombreuses de la fonction publique, il n'en demeure pas moins qu'il n'y aura pas d'attractivité nouvelles s'il n'y a pas de revalorisation mais au-delà et pour y arriver, il faut réfléchir à l'individu les des parcours avec Françoise Laborde, nous avions proposé dans notre rapport, le recours aux contrats de mission, le système éducatif gagnerait des professeurs expérimentés et des équipes stables, là où les besoins se font sentir et les professeurs, eux, aurait ou l'ancienneté ne serait pas le seul critère majeur de la mobilité et de la promotion comme vous la si fort bien dit Gérard Longuet au début, d'autres travaux, mais pour cela il faut davantage rompre avec l'indifférenciation des postes à pourvoir et des profits, c'est ainsi que le métier, c'est ce qui ira dans la logique des jeunes générations qui n'entre plus dans la carrière pour la vie, ans de tôt ou tard un métier dont il tire une expérience qu'qui pourront valoriser ailleurs penser le professeur du XXIe siècle, c'est également souhaité un professeur, mieux formés, c'est pour vous ne priorité pour nous aussi, avec la loi pour une école de la confiance, vous voulez mieux assurer la formation des professeurs centré sur les apprentissages fondamentaux et vous avez raison, vous réfléchissez à mieux articuler formation initiale et prérecrutement et nous vous accompagnons formation initiale et formation continue et c'est la clé, formation continue et rendez-vous de carrière ou souhaitez d'ailleurs relancé cette formation continue au travers d'un nouveau schéma directeur mais il reste que dans le même temps, j'allais dire en même temps vous laisser stagner les crédits dans le second degré, vous voulez laisser même baissé de 3 avec 47 pourcent enfin penser le professeur du XXIe siècle, c'est penser aussi une profession débarrassé de toute différenciation de salaire entre les femmes et les hommes, et elle est encore de 13 pourcent en faveur des hommes et le fait que les femmes soient plus nombreuses en proportion dans le 1er degré n'explique pas tout, puisque parmi les professeurs des écoles, le salaire Net des hommes demeurent supérieurs de hausse pourcent à celui des femmes, or la mission éducative est par essence une affaire de femmes et d'hommes, de femmes et d'hommes, soutenus par la société confortés par leur ministre et respectées par les élèves et les parents l'actualité tragique de ces derniers mois montre que ce n'est hélas pas encore le cas, le recul des inscriptions au concours cette année, souligne au contraire le chemin qui reste à parcourir, pourtant mieux formés, mieux payés davantage écoutés quant à leurs aspirations individuelles au service de leur mission, les professeurs du fait unième siècle seront alors mieux à même de répondre aux défis de notre école, donc vous savez Monsieur le Ministre, qui sont largement les défis de notre société, je crois, Monsieur le Ministre, que nous partageons cette ambition et vous ne ménageait pas votre peine et si mon groupe votera les crédits de la mission dans le prolongement des propos de Gérard Longuet, je regrette que ce budget ne soit pas encore celui où l'on pourra dater l'émergence progressive de cadre rénové pour renouer avec l'attractivité du métier de professeur pour merci. Si la parole est à Madame Françoise. Pour 7 minutes. Madame la présidente, madame la présidente de la commission, messieurs les rapporteurs, monsieur le Ministre, mes chers collègues, cela a été dit par beaucoup d'orateurs précédemment, ce projet de loi de finances pour 2020 voix les crédits de la mission enseignement scolaire s'élever à plus de 74 milliards d'euros en autorisations d'engagement, un constat : les dépenses en faveur de la mission, anciennement scolaire qui est le 1er poste de dépenses de l'État progresse cette année encore de près de 2 pourcent par rapport à la loi de finances précédente, un budget en hausse de 1,37 milliard la dynamique budgétaire de cette mission demeure principalement portée par l'évolution des rémunérations de personnel, soulignant que c'est près d'un 1000000 de personnes qui sont concernées, représentant ainsi 92 pourcent de la somme dont nous débattons aujourd'hui ces dépenses sont à la hausse et ce pour 2 raisons principales : la reprise du protocole, parcours professionnels carrières et rémunérations et ce, pour plus de 304 millions d'euros et également la revalorisation de l'indemnité de suggestions des agents en grève plus après une première revalorisation lors de l'année scolaire 2018, 2019 une nouvelle revalorisation a été annoncé pour l'année 2019, 2020, d'un montant de près de 1000 euros elle est budgété à hauteur de 58,6 millions d'euros, enfin je voudrais noter la création des 440 postes supplémentaires alors que nous sommes dans un contexte de baisse démographique ce qui s'est traduit, en particulier pour le soutien à l'école rurale, en outre, les priorités politiques s'inscrivent dans une certaine continuité et elles sont pertinentes, cette continuité il font dans la saluer la soutenir, je pense évidemment, et surtout au soutien apporté au 1er degré mais aussi à une série d'initiatives je mettrais entre guillemets à vocation sociale qui permettent d'accompagner mieux l'ensemble des élèves vers la réussite qu'il mérite ainsi le programme 140 relatif à l'enseignement public primaire connaît une nouvelle fois une augmentation, pourquoi pas la poursuite du dédoublement des classes de CP, CE1 dans les établissements, classé réseau d'éducation prioritaire REP et REP plus et par l'obligation de l'instruction des 3 ans que nous avons voté ici au 1er semestre et qui porte un impact budgétaire supplémentaire estimée à 117 millions d'euros, 2 mesures qui visent en particulier à aider les enfants qui sont issus des milieux les plus fragiles, le programme 141 consacré à l'enseignement public secondaires représente quant à lui 33 pourcent des l'augmentation des crédits, ce sont les montants de dépenses de personnels qui sont en hausse par rapport à la loi de finances initiale de pour 2019, l'augmentation de plus de 290 millions d'euros du programme 230 pour la vie de l'élève traduit principalement la priorité du gouvernement en faveur de l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap depuis la rentrée 2012, 2013, les mesures d'accompagnement sont en augmentation de près de 50 pourcent et ce sont 3 milliards d'euros qui y sont consacrés, certes du chemin reste à parcourir, je pense en particulier aux soucis que nous devons apporter au recrutement et à la formation de ces AESH 4000 de plus sont prévus pour la rentrée 2020, espérons que cela répondra à la grande attente des parents et, justement, de leurs enfants, cette priorité, nous la soutenons bien sûr ici et je crois sur tous les bancs, en conclusion, je voudrais rappeler que l'augmentation en valeur des crédits de paiement par rapport à 2019 constitue la 3ème plus importante du du budget général après l'émission, défense et Solidarité, insertion et égalité des chances, je partage par ailleurs entièrement les propos tenus par mon collègue Antoine Karam sur le programme relatif à l'enseignement agricole, nous soutenons la hausse du budget dédié la volonté d'accompagner l'effort de communication et de valorisation de ces établissements que je pourrais qualifier d'excellence au niveau local, de même que nous nous félicitons du rapprochement opéré entre le ministère de l'Éducation nationale et celui de l'agriculture. Pour les années futures, le président de la République a annoncé à l'issue du grand débat national de grandes mesures, la limitation du nombre d'élèves par classe à 24 élèves en grande section, CP, CE1, sur l'ensemble du territoire d'ici la rentrée 2022 ainsi que le dédoublement des classes de grande section de maternelle en REP et REP, plus 2 annonces fortes mais aussi d'autres chantiers sont là face à nous, il conviendra de les faire avancer mon prédécesseur Max Brisson un peu rêver autour de de cet enseignant du XXIe siècle et je crois que nous avons plusieurs justement où un chantier à ouvrir le statut du directeur d'école, son rôle, sa mission, la redéfinition du métier d'enseignant et son évolution avec bien évidemment à la clé : sa revalorisation mais aussi ce grand chantier dont on parle depuis des années l'orientation afin afin que cette orientation ne s'assimile pas à une assignation pour les élèves dans des formations qui n'ont pas véritablement choisi. Conserver la priorité à l'école primaire et celle accordée aux élèves les plus en difficulté est essentiel si nous voulons construire cette école de la réussite pour toutes et tous pour cette raison et votre volonté affichée très fortement, bien évidemment, mon veau mon groupe votera en faveur des crédits dans le cadre de ce projet de loi de finances pour 2020 pour une école de la réussite, accessible à tous.

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur, les rapporteurs, madame la présidente de commission, mes chers collègues, au moment d'examiner son plus gros postes budgétaires, avec ses quelque 74 milliards d'euros en légère hausse de 1,8 je mesure avec vous l'engagement de l'État a former les nouvelles générations à investir pour proposer un enseignement de qualité qui correspondent aux attentes de nos concitoyens in fine et à dessiner tout simplement l'avenir de notre pays. Monsieur le ministre je considère très sincèrement que certaines de vos orientations vont indéniablement dans le bon sens et comme plusieurs de mes collègues qui m'ont précédé, je veux les saluer. Dès votre arrivée au ministère de l'Éducation nationale, vous avez annoncé votre choix de donner la priorité au 1er degré j'approuve ce cap, le cap que vous fixez sur ce point avec une attention particulière sur l'acquisition des savoirs et savoir-être fondamentaux, lire, écrire, compter et respecter autrui. Mais on est souvent tenté de donner à l'école d'tas de nouvelles missions forcément toutes plus vertueuse les unes que les autres, mais compte tenu du temps non extensible dont dispose à la fois nos enseignants et leurs élèves, je suis pour ma part convaincu qu'il faut se concentrer sur l'enseignement de discipline qui permettront à l'enfant d'acquérir un socle de connaissances indispensables à sa construction et plus tard à sa vie d'adulte. La poursuite du dédoublement des classes de CP et de CE1 en zone prioritaire Rep et Rep plus va là aussi dans le bon sens est une bonne chose, tant le dispositif fait actuellement ses preuves, c'est évidemment un effort financier important, mais les dividendes seront précieux dans quelques années. même le plafonnement à 24 élèves par classe de grande section de CP et de CE1 à l'horizon 2022 est aussi une bonne mesure puisqu'elle favorise un enseignement plus personnalisé et donc plus efficace pour les élèves. Cependant, sur ces 2 points, nous serons très sont particulièrement vigilants sur les moyens tant humains que matériels qui seront mis en place pour assurer cette réforme, le dédoublement combinée au plafonnement pose la question du bâti scolaire et des investissements que vont devoir réaliser bon nombre de communes pour accompagner ces décisions gouvernementales. Vous avez indiqué en commission, monsieur le Ministre, que le processus pourra connaître des ajustements au fur et à mesure de son déploiement. Dans la logique qui commande paie l'État doit aller beaucoup plus loin en garantissant aux communes qu'il ne s'agit pas comme nous avons pu le le regretté par le le passé d'une charge nouvelle non compenser tout en maintenant, sur les communes l'taux de la règle de Cahors. Soyez assuré qu'avec mes collègues de la commission culture, nous suivrons cela avec la plus grande attention. Le sujet compensation financière se pose aussi en ce qui concerne l'obligation d'instruction dès l'âge de 3 ans. Contenu dans la loi, école de la confiance comme vous avez pu l'entendre régulièrement ce sujet indique inquiète particulièrement mes collègues de tous bords confondus d'ailleurs. En réponse à nos questions lors de votre audition en commission, vous avez évoqué l'évolution démographique pour atténuer le surcoût que représente l'abaissement de l'âge obligatoire. Permettez-moi de vous dire que cela ne nous a pas vraiment assuré : nous attendons encore des réponses précises et chiffrées sur la compensation aux collectivités. Ici, au Sénat, nous sommes le relais de l'inquiétude des maires, des élus locaux, et vous êtes en quelque sorte que le ministre-le dernier relayeur. C'est dire à quel point l'issue de cette course aux compensations financières dépend de votre capacité à tenir le bâton jusqu'au bout en résistant aux concurrents et néanmoins ami, qui figure dans les autres couloirs de la piste tortueuse que constitue ce projet de loi de finances 2020 nous comptons sur vous, mais je voudrais pour terminer aborder un autre sujet qui relève également de votre ministère. Lors de l'audition en commission, cette semaine, votre collègue de Madame la ministre des Sports a suggéré un travail collaboratif pour faire en sorte que le sport et toute sa place au sein de notre système éducatif. Facteur d'équilibre physique et psychologique, porteur de valeurs indémodable, la pratique d'une activité sportive fait partie à mon sens de ces fondamentaux qu'il faut inculquer à tous les enfants. Madame Maracineanu a évoqué dans un monde certes quelque peu idéal de solides partenariats qui pourrait voir le jour entre les associations sportives locales et l'éducation nationale pour affermir l'éducation physique et sportive, dans le 1er degré. Cela pourrait prendre la forme par exemple de semaine thématique dans des classes dédoublées, prise en charge en partie par ces associations. Sincèrement je souscris pleinement et avec enthousiasme à cette démarche, mais j'attire tout de même votre attention sur un point de vigilance, les bénévoles des associations sportives locales, associations, qui ont par ailleurs souvent bien du mal à se financer, ne doivent pas être mobilisés pour pallier les manques de l'Éducation nationale aussi, j'aimerais connaître votre ambition en la matière, ambition qui donc vous avez compris évidemment être accompagnée d'un dispositif budgétaire à la hauteur, je vous remercie. Merci, la parole est à Madame Maryvonne Blondin. Pour 5 minutes chers collègues. Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, Gaston Jays, écrivait en 1922 le budget est essentiellement un acte politique, alors que nous révèle le donc les crédits de la mission enseignement scolaire sur le projet de société du gouvernement pour notre jeunesse, vous nous soumettez monsieur le ministre : un budget en augmentation d'un milliard d'euros, et avait déclaré : un pays qui a confiance dans son avenir investit massivement dans son école, si nous ne pouvons que saluer cette augmentation et l'ambition qu'elle entend porter, permettez-moi de modérer votre enthousiasme depuis plusieurs mois, les personnels enseignants ont attiré votre attention sur la dégradation de leurs conditions de travail leur désarroi face aux souffrances de leurs collègues et élèves et les difficultés avec leur hiérarchie, vous vous félicitez d'une sanctuarisation du nombre de postes, vous prenez 440 postes dans le second degré et je rappelle qu'il y a eu près de 6000 suppressions d'depuis 2018 dans ces mêmes établissements qui doivent faire face à la réforme d'ampleur du lycée et dont les effectifs sont en augmentation, vous lirez au 1er degré mais l'extension des dédoublements nécessitera de plus en plus effectif et le pool de rentes de remplacement est déjà épuisé vous rappeler que 80 pourcent de la hausse budgétaire sera dédié à la masse salariale, témoignant de l'effort sans précédent que le ministère voudrait ainsi assez personnel, qu'en est-il réellement environ 500 millions sont destinés à financer le gvt, ainsi qu'à l'application du PPCR que vous aviez précédemment repoussé d'un an, le doublement des primes en aurait plus ne concerne qu'une partie des enseignants, alors même que d'autres exercent dans des territoires aux caractéristiques similaires, les heures supplémentaires sont régulièrement présenté comme une mesure à la faveur du pouvoir d'achat, travailler plus pour gagner plus est-ce cela la conception ministériel de la revalorisation des carrières dans le contexte actuel nous sommes loin de l'école bienveillante, un poste de médecin de prévention pour 16000 et lors du CHSCT extraordinaire du 6 novembre dernier, le ministère a présenté pour la première fois, je reconnais le nombre d'enseignants ayant mis fin à leurs jours 58 de de 2018 à 2019, et déjà 11 pour la rentrée mais aucun poste supplémentaire n'budgétés pour 2020, vous nous répondez que cet état de fait procès de des difficultés de recrutement réels auxquels vous savez confrontés, mais vous ne pourrez restaurer l'attractivité de la médecine de province de prévention comme de la médecine scolaire qu'garantissant à assez personnels omissions cruciales la considération qu'il mérite le programme vide, l'élève est en hausse de 29 millions et recouvre de multiples actions mais là aussi, aucun poste de médecin scolaire de CPE, d'assistantes sociales, de psychologues supplémentaires n'est budgétée et les conventions peinent à se mettre en place à l'heure où les inégalités se creusent l'éducation nationale est un acteur incontournable d'une prévention durable et nous nous devons d'enrayer les déterminismes sociaux ne serait-ce qu'en matière de santé dès l'école, de plus, nous ne pouvons que déplorer la baisse drastique des fonds sociaux divisé par, par 2, vous évoquez une mesure de sincérité financière plutôt que de lutter, lutter contre le non-recours à ces aides financières, alors même que vous plaidez pour davantage de justice sociale, enfin plus de 330000 élèves en situation de handicap, un chiffre en hausse sont l'équipe dans l'école dite ordinaire en 2018, 2019 si l'on peut se féliciter de cette politique en faveur d'une école toujours plus inclusive, si 4000 AESH supplémentaires ont été recrutés à la rentrée, de nombreuses familles restent encore sans solution d'accompagnement, la Générale des pial sans réelles évaluations préalables et difficile à se mettre en place dans sur le territoire national, l'inclusion, monsieur le ministre ne se réduit pas à un simple vocale communicationnel, elle nécessite un investissement conséquent en terme de formation et de rémunération afin d'assurer un suivi à la mesure des besoins, monsieur le ministre, votre budget est habilement présenté, mais hélas, le défi est colossal, c'est pourquoi mon collègue l'a dit, nous ne voterons pas votre budget. Merci, la parole est à madame Annick Billon. Pour 3 minutes. Madame la présidente, monsieur le midi c'est mes chers collègues, en cette journée de mobilisation du monde agricole, je souhaite renouveler mon soutien à tous les agriculteurs et toutes les agricultrices traité de l'enseignement agricole, c'est avant tout s'enquérir de l'agriculture de demain, c'est pourquoi nous ne pouvons que nous féliciter de la volonté du gouvernement d'augmenter les crédits du programme enseignement technique agricole cette filière d'excellence garante d'une culture et d'un élevage respectueux de la nature et des attentes des consommateurs pour autant la filière peinent à attirer de nouveaux élèves cette voie d'orientation est souvent peu connu et mal considérés pour les établissements publics agricoles, le nombre d'élèves et d'étudiants en 2017 a atteint son plus bas niveau depuis 96 avec moins de 100000 inscrits, la rentrée 2019 vous heureusement une hausse de 750 élèves par rapport à 2018 ce fléchissement doit être soutenue par des formations, intégrant la révolution technologique du monde agricole, il est donc indispensable de donner la possibilité aux étudiants issus des filières agricoles de choisir parmi un panel plus large de discipline en proposant des enseignements tels que les sciences économiques et sociales, le numérique et sciences de informatique ou encore l'agro-écologie par ailleurs la suppression des aides fléchés pour les TPE, vers les 10 diplômes post-bac est une mesure inquiétante quand on sait qu'aujourd'hui le diplôme le plus recherché de la filière agricole est le BTS analyse conduite et stratégie de l'entreprise agricole dans la mesure où il permet l'embauche de salariés hautement qualifiés cette suppression risque de pénaliser une profession qui cherche pourtant à monter en compétences, enfin je souhaiterais évoquer la situation préoccupante des accompagnements, des accompagnants, de handicap AESH dans l'enseignement agricole : l'enseignement agricole est particulièrement inclusif et il faut le saluer cependant sur le terrain des retards perdurent dans l'affectation aux jeunes d'un accompagnant. les salaires peu élevés, leur statut précaire, l'absence de formation encore et les déplacements répétés conduisent en effet à des difficultés de pérennisation des personnels, à titre d'illustration, nous comptons en Vendée, déjà 40 8 démission depuis la rentrée, j'en profite également pour évoquer la question des sommes attribuées aux assistants d'éducation dans le rôle d'encadrement durant le temps périscolaire est essentiel, alors que la rémunération de ses assistants a été revalorisée dans l'enseignement scolaire pour 2020, ce n'est le pas le cas pour ceux issus de l'enseignement agricole, le différentiel s'élève aujourd'hui à 1411 euros, il est essentiel, monsieur le Ministre de pallier cette disparité, ce faisant, le budget consacré à l'enseignement agricole en hausse de 0,5 pourcent est encourageant et c'est la raison pour laquelle le groupe Union centriste votera l'adoption des crédits du groupe programme enseignement technique agricole, je vous remercie et j'ai tenu presque dans les. Merci, la parole est à madame Nicole Duranton. Pour 4 minutes chers collègues. Madame Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, messieurs les rapporteurs, chers collègues, en préambule, permettez-moi de citer la harangue que faisait Jules Ferry, dans un discours devant les directeurs d'école en juin 1889 messieurs, ce que nous vous demandons à tous c'est de nous faire des hommes avant de nous faire des grammes rien la mission ancienne enseignement scolaire représentant 22 pourcent du budget général est une mission cruciale puisqu'il s'agit là de l'éducation de nos enfants, il faut vraiment la prendre au sens 1er du mot mission car de son succès dépend celui de beaucoup d'autres, dont l'avenir de la France, en effet, si la compréhension des valeurs républicaines se fait tout au long de la vie, c'est bien à l'école que se forment des qualités essentielles à l'intégration de ces valeurs, ses qualités sont la rigueur morale, le respect d'autrui et de la loi, l'amour du savoir, l'esprit critique, la curiosité intellectuelle, je constate que les dépenses en faveur de cette mission, progresse de 2 par rapport à la loi de finances initiale de 2019 avec 74 1 milliard d'euros de crédits demandés pour 2020 en août lorsque l'on s'attarde sur cette hausse, on s'aperçoit qu'elle n'abondent pas que des projets d'avenir nécessaire à la modernisation de l'acte d'enseigner et de l'acte d'apprendre en réalité 92 pourcent de la hausse des crédits de la mission provient de celle des dépenses de personnel de 68,7 milliards d'euros avec l'injection de 304 millions d'euros dans la reprise du protocole, parcours professionnels carrières et rémunérations et la revalorisation de l'indemnité de sujétion des agents aurait toutefois, il faut noter que les plafonds d'emplois prévus sont négatifs, ce qui est un signe de bonne volonté dans la gestion du déficit, encore faut-il équitablement et efficacement répartir ces employes en améliorant également les conditions d'exercice des métiers consolidant l'action de l'enseignant, il s'agit notamment des accompagnants des élèves en situation de handicap A. E. S H, fonction créée en 2005 suite à la réforme handicap et inclusion scolaire si l'ouverture au service civique en 2018 est louable, il faut noter la précarité de certains contrats avec 6 ans de CDD requis pour obtenir un CDI par ailleurs aujourd'hui les primes Rep et Rep plus sont versés au corps enseignant par le ministère, mais les AESH pourtant essentiels au fonctionnement scolaire est confrontée aux mêmes situations difficiles ne sont pas concernés le rouvrir ce droit et étendre leur cadre de travail à l'accompagnement périscolaire chose actuellement possible uniquement sur dérogation municipale méritent également réflexion cela représentera forcément un coût pour l'État, le rapport pour avis numéro 145 fait au nom de la commission de la culture s'intéresse à ce titre à 2 problématiques d'actualité, je salue le travail effectué par mon collègue Jacques Grosperrin qui s'est intéressé à la rémunération des enseignants et aussi mon collègue Antoine Karam, qui a étudié l'inclusivité de l'enseignement agricole, ils ont été évalués la cohérence des objectifs tracés par le gouvernement et des moyens mis en oeuvre pour les réaliser, le dédoublement des classes en primaire et dans les grandes sections maternelles vont dans le bon sens, il faut soutenir le 1er degré avec 2 34 pourcent de progression par rapport à 2019 réformer le second degré, avec 1,35 pourcent de plus et mettre l'accent sur le programme 230 Vie de l'élève avec 5,11 pourcent d'augmentation dans son programme l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap représente 220 millions d'euros sur 290 tout cela est une équation sensible qui doit donc s'inscrire, s'écrire, pardon, sur un double dénominateur commun l'inclusion de tous les élèves et l'attractivité des métiers éducatifs, il faudra demeurer vigilant lors de la mise en oeuvre et de ce budget et surtout produire les efforts d'attractivité d'attractivité pour redonner envie à nos jeunes d'enseigner, ce qui ne passe pas seulement par des mesures budgétaires, je vous remercie. Merci, la parole est à monsieur Jean Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Vous disposez de vingt minutes Monsieur le Ministre. Madame la présidente, madame la présidente de la commission sur la rapporteur général, messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les sénateurs, le budget de l'enseignement scolaire que je présente aujourd'hui devant vous, traduit la priorité accordée à l'éducation par le président de la République et par le gouvernement. C'est un budget de confirmation de nos engagements, vous l'avez noté vous êtes plusieurs à l'avoir noté qui prolonge la loi pour l'école de la confiance que vous avez voté cet été et que j'ai présenté devant vous encore récemment ce budget permet la mise en oeuvre effective de nos réformes dont l'ambition est claire la réussite de tous les élèves et selon un sillon on, on qui fait que je pense que l'on peut dire qu'il y a une cohérence que certains d'entre vous ont noté entre ce budget les précédents Budgets, le budget de la mission enseignement scolaire qui vous est proposé pour 2020, s'établit à 52 ans 1 milliard d'euros hors cotisations aux pensions de l'État, cela représente une augmentation de près de 2 c'est-à-dire plus d'un milliard d'euros supplémentaires, il m'a semblé entend dans les discours que l'Inde est l'une des sénatrice a dit que c'était inférieur à l'inflation, l'inflation prévue autour de 1 pourcent c'est une augmentation de 2 pourcent donc je pense que nous pouvons en déduire autre chose que ce qui a été dit, avec un milliard d'euros supplémentaires, nous poursuivons la transformation profonde du système éducatif. Parce que ce budget réaffirme l'ambition pour l'école primaire qui doit conduire à la maîtrise par tous les élèves des savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, respecter autrui si nous réussissons cela nous le réussissons non seulement pour l'école primaire, mais évidemment pour l'enseignement secondaire, ne l'oublions jamais la qualité de la formation des élèves lorsqu'ils arrivent en classe de 6ème est absolument essentielle pour l'enseignement secondaire, l'effort en faveur du 1er degré et la première de mes priorités parce que c'est une priorité, en soi, pour les raisons que d'ailleurs le président de la commission, a bien voulu rappeler, je l'en remercie le sénateur Gérard Longuet, mais aussi parce que c'est une priorité logique et enfin parce que c'est une priorité de compensation n'oublions pas que la France a fait le choix ou le non-choix là pris la pente fatale pendant plusieurs décennies de dépenser plus que les pays de lancer l'OCDE pour son enseignement secondaire et moins que les pays de l'OCDE pour son école primaire, cela n'a strictement aucun sens d'un point de vue rationnel comme les années précédentes. Créations de postes sont prévues dans le 1er degré 440 postes supplémentaires sont créés. Alors même que nous sommes dans un contexte de baisse démographique, il y a 50000 élèves en moins à la rentrée 2020 à l'école primaire ce double effet nous permet d'assurer les différentes mesures que vous avez bien voulu rappeler puisque nous avons à la fois moins d'élèves plus de postes, ce qui nous permet donc d'améliorer le taux d'encadrement à chaque rentrée scolaire, tout au long du quinquennat et donc à la rentrée 2020, comme à chaque rentrée, autre rentrée dans chaque département de France, qu'il soit à dominante rurale ou à dominante urbaine, ce pur ce budget poursuit donc l'une des mesures. Sûr de justice sociale, les plus importantes du gouvernement, notamment la réduction du nombre d'élèves. Dans les classes où se jouent les bases de l'apprentissage, c'est-à-dire notamment l'école maternelle, le CP et le CE1, nous consolidons le dédoublement des classes de CP et de CE1 en REP et en REP, plus 300000 élèves sont concernés, c'est aujourd'hui 20 pourcent d'une classe d'âge,

comme vous le savez, les évaluations de CP et de CE1 qui sont arrivés maintenant leur 3ème édition il y a une forme de pleine maturité nous permettent de mesurer ce qui s'est passé, notamment pour les élèves de CP de l'année précédente, elle nous permet aussi de voir les différences entre Ray près plus et reste du territoire, comme vous le savez aussi l'enjeu qui est un enjeu d'ailleurs qu'on trouverait dans dans d'autres pays, c'est de réussir à en finir avec cette différence, constate table entre eux, c'est 20 pourcent de territoires défavorisés et le reste de la France, hé bien oui mesdames et messieurs les sénateurs, les premières évaluations nous montre, non pas que nous en finissons avec cet écart, c'est un objectif qui prendra plusieurs années mais nous avons diminué cet écart et je vous renvoie au document que j'ai publié il y a environ 3 semaines à la suite de ces, de ces évaluations, c'est quelque chose qui doit tous nous réjouir, parce que c'est un défi commun a pratiquement tous les pays et ce défi pour l'instant n'a été relevée par personne le fait que nous réussissions à être sur le bon chemin en la matière, à quelque chose de décisif qui, bien entendu, correspond à un effort qui doit être poursuivi, je pense que ça justifie pleinement le fait d'y consacrer les moyens qui vous sont présentées dans ce budget, l'objectif est même d'aller plus loin, le président de la République l'a dit dans sa conférence de presse de sortie du grand débat, nous voulons vous le savez. Aussi les grandes sections de maternelle en éducation prioritaire. nous aurons à la fin du quinquennat non plus seulement 300000 élèves concernés, mais 450000 c'est-à-dire 3 générations de 150000 élèves en limitant aussi progressivement à 24 élèves par classe, à partir de la rentrée scolaire 2020 les effectifs de grande section. Et en suivant ensuite ceux de CP et de CE1, nous voulons aussi avoir une mesure pour l'ensemble de la France. Avec des effets qui sont immédiats, ensuite nous accueillerons aussi. Au travers de cette rentrée 2020, 26000 élèves supplémentaires du fait de l'instruction obligatoire à 3 ans, c'est 26000 élèves supplémentaires, c'est 26000 en plus alors qu'il y a 50000 élèves en moins, ce qui devrait faire honte au manque de 24000 élèves en moins, au lieu de 50000 élèves ont je le rappelle, pour bien que ce qu'il soit clair pour chacun que les effets démographiques évidemment contribue aussi à l'accompagnement de ces mesures, c'est un budget qui accompagne tous les élèves vers la réussite, le volume d'enseignement du second degré public sera maintenue en 2020, vous l'avez noté, soit pour le saluer, soit pour le critiquer, mais il y a en effet une augmentation du volume des heures supplémentaires dans ce budget, ce volume d'heures supplémentaires permet de maintenir un taux d'encadrement équivalent dans le second degré, il permet aussi, notamment pour les professeurs qui le souhaitent le plus et ils existent, je les rencontre sur le terrain de bénéficier d'une augmentation de leur pouvoir d'achat en rappelant aussi que ces heures supplémentaires sont défiscalisées en vertu des mesures annoncées par le président de la République en décembre dernier, ce qui, clairement, représentent des mesures de soutien du pouvoir d'achat des professeurs, bien sûr, je ne prétends pas que ces mesures sont suffisantes en elles-mêmes, mais elles font partie de ce paysage de revalorisation, ce budget renforce aussi le soutien aux élèves les plus fragiles, fragilité sociale, avec une augmentation de 5 pourcent des moyens alloués en faveur des bourses de collège et de lycée, là aussi, cette augmentation des bourses, c'est un point très important, qui je crois doit être souligné il n'y aura pas de baisse des fonds sociaux, contrairement à ce que j'ai pu entendre, je m'en étais expliqué en commission, je le redis, nous avons pris comme référence les fonds utilisés effectivement en 2018 et en 2019, et à ce titre, les fonds dépensés. En

le seul moyen d'action sociale que nous avons, il y a les bourses dont je viens de parler il y a aussi les projets, comme les cités éducative que nous concevons avec le ministère de la ville et qui nous permettent d'aller plus loin sur le plan social et d'une manière qui correspond à des à des projets puisque ce sont des projets. Sociaux sur les territoires qui vont accompagner la réussite scolaire, c'est à souligner, il y a 80. Cité éducative que nous avons annoncé avec Julien Denormandie, et qui représentent une efficacité sociale pour agir sur les facteurs sociaux de la réussite scolaire. En 2020 le le ministère au travers de ce budget consacrera plus de 3 milliards d'euros par an à l'accompagnement des élèves en situation de handicap, cela représente depuis 2017, une hausse de 44 C'est évidemment considérable, il n'y a pas d'autres domaines sur lesquels nous pouvons trouver une augmentation comparable, mais cette en termes d'organisation, un budget qui permet ainsi le déploiement de 3000 pôles inclusifs d'accompagnement localisé des et ses pial, là aussi, contrairement à ce que j'ai pu entendre représente un bon qualitatif extrêmement important parce qu'il permet d'avoir une organisation de notre système depuis le terrain et ce, non pas pour faire des économies puisque je viens de le dire, nous avons 40 d'augmentation en 2 ans de notre budget, mais tout simplement pour que nos moyens soient plus directement au service de nos fins, c'est pourquoi nous avons réussi des réussites déjà en cette rentrée 2019 nous avons divisé par 2 le nombre d'élèves sans solution ne sont passés de 8 pourcent à 4 pourcent et ce chiffre va encore baisser au cours des prochains mois et Madame la sénatrice, je crois qu'en Seine-Maritime, à ma connaissance, les problèmes sont résolus et mais je veux bien continuer à à regarder ce qu'il en est la loi crée également un service de gestion dédiée aux accompagnants et ce budget 2020 des. Précarise les personnels par l'achèvement de la transformation des contrats aidés. En contrats d'AESH souhaite que chacun mesure le chemin parcouru, il y a à peine plus de 2 ans, il n'y avait pratiquement que des contrats aidés pour accompagner les élèves handicapés et tout le monde se plaignait à juste titre de la du caractère trop précaire de ses statuts d'un compagnon, un peu plus de 2 ans plus tard, presque tous les et les accompagnants ne sont plus contre et son âme, et par-dessus le marché il y a plus d'un donc personne ne peut prétendre que dans ce domaine-là, nous avons régressé non, nous avons amélioré le système, et nous l'avons amélioré, non seulement quantitativement mais qualitativement, bien sûr, il reste des insuffisances, bien sûr, il y a des imperfections mais le chemin pris est clairement un chemin à la hauteur de la priorité qui a été fixée et nous avons évidemment ont visé cette ce principe que les AESH soit pleinement considéré comme membre du système scolaire avec de véritables carrières de véritable formation et une possibilité de s'inscrire dans la durée, dans le système éducatif, c'est un service meilleur qui est rendu aux élèves et à leurs familles par les mesures que nous avons prises et à la rentrée 2019. Et pour la rentrée 2020 la rentrée 2020 sera également celle de l'aboutissement de la refonte du Baccalauréat et des programmes du lycée, cela doit permettre à tous de ça. Approprier progressivement cette réforme, nous allons de ce fait, avoir un lycée général et technologique qui, au cours de l'année 2020, 2021 arrivera l'aboutissement de la réforme du Baccalauréat, tandis que la voie professionnelle continuera, elle aussi, ça ça sa mutation, c'est un budget qui. Coeur de renforcer l'attractivité du métier de professeur, mais aussi de l'ensemble des personnels concourant à nos missions d'éducation et je remercie l'ensemble de. Sénateur qui, à cette tribune, ont marqué leur intérêt pour cette question qui a en effet été essentielle, comment nous pouvons réussir et là aussi c'est un dessin défis commun à tous les pays à rendre pleinement attractive cette mission de professeur au 21ième siècle, je crois que c'est le chemin que nous prenons, mais qui bien entendu se situe dans la durée, d'abord par l'approche qualitative que nous avons du métier de professeur, c'est la réforme de la formation des professeurs qui vous a été présenté au type de la loi pour l'école de la confiance et plus généralement les 10. à des pratiques que nous avons sur les évolutions du métier de professeur au XXIe siècle, non seulement pour sa mission, qui évoluent, qui s'enrichit. Mais aussi pour ses conditions de travail, qui doivent se caractériser par un meilleur appui social, meilleures conditions de santé, meilleures conditions de sécurité plus généralement un bien-être au travail, dont les premiers éléments se voient en cette rentrée 2000 19 et vont s'accentuer à la faveur du budget 2020, je pense notamment à la gestion des ressources humaines de proximité qui est déjà une réalité pour une partie de nos professeurs et qui signifie que nous avons de véritables conseiller à la disposition des professeurs à moins de 20 minutes de leur lieu de travail dans une partie de la France aujourd'hui dans la totalité de la France, demain c'est cette vision beaucoup plus personnalisée de la carrière du professeur qui est en effet une des grandes pistes d'amélioration, nous avons aussi sanctuariser le schéma d'emplois du ministère, je crois que c'est un point important, il a été souligné par plusieurs d'entre vous, je crois que nous avons désormais une maturité du débat sur l'enseignement, qui doit nous permettent de considérer que, avec environ un 1000000 de personnel pour 12 millions d'élèves, nous avons en réalité un ratio qui qui correspond à ce dont le pays a besoin, la question est beaucoup plus désormais sur notre façon de nous organiser de façon d'utiliser nos heures notre force de travail au service des élèves et je serais heureux que nos débats successifs, que ce soit pour la loi pour l'école de la confiance ou pour les discussions budgétaires nous permettent de comprendre qu'au fond, le sujet n'est plus la création globale ou la suppression globale de postes, sujet qui a pu parfois opposé la gauche et la droite, mais au contraire à partir d'un nombre suffisant de postes et si nous nous comparons aux autres pays, nous avons ce nombre aujourd'hui nous réussissons en l'affectant aux dans le 1er degré ou dans le second degré, selon les analyses que nous faisons et je vous en ai proposé une en ayant une vision de l'organisation des missions, hé bien nous réussissions à partir de ce de cette ce nombre de professeurs déjà importants et dont il faut rappeler que si nous le faisons trop bouger à la hausse, hé bien ça nous crée autant de difficultés pour valoriser ce pouvoir d'achat que nous voulons valoriser hé bien comment ce schéma d'emplois donc sanctuarisé nous permet tout simplement d'avoir une vision qualitative de l'évolution de nos. Au système scolaire, nous arrivons aussi à une stabilisation des emplois administratifs du ministère et je suis, j'assume. Complètement cela parce que je pense qu'il faut aussi contrecarrer un vieux cliché au sujet de l'Éducation nationale, non l'éducation nationale n'est pas sûr administrée cette quelque chose qu'il faut avoir bien l'esprit, je l'ai dit à la commission des finances de l'Assemblée, je l'ai dit aussi ici au Sénat en commission, je le redis maintenant parce que je pense que dans nos raisonnements, nous devons bien voir que le ratio de personnel administratif par rapport au personnel, professeur au est un ratio qu'on ne trouverait pas dans la plupart des structures publiques et privées de grande taille comme l'éducation nationale et nous avons besoin justement d'avoir un encadrement de qualité. C'est un débat que nous pouvons avoir très au delà de cette discussion budgétaire. Sur le milliard de hausse de ce budget, ce sont aussi essentiellement les crédits de masse salariale qui font l'objet d'un abondement Net de 823 millions d'euros, là aussi vous êtes plusieurs à la. Voir noté mais cela représente donc 80 pourcent de l'augmentation générale et même un peu plus qui vont bénéficier au personnel du ministère, et donc vont constituer des augmenter. Si on du pouvoir d'achat pour moitié cette hausse résulte. Principalement de la progression naturelle du déroulement des carrières, cela représente donc 300 millions d'euros. Pour l'autre moitié 400 millions d'euros, cette augmentation se traduira dans des mesures catégorielles pérenne, c'est la revalorisation des carrières au titre du protocole, parcours professionnels carrières et rémunérations : le PPCR 300 millions d'euros, 60 millions d'euros pour la troisième revalorisation des personnels exerçant. et une enveloppe indemnitaire de 30 millions d'euros pour accompagner les mesures. De ressources humaines de l'agenda social, par exemple, en améliorant le taux d'accès à leurs classes, des professeurs, des Échos. Plusieurs d'entre vous ont parlé de l'enseignement agricole et je les en remercie, c'est l'occasion pour moi de dire que je tiens toujours des discours très positifs sur l'enseignement agricole, je l'ai encore fait au salon de l'éducation, samedi dernier tout simplement à ce que je crois en effet aux vertus de l'enseignement agricole et à tout ce qu'il nous propose comme perspective, c'est pourquoi nous parlons de façon et de l'enseignement agricole en collège comme nous parlons de l'enseignement professionnel de l'apprentissage de l'enseignement général de l'enseignement technologique dans les mêmes termes, avec la même dignité c'est ce qui a permis d'avoir de premiers résultats parce que, soulignons-le, il y a 750 élèves de plus qui ont choisi l'enseignement agricole en cette rentrée, alors même que nous constatations depuis de nombreuses rentrer une diminution du nombre d'élèves dans l'enseignement agricole, certains pourraient comparer ce chiffre avec les évolutions budgétaires d'enseignement agricole et ça a été fait à cette tribune, il y a un instant, je voudrais dire que l'enseignement agricole et sans sans parler à la place de de mon collègue Didier Guillaume, l'enseignement agricole à des places vacantes et que donc c'est un bon usage de nos moyens éducation que d'envoyer dans d'excellents lycées agricoles plus d'élèves, où il y a des places je crois que nous faisons d'une Pierre plusieurs coups : en faisant cela, et que c'est bon aussi bien sûr pour le futur de notre agriculture, bon vous avez souligné les enjeux de transition actuellement qui passe en effet par la modernité et la qualité de notre enseignement agricole que j'ai plaisir à souligner, voilà donc, mesdames et messieurs les sénateurs, les grandes lignes de ce budget cette un budget au service de projets, c'est un budget au service d'objectifs qualitatifs qui sont explicitées ces objectifs bien sûr sont à à discuter démocratiquement, c'est ce que nous faisons, je crois pouvoir dire qu'ils ont un sens, la priorité à l'école primaire et donc le socle de la suite de tout le parcours de tous nos élèves, mais aussi l'évolution de la qualité de vie au travail de nos professeurs et donc nos personnels, parce que cela conditionne aussi la réussite de nos élèves, c'est donc un projet qui de budget qui est cohérent avec les objectifs que nous nous sommes fixés aussi au travers de la loi pour l'école de la confiance et donc je vous remercie pour le soutien que vous voudrez bien accorder à ce budget. Merci, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous allons procéder à l'examen des amendements portant sur les crédits de la mission enseignement scolaire figurant à l'état B article à l'article 38 un amendement 155 c'est madame brûlant qui va nous présenter. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, c'est un amendement qui vise à compenser véritablement je dirais l'obligation scolaire qui est désormais à 3 ans une mesure, vous le rappelez souvent et vous avez raison, qui avait été adopté ici-même à l'unanimité, mais qui ne doit pas à nos yeux et aux yeux de nos collègues élus, notamment dans les communes, prendre un goût amer et pour cela il faut compenser totalement cette obligation scolaire à 3 ans puisque un certain nombre de communes faisaient déjà en sorte de scolariser les enfants à 3 ans auparavant que d'autres compenser en partie au moins, les dépenses dans l'enseignement privé et que du coup ça crée 2 poids 2 mesures entre les communes. Puisque toutes ne sont pas compensés à hauteur de la dépense tout ça dans un contexte que je rappelle très brièvement, compte tenu de leur tardive mais où le dédoublement des classes pèse aussi ce sont de nouvelles charges pour les communes où des réformes fiscales risque d'aggraver la situation financière de nos communes et où, pour les plus grandes d'entre elles ou ces dépenses sont encadrés par la fameuse règle de Cahors et enfin, il nous semble que compenser est une question tout simplement d'égalité car si la République décident de scolariser ses enfants, à 3 ans, alors elle doit faire en sorte qu'ils le soient dans les meilleures conditions et je dirais quel que soit le territoire où ils sont scolarisés et en l'occurrence pas au détriment d'autres activités éducatives qui sont initiées par les communes, ce qui peut être le cas, compte tenu des difficultés financières qu'elles peuvent être amenés à connaître vu cette non-compensation. Merci, monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission sur cet amendement. Madame la présidente, la commission n'est pas favorable à cet amendement, considérant que la l'article 17 de la loi sur l'école de la confiance, a mis en place la compensation par conséquence, cette demande est déjà satisfaite et on nous arrêterons là, à cet instant, parce que je ne saurais pas aller plus profond dans cet examen, de peur d'alourdir le débat. Monsieur le Ministre, quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement. Merci madame la présidente, alors j'ai j'hésite entre la peur d'alourdir le débat à mon tour et et et la volonté quand même de de dire quelques mots, parce que ça a été abordé à plusieurs reprises ce sujet : nous en avons beaucoup débattu à l'occasion de la loi pour l'école de la confiance, le Conseil constitutionnel a un peu trancher certaines des choses qui souhaitait dit à ce moment-là, ce qui nous permet d'avoir ce débat une à une autre étape, puisque comme vous le savez il a validé les modalités d'accompagnement que nous avons retenus et ses modalités d'accompagnement rappelons quand même qu'elles sont là, les conséquences de règles juridiques essentiellement et que nous avons sur ce sujet-là était finalement dans un cadre assez, assez, fixé par le droit, ce qu'il faut ce qu'il faut rappeler d'abord que c'est que c'est dans le budget 2021 que l'on verra les véritables conséquences budgétaires puisque c'est ex Post comme vous le savez, que nous ferons les les compensations les crédits nécessaires sont autour de 100 millions d'euros, rappelons que c'est et pour l'enseignement public et pour l'enseignement privé hein je j'entends parfois qu'c'est que pour l'enseignement privé, ça n'est pas ça n'est pas exact seront inscrits sur les programmes 139 pour l'enseignement privé et 140 pour l'enseignement public, on s'interroge parfois sur le ce qui se passera pour les communes qui dépensent des gens qui ont déjà fait le choix et ce que vous avez dit de payer dans le passé pour leurs écoles maternelles, donc comme vous le savez le ces ces communes dans la mesure où elles dépensaient déjà et dans la mesure où le nouveau système est un système qui tient compte de la différence d'une année sur l'autre, donc de la différence de l'année 2019, 2020 comparé à l'année 2018, 2019 ces communes ce ne sont a priori pas remboursé, sauf, je tiens quand même à donner ces 2 éléments-là, sauf s'il y a une hausse des dépenses obligatoires, donc incluant maternelle plus élémentaire et ce, malgré la baisse de la démographie, donc dans la plupart des cas, la baisse de la démographie fait qu'il n'y aura pas cette hausse de la dépense obligatoire mais on peut imaginer que maternelle plus élémentaire dans une commune, conduisent à une hausse des dépenses obligatoires et si cette condition est remplie, il faut que la hausse soit liée à la scolarisation des enfants de 3 à 6 ans,

perd de l'argent dans la nouvelle configuration quand il y a une hausse des dépenses, il y a une un remboursement du Delta, c'est pour ces raisons que j'aimais à mon tour un avis défavorable à votre amendement. S'il n'y a pas de demande d'explication de vote, je vais mettre aux voix l'amendement 155 avec 2 avis défavorables qui est pour son adoption. Il n'est pas Il n'est pas adopté. à présent, 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune le 88. Ratifier c'est. Madame De Lattre qui va nous Madame Laborde, pardonnez-moi, Françoise Laborde. Il y a pas de soucis, madame la présidente, c'est en effet l'amendement de ma collègue Nathalie Delattre qui trouvait embêtant que l'on supprime 450 postes dans le second degré et qui donc s'est dit que, au lieu donc supprimer 440 il fallait en créé 1500 parce qu'elle a été alerté par un certain nombre de syndicats qui lui ont fait remarquer que dans beaucoup de lycées et d'établissement même collège il n'y avait pas de professeur d'éducation physique, alors que l'on a un plan développement pour lutter contre la sédentarisation et l'obésité, j'en profite, madame la présidente, pour défendre le mien puisque moi je me contentais de revenir sur la suppression de 440 postes de l'enseignement donc scolaire public du second degré et je n'avais pas d'idées pour l'affecter je laissais le ministre de l'Éducation nationale désaffecté où il lui semblait nécessaire, je vous remercie. Merci madame Laborde, monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements. Défavorable la commission estime que les moyens humains sont suffisants à condition qu'il soit bien géré, ce qui est certainement le cas. Monsieur le Ministre, quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements. Même avis même un président. Je vais mettre aux voix l'amendement 88 rectifié avec 2 avis défavorables qui est pour son adoption.

Il n'est pas adopté. 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune le 103 rectifié, c'est toujours Madame Laborde. Emmanuel santé ce sera très rapide, comme je l'ai dit en discussion générale alors que la pauvreté ne cesse de progresser en France, il n'était pas souhaitable pour moi et certains membres de mon groupe, de voir les fonds sociaux des établissements diminuer drastiquement de moitié, bien sûr, peut-être qu'ils ne sont pas consommés, mais ils ne sont pas consommés parce qu'ils ne sont pas connues et s'ils ne sont pas connus, ils ne seront pas consommés, je vous remercie. Merci madame sénatrice le 110 et monsieur Magnier, qui va nous le présenter. Oui, cet amendement revient à ce qui vient d'être présenté par ma collègue Françoise Laborde et je je rajouterai que l'argument du gouvernement selon lequel la baisse de ces fonds se justifierait, au vu de la non-consommation des crédits ne tient pas, nous pensons que cette non-consommation au lieu de servir de caution à une baisse des crédits devrait au contraire inciter le gouvernement à réfléchir sur le pourquoi de cette non-consommation à l'heure où de nombreuses familles vivent dans des conditions précaires, voire sous le seuil de la pauvreté, les difficultés alimentaires parfois de certains élèves dans nos établissements scolaires que nous connaissons, dont nous parlons souvent mais est-ce que ces familles sont sous toujours informés de leurs droits, est ont été mis en place, relativement récemment mais qui aujourd'hui pourrait être mieux utilisé. Si monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements. Madame la présidente de la commission est défavorable à ces deux amendements constatant en effet par un objectif de sincérité qu'il n'appartient au ministère de montrer que ces crédits et là ce ne sont pas utilisés et que les chefs d'établissement soit doit prendre des initiatives soient restituées cet argent au ministère, manifestement il y a aujourd'hui des reliquats inutilisés qui rentre. enfin est fictif et j'. Que nous souhaitons, c'est la réalité de la dépense, il a les demandes augmentent évidemment il faudra rétablir les fonds sociaux des établissements naturel pour répondre à une exigences identifiées, ce qui n'est pas le cas cet instant. Merci, Monsieur le Ministre, quel est l'avis du gouvernement. Merci madame la présidente, en matière sociale il y a les mots et puis il y a les actes et je voudrais, à la fois préciser ce que j'ai dit à la tribune tout à l'heure et puis vous donner quelques chiffres, donc ce sera les chiffres et les lettres

en 2018, que nous avons dépensé 39 donc c'est ce 39, qu'il faut comparer à 27 et ce que nous nous proposons de dépenser l'année prochaine, c'est 40. Alors je sais que je vais entend pendant des mois, enfin sauf si j'ai réussi à vous convainc maintenant parce que je vais essayer de faire, mais je vais entendent pendant des mois que les fonds sociaux ont diminué, que le gouvernement est antisocial etc et donc ce qui feront ça s'opère en 2 mots parce que la réalité, c'est celle que je viens de dire là, c'est 27 millions d'euros en moyenne pendant les 5 années de la part du gouvernement que vous avez soutenu un peu plus que celui-ci, et donc là cette fois-ci, ça va être 40 dont 40 est supérieur à 27 et comme ce n'est pas la première fois que je le dis, je crains que ça n'est pas la dernière, mais l'honnêteté intellectuelle commande de dire ce que je suis en train de dire, et par dessus le marché, ça aussi, n'est pas l'ensemble de l'action sociale, il y a bien d'autres choses, vous venez d'évoquer la cantine, nous avons pris et d'ailleurs ça a été évoqué tout à l'heure, les mesures de petits déjeuners gratuits qui sont en train de réussir dans les quartiers qui ont qui en ont besoin et aussi d'ailleurs, il faut effectivement nous devons progresser en milieu rural, sur ce point le dès le déjeuner, un Euro qui est pertinent dans certains cas, pas dans d'autres, là où les mairies font déjà beaucoup et je veux saluer cela ceci s'ajoute à l'augmentation des bourses de 5 je prends au mot ce que vous dites, c'est-à-dire je reviendrai devant vous, certainement à d'autres occasions, bien entendu, et on pourra regarder l'action sociale, éducative, on ajoutera ce qu'on fait aussi des cités éducatifs, ce qu'on fait, déboursent ce qu'on ne fait aussi de l'éducation prioritaire, ce que nous faisons, otites, des fonds sociaux la réalité de ce qui est fait sur le plan social apparaîtra de façon éclatante, je suis extrêmement confiant sur ce point parce que, en effet, nous y consacrons plus de moyens, simplement, un : nous ne nous payons pas de mots, de nous sommes sincères sur les chiffres et 3 nous raisonnons par objectifs, pour être efficace sur le plan social, c'est quand on raisonne trop par sur le plan social, on est peu efficace, si cette sinon on aurait eu de meilleurs résultats en matière d'inégalités au cours des années passées, on ne ce n'était pas sous la responsabilité de ce gouvernement. Il n'est pas adopté l'amendement 110 avec 2 avis défavorables qui est pour son adoption. Qui est contre, il n'est pas adopté. Nous examinons l'amendement 153 c'est madame brûlant qui va nous le présenter. Merci madame la présidente, il s'agit par cet amendement de créer davantage d'unité Ulysse pour se rapprocher de ce que préconise le rapport conjoint des inspections générales des affaires sociales et de l'éducation nationale qui préconise la création de 240 unités chaque année pour répondre aux besoins également de se rapprocher d'un d'une centaine d'élèves, encadrés par les enseignants référents alors qu'on est aujourd'hui beaucoup plus proche de 174 enfants voir bien au-delà dans certains départements, je ne reviens pas sur le cas de la Seine-Maritime et enfin. D'améliorer les moyens de la médecine scolaire, qui est évidemment aussi décisive dans le suivi et le dépistage du handicap, tout cela pour aller d'un pas un peu plus rapide et déterminé vers l'école inclusive que nous appelons tous de nos voeux. Merci, quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. La à la Commission ne partagent naturellement la préoccupation de notre collègue, mais considère que les efforts accomplis effectivement par le gouvernement tant depuis 2 ans, en ce qui concerne le l'inclusion des élèves en situation de handicap et fort et doit être prise en considération, il faut en mesurer l'impact, nous avons là. la transformation en CDI de plus de 6400 postes d'un SH, ce qui est important et ce qui permet à ces général personne plus jeune de pouvoir bâtir leur leur carrière envisager un effort plus continue et, par ailleurs, ont été créés au service des parents des pôles inclusifs d'accompagnement localisé qui permettent aux parents d'enfants handicapés de bénéficier d'un soutien et d'une prise en charge avant même la scolarisation et tout au long de la scolarisation et donc la commission des finances, a estimé qu'il fallait donner toutes leurs chances à ces initiatives et faire confiance au gouvernement dans sa prise en charge d'une politique d'inclusion qui est unanimement soutenu mais qui est désormais mis en forme avec une réalisme du quotidien. Quel est l'avis du Gouvernement, monsieur le ministre. Merci madame la présidente, le comme j'ai pu le dire à la tribune tout à l'heure, il y a une hausse de 237 millions d'euros dans le budget 2020 pour les actions notamment de recrutement des à message et c'est ce qui nous va nous faire dépasser en 2020, plus des 3 milliards d'euros dans le budget de la mission enseignement scolaire pour l'école inclusive, s'agissant de la médecine scolaire, comme vous le savez, la principale difficulté n'est pas une difficulté budgétaire mais une difficulté de recrutement et donc si je reconnais bien volontiers que nous avons de grands progrès à faire, ce n'est pas en travers d'une telle mesure budgétaire que nous pourrions progresser je profite aussi de, de, de votre question, pour préciser un point pour lequel j'ai été interpellé tout à l'heure à la tribune, c'est-à-dire dire que oui conformément à d'ailleurs à ce qui a été votée dans la loi pour l'école de la confiance, chaque élève en Ulysse compte comme un comme dans notre système scolaire, donc pour toutes les raisons précédente que j'ai évoqués, je suis défavorable à à cet amendement. Je vais mettre aux voix cet amendement 153 avec 2 avis défavorables qui est pour son adoption. Qui est contre, il n'est pas adopté. L'amendement 47 rectifié c'est madame Moret Richaud, qui va nous le présent. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement d'appel vise à attirer l'attention du gouvernement sur la participation d'acteurs extérieurs à l'éducation nationale au service public de l'enseignement, notamment sur les sujets mémoriel à titre d'exemple, avec plusieurs de mes collègues, j'ai eu récemment l'occasion de me rendre au mémorial de la Shoah à Paris cette institution joue un rôle majeur dans l'enseignement d'un pan important de notre histoire en intervenant auprès d'élèves et d'enseignants, j'ai été surprise d'apprendre que, alors que les actions éducatives et de formation représente près de la moitié des dépenses de cet organisme Swat près de 8 millions d'euros, il ne perçoit que 3 millions d'euros de fonds publics, État, collectivités, etc, soit environ 20 pourcent de ses recettes si l'éducation nationale peut s'appuyer sur des partenaires pour concourir à ces missions, c'est à elle dans ma suite, mais l'écoute le présent amendement propose donc de transférer 5 millions d'euros de l'action, pilotage et mise en oeuvre des politiques éducatives du programme 214 vers l'action 6 actions éducatives complémentaires aux enseignements du programme 230 qui, aux termes du projet annuel de performance vise à faire de l'école, un espace de socialisation et de respect d'autrui, d'apprentissage et de responsabilité et de la citoyenneté. Merci, quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. la commission souhaite connaître l'avis du gouvernement, pourquoi, parce que il y a en faveur du Mémorial de la Shoah, une action dans une mission gouvernementale. N'intervention qui est assez modeste, je le reconnais bien volontiers, mais nous avons et c'est l'élu du Grand-Est que je suis qui qui s'expriment à cet instant la responsabilité sur l'ensemble de notre territoire de d'assez d'assez nombreux et d'acier et de très légitime, institutions, de mémoire, madame la présidente, je pense au musée d'le mémorial de l'annexion autour du Struthof je pense naturellement Mémorial de Verdun, je pense à ce qui a été fait par notre par le monsieur le maire de Meaux sur la première guerre mondiale à la fin, le musée de la paix à Caen et et il y a une question de principe, l'éducation nationale peut-il peut-elle pardon, prendre en charge d'une façon significative ces fonctionnement ce qu'elle ne fait pas à cet instant, alors je je souhaiterais connaître le point de vue du ministre et et en réalité plutôt le point de vue du gouvernement sur une action qui est nécessairement collective, même si, comme vous l'avez dit très justement Madame l'éducation des jeunes générations et sans doute la meilleure façon de leur donner une compréhension exacte de l'histoire de notre pays de de s'efforce de ses faiblesses, de ses pages de gloire et de ses pages plus difficile et plus sombres. Monsieur le Ministre, quel est l'avis du gouvernement. Madame la présidente, d'abord je vous remercie de nous cet amendement et de et et des propos qui l'accompagnent, puisque, comme vous l'avez dit, c'est un amendement d'appel et c'est donc, comme nous y invite le président Longuet à l'occasion de, de, de faire le point sur un sujet qui est encore plus qualitative, je dirais, et pédagogique que que budgétaire et je ne dis pas ça pour m'exonérer des des conséquences budgétaires des politiques mémorielles mais il y a évidemment un sujet de programmes et je crois que, aussi bien la façon dont ont été recomposé les programmes de lycées que tout un chacun peut peut voir que ceux qui accompagne les nos programmes de l'école primaire et du collège font largement droit à cette à cette dimension mémorielle que soit au type de l'histoire ou au titre de l'éducation civique et morale, il y a évidemment beaucoup de sujets qui progresse sur ces questions, certains ne correspondent pas à des coûts lorsque nous arrivons à la systématicité d'une présence des élèves le 8 mai le 11 novembre devant les monuments aux morts, nous il n'y a pas de coup particulier, il y a ensuite des efforts spécifiques que nous faisons, il se trouve que vous avez cité le Mémorial de la Shoah, c'est évidemment un très bon exemple, hein, c'est un de nos principaux partenaires, j'ai les chiffres sous les yeux, notre soutien est passé de 150000 euros à 200000 euros en 2000 19 et devrait passer à 250000 l'an prochain, donc c'est une progression en en pourcentage qui est assez remarquable et au-delà des enjeux budgétaires, je ne vois fréquemment les responsables de du mémorial encore récemment et je crois que il y a plein de satisfactions de part et d'autre, a, à ce qui se passe, notamment, notre capacité à ce qui est de plus en plus d'élèves concernés par par l'action du Mémorial de la Shoah par l'ensemble des initiatives que nous prenons à ce titre, j'étais plusieurs fois d'ailleurs sur le terrain, j'en profite de la pour le dire parce qu'on souligne souvent le fait que le enfin, les problèmes de transmission de la mémoire de la Shoah, ces problèmes sont bien réelles, je les regarde en face, mais ils ne doivent pas nous masquer que nous réussissons de belles choses aussi en la matière grâce justement au travail qui existe entre le Mémorial de la Shoah et et le ministère de l'Éducation nationale, la question évoquée par le président Longuet à l'instant, c'est-à-dire le fait que évidemment les données budgétaires en la matière ne relève pas que du ministère de l'Éducation nationale, mais aussi du ministère des armées et ainsi que du ministère de la culture, ainsi que des collectivités locales, et je crois que si nous croisons l'ensemble des données budgétaires, nous voyons qu'il y a un bel effort qui est fait par l'ensemble des des pouvoirs publics que nous progressons sur bien des sujets comme le concours national de la Résistance et de la déportation qui me maintenant depuis cette année mobilise plus de 40000 candidats, je ne vais pas vous citer l'ensemble des des concours et actions qui sont développés, mais elles sont nombreuses, et je pense qu'on peut dire qu'il y a une certaine vitalité de cette politique politique de, de, de la mémoire et encore tout récemment, nous l'avons vu avec le monument, inauguré par le président de la République pour rendre hommage à nos soldats morts en opérations extérieures, ce qui est malheureusement correspond à une activité à une actualité douloureuse aussi, mais qui montre bien que l'éducation nationale est pleinement engagée dans ce devoir que nous avons vis-à-vis de ceux qui nous ont précédés. L'avis est donc défavorable. Oui, monsieur le rapporteur, je vous en prie. Je dirais à à mon excellent collègue madame Moret Richaud que un retrait serait bienvenu, l'appel a été entendu, oui je plutôt retraite défavorable, merci, je vous remercie. Nous poursuivons avec l'examen de 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune le 89 rectifié c'est Madame Mireille Jouve qui va nous le présente. Merci madame la présidente en l'espace d'une dizaine d'années, le nombre de médecins scolaires a été divisé par 2 dans le même temps, la liste des missions qui leur ont sont confiés s'est considérablement étoffée, ce sont aussi les médecins, les moins bien rémunérés de la fonction publique, il faut redonner à la médecine scolaire, le rôle qu'elle mérite un nombre croissant d'enfants du fait de difficultés économiques et sociales accrues au sein de leur famille et n'ont pas accès en dehors du milieu scolaire à une médecine préventive, cet amendement a pour objet d'attribuer 5 millions d'euros à l'axe sont santé scolaire afin de renforcer l'attractivité de la profession de médecin scolaire et le nombre de postes. Merci. Le second amendement le sang de rectifier si Madame Laborde, qui va nous présent. Alors c'est le même, mais nous n'avons pas cosigné l'un l'autre, en fait, parce que nous ne les retirions pas sur les mêmes lignes, donc ma collègue le prélevée sur les actions de communication et moi je le prélever sur l'enseignement scolaire privé mais c'est le même combat, c'est pour la médecine scolaire. Merci, monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements. La commission de me souhaite l'avis du gouvernement, car elle n'est pas d'une compétence totale sur la médecine scolaire, qui est un problème récurrent, ancien et apparemment sans véritable solution satisfaisante. Monsieur le Ministre, quel est l'avis du gouvernement. Merci madame la présidente, c'est un sujet structurelles sur lesquelles je reconnais bien volontiers, je l'ai fait tout à l'heure que la situation n'est pas satisfaisante, mais bien entendu dire cela ne doit pas nous exonérer de, de, de la prise de responsabilité sur sur ces questions, il faut bien le identifier le problème, je l'ai dit-il, la question n'est pas tant d'y consacrer plus de budget mais d'être capables de recruter sur des postes qui déjà sont vacants, et donc nous devons nous travailler sur l'ensemble des facteurs, c'est tout l'enjeu du travail que fait actuellement la ministre de la santé, notamment pour arriver à ce qu'il y ait plus de médecins dans les temps qui viennent, mais aussi pour que les postes de ministre de de médecins du travail soient plus attractif avec une véritable filière tout ceci ne nous a pas exonérer quand même de mesures favorables à l'attractivité de la médecine scolaire, je voudrais les mentionner, c'est la mise en Oeuvres du PPCR aussi pour les, pour les médecins de l'Éducation nationale, c'est la création au 1er septembre 2017, d'un 3ème grade hors classe culminant à la hors échelle B c'est l'amélioration du taux de promotion à la 1ère classe des médecins

tout ceci évidemment n'est pas n'est pas suffisant mais vous montre bien qu'il y a une action pour la valorisation de la médecine scolaire, les grandes solutions structurelles sont notamment par la collaboration entre médecine de ville et médecine scolaire c'est cela se traduit par exemple pour la visite médicale à 3 ans par le fait que nous allons beaucoup plus coopérer avec les PMI, entre les PMI et l'éducation nationale et donc cette un chemin de progrès qui est enclenchée, avec quelques mesures de court terme pour l'attractivité et des mesures dans la durée pour avoir plus de plus de médecins scolaires, donc pour toutes ces raisons, l'avis est défavorable. Monsieur le rapporteur. également défavorable. Je vais mettre aux voix l'amendement 89 rectifié avec 2 avis défavorables qui est pour son adoption. Il n'est pas Il n'est pas adopté l'amendement 100 de rectifier avec 2 avis défavorables qui est pour son adoption. Qui est contre, c'est le même vote il n'est pas adopté. à présent, 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune le 154 c'est monsieur Ouzoulias ce qui va nous présente. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, 2 amendements sur l'enseignement agricole porté par un sénateur d'un département qu'il est éminemment Les Hauts-de-Seine je crois que nous partageons tous le même intérêt collectif pour l'enseignement agricole, ça a été dit à multiples reprises et le fait que je sois sénateurs d'un département extrêmement urbanisé, dans lequel il y a pour tous, en tout et pour tout 2 vaches montre que l'enseignement agricole, c'est aussi l'affaire des citadins, parce que ça ne nous concerne directement notamment par notre alimentation et je pense que c'est un point, un point important, alors si les 2 amendements se situe finalement comme on peut les considérer comme la transposition sous forme d'amendement des 2 conclusions de notre rapporteur Monsieur Monsieur Karam, qui soulignait que, en effet, il n'était pas normal que dans le contexte actuel, il y ait une soixantaine de de postes qui soient supprimés, d'une part, je pense que c'est pas un encouragement pour pour les personnels et puis d'autre part, je crois que vous l'avez dit, monsieur le ministre, il y a la situation non résolue des assistants éducatifs qui sont sous la double tutelle la vôtre et celle du du ministère de de de l'agriculture et qui aujourd'hui ont un écart de rémunération qu'il faudrait résoudre complètement, il y a eu déjà des efforts de fait ce que vous nous proposons aujourd'hui, c'est de finir ce travail alors bien évidemment LOLF oblige, nous prenons cet argent sur 2 secteurs : l'enseignement privé, par la force des choses, et aussi les moyens informatiques de des établissements pour tenter de forcer les établissements à se passer des logiciels qu'ils achètent, d'utiliser des logiciels libres, il y a aussi une insistance de notre commission sur sur ce dernier point, merci. Merci, un amendement 86 rectifié c'est madame Jouve qui va nous le présente. Merci madame la présidente, qu'il s'agit d'un amendement de ma collègue Nathalie Delattre, le schéma d'emploi pluri-pluriannuel sur la période 2019, 2022 prévoit une réduction de 60 équivalents temps plein en 2020 dans l'enseignement technique agricole dont 39 postes d'enseignants, or pour cette rentrée 2019, on constate une hausse de 750 élèves pourtant les diminutions d'emplois de professeurs auront des effets immédiats sur la qualité de l'enseignement délivré puisque l'enseignement agricole est une petite structure, c'est pourquoi cet amendement annule la suppression d'équivalents temps plein agricole, il vient en soutien aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole qui, du fait d'un manque de visibilité vis-à-vis de l'éducation nationale et des conséquences de la réforme du Baccalauréat tentent de maintenir la qualité de la formation agricole public en France. Merci, monsieur le rapporteur, quelle est la ville de la commission sur ces deux amendements. L'avis de la commission consiste à demander l'avis du gouvernement et je vais vous expliquer pourquoi, à titre personnel, il se trouve que 2 rapporteurs sur 3 ont été président de conseil d'administration de lycée agricole, nous sommes donc très favorable à l'enseignement agricole en général et à l'enseignement public agricole en particulier, donc nous n'avons pas d'opposition de principe aux demandes qui ont été formulées par les auteurs d'amendements mais ne la commission n'a pas bénéficié de la part du ministère de l'Agriculture, ça ne vous concerne pas directement Monsieur le Ministre des informations suffisantes pour former son jugement et pour comprendre en particulier pourquoi cet enseignement qui est demandé sous sous ses 3 formes principales lycée public lycée privé maisons familiales rurales, pourquoi nous on n'a, on n'a pas eu l'explication de l'évolution des chiffres alors que nous sommes élus du territoire très conscients de l'utilité de cette filière qui est qui, autrefois, était une 2ème chance pour les non-agriculteurs et qui devient tout simplement une filière d'intégration dans la vie économique locale en partant naturellement de cette culture, agricole, rural et en allant progressivement vers l'ensemble des métiers, présent sur les territoires non métropolitains pour prendre une une formule que chacun ici pourra comprendre, or nous n'avons pas eu les réponses à nos questions des enseignants, des renseignements demandés ont été fournis par l'administration de l'agriculture, c'est donc pas la vôtre, je ne veux pas monter une administration contre une autre, mais on a vraiment l'impression ce cet ensemble au sur lequel comptent les familles, les milieux professionnels, les territoires, manque de considération de la part de l'administration centrale et je suis certain, monsieur le Ministre, que vous allez apaiser nos inquiétudes et c'est la raison pour laquelle nous vous interrogeons. Monsieur le Ministre, quel est l'avis du gouvernement. Merci madame la présidente, le j'ai commencé un petit peu à répondre par avance à cette question dans mes dans mes propos généraux, c'est-à-dire il y a d'abord un, premièrement, à rendre un hommage que je crois, chacun a rendu au lycée agricole, c'est vraiment l'occasion de le dire. Il joue un rôle extrêmement important et dire cela de la part du ministre de l'Éducation nationale ne va pas ça de soi que cela puisque parfois dans le passé, il y a pu il y avoir un esprit de compétition, disons, entre les 2 ministères, cela n'a aucun sens, je n'ai donc aucune difficulté à rendre hommage au lycée agricole et où est et aux maisons familiales rurales d'ailleurs de la même façon, joue un rôle extrêmement important et j'ai l'impression que tout le monde est d'accord avec cela et nous joignons là les actes aux paroles puisque ça s'est traduit notamment par une convention assez volontariste entre le ministre de l'Agriculture et moi-même, que nous avons présenté au salon de l'agriculture pour que notre système d'orientation soit plus volontariste au service des lycées agricoles et c'est ce qui permet ce rebond dont j'ai parlé de 750 élèves à la rentrée, dont on doit se réjouir et qui encore une fois inverse une tendance qui était lourde et continue depuis plusieurs années, donc ce rebond est positif, mais ce que l'on doit dire en même temps évidemment, je ne veux pas être trop rentrer dans trop de détails sur ce point parce que je ne veux pas non plus parler à la place du ministre de l'Agriculture, mais le fait est que les taux d'encadrement dans les lycées agricoles sont extrêmement favorables aujourd'hui et que ce que l'on pouvait regretter, c'était une forme de, d'anomie dans un certain nombre de cas par manque d'élèves donc aujourd'hui nous savons que le sujet n'est pas tant le taux d'encadrement au lycée agricole que notre capacité à y envoyer des élèves, correspondant à une bonne qualité d'enseignement qui est là et donc je crois que. Nous faisons d'une Pierre 2 coups, c'est-à-dire nous réussissons à ce qu'il y ait plus d'élèves,

encore une fois, c'est, c'est l'occasion de dire que nous soutenons les lycées agricoles qu'il y a derrière ça des enjeux de société, que le sénateur Ouzoulias ça parfaitement rappelé et et que nous en sommes très conscients, et que donc nous allons avancer de plus en plus la main dans la main, la réforme du Baccalauréat et d'ailleurs, une occasion de souligner cela, parce qu'il y a certains en en jeu d'environnement qui sont beaucoup plus explicites et qui parfois créeront des passerelles plus forte d'ailleurs entre l'enseignement agricole et l'enseignement général et technologique et professionnel, donc toutes ces raisons militent en ce sens de la valorisation de l'enseignement agricole, mais sans pour autant la l'amendement n'est pas pertinent pour aller dans ce sens, donc c'est pourquoi l'avis est défavorable. Monsieur le rapporteur. En demandant l'avis du gouvernement, la Commission avait l'intention de suive l'avis du gouvernement, et donc les est défavorable. Pour explication de vote. et que quand il s'agit par exemple de manipuler du bétail, il y a bien évidemment un taux d'encadrement qui doit être beaucoup plus élevé que dans les d'autres disciplines, donc c'est ce qu'il faut prendre en compte aussi c'est tout. S'il n'y a pas d'autres demandes d'explications de vote, je vais mettre aux voix l'amendement 154 avec 2 avis défavorables qui est pour son adoption. Il n'est Il n'est pas adopté l'amendement 86 rectifié mes bottes. Il n'est pas adopté. Un amendement 158 c'est monsieur Ouzoulias. Oui présenté également très rapidement, encore une fois, après la fermeture de de la section de Moissac, dans le Tarn et Garonne, il n'y a plus que, aujourd'hui, une seule Ulysse dans l'enseignement agricole public ce qui est bien évidemment absolument pas, pas possible, donc l'objectif de notre amendement s'est mobilisé davantage de crédits pour permettre la réouverture du lycée, dont on a absolument besoin, dans l'enseignement agricole public. Merci, quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Hélas pour les mêmes raisons, manque de renseignements réponse dilatoire et et partielle, nous sommes obligés d'interroger directement le le le ministre de lancer de la mission de l'enseignement scolaire ce soir. Monsieur le Ministre, quel est l'avis du gouvernement. monsieur le sénateur, on a de de nouveau l'illustration justement de l'intérêt d'une alliance forte entre le l'Éducation nationale et l'enseignement agricole, autrement dit ce que nous poursuivons comme objectif c'est un maillage du territoire national par des Ulis dans les établissements de l'Éducation nationale et donc, l'objectif est que tout élève puisse avoir une Ulysse.

pas qu'il ait peu d'Ulysse dans l'enseignement agricole ne signifie pas forcément qu'il n'y ait pas une logique d'école inclusive dans l'enseignement agricole, l'accompagnement par un un message pouvant évidemment se se se passer, c'est ce qui se réalise, donc c'est la coopération entre l'éducation nationale et l'enseignement agricole pour des cons, enjeux de de masse critique de l'enseignement agricole qui permet de compenser le problème que par ailleurs vous soulevez à juste titre, donc, pour ces raisons, l'avis est défavorable. Monsieur le rapporteur.

Il n'est pas adopté, nous allons procéder au vote des crédits de la mission enseignement scolaire figurant à l'état B je n'ai été saisi d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite je mais on voit les crédits de la mission qui est pour l'heure. qui est pour l'heure. Et sont adoptés. J'appelle en discussion : les articles 76 assez 76 obtiennent et les amendements portant articles additionnels qui sont rattachés pour leur examen au crédit de la mission enseignement scolaire à à l'article 76, cette pièce, nous avons un amendement de monsieur le rapporteur Gérard Longuet au nom de la commission des finances. Oui c'est c'est un amendement de de parlementaires de parlementaires, peut-être un peu ancien, peut-être un peu chevronnés, peut-être un peu routinier, attachés à un principe simple : c'est que le Parlement contrôle l'action du gouvernement, or nos collègues de l'Assemblée nationale ont introduit dans ce texte un amendement qui demande un rapport en général, on n'est pas très chaud pour les rapports mais on l'est encore moins nous ici au Sénat, lorsque ce rapport demandé porte sur des des questions sur lequel le Parlement a déjà travaillé et à exercer son activité de contrôle, en l'occurrence il s'agissait d'un un rapport sur les pardon sur les contractuels ah oui, c'était le serpent de mer de l'Éducation nationale sur les contractuels au sein du ministère de l'Éducation nationale, or si nos nos excellents collègues députés avaient regardé les travaux du Parlement dans son ensemble et notamment cette assemblée qui s'appelle le Sénat, il serait constaté qu'avec l'appui de la Cour des comptes nous avons assumé ce contrôle très récemment et présenté un rapport donc sur des turpitudes, il vaut mieux demander à turpitudes du gouvernement éventuelle, c'est-à-dire l'abus de l'utilisation des contractuels, il vaut mieux que le Parlement se saisisse lui-même plutôt qu'il confie à l'exécutif le soin de justifier ses propres Terres Titudes, au nom du principe que personne ici ne contestera Nemo Audi Propriano turpitudes idem allégeance et vive le Parlement qui a enfin le droit de parler chère présidente. Monsieur le Ministre, quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement. dire que j'avais émis un avis favorable donc, nonobstant les, les, les arguments que nous venons d'entendre tout simplement pour bien montrer que le gouvernement n'a rien à cacher sur un tas de sujets et que, en réalité, nous avons même de je pense des vues assez convergentes entre les différents parlementaires et et le gouvernement, c'est-à-dire que c'est un sujet qui doit être à la fois évidemment transparent et en même temps pour lequel on doit éviter toute forme de de dérapage, c'est évidemment la la ligne de conduite que que que je tiens donc cette mais néanmoins les arguments que nous venons d'entendre sont en effet juste, c'est pour ça que je dirais sagesse. Je vais mettre aux voix l'amendement numéro 15 de la commission avec un avis de sagesse du gouvernement qui est pour son adoption. qui est contre, il est adopté, je mais aux voix, l'article 76 quater, qui est pour son adoption. Qui est contre, il est adopté. pour l'examen de la mission Sport, jeunesse et vie associative du projet de loi de finances pour 2020 la séance est levée.